La séance est ouverte le compte-rendu intégral de la séance du jeudi 6 octobre a été publié sur le site internet du Sénat : il n'y a pas d'observation. Le procès verbal est adopté. L'ordre du jour appelle le scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République, mes chers collègues, il va être procédé dans les conditions prévues par l'article 86 bis du règlement au scrutin secret pour l'élection à la Cour de justice de la République ce. Scrutin se déroulera dans la salle des conférences et la séance ne sera pas suspendu durant les opérations de vote, je rappelle que la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être élu, une seule délégation de vote est admise par sénateur et je remercie nos collègues victoire Jasmin et Marie Mercier, secrétaire du Sénat qui vont superviser ce scrutin. Le juge à la Cour de justice de la République nouvellement élue sera immédiatement appelé à prêté serment devant le Sénat. Je déclare ouvert le scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République, il sera clos dans une demi-heure. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi d'orientation et de programmation. Du ministère de l'Intérieur, la procédure accélérée. Engagé sur ce texte et dans la discussion générale, la parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Monsieur le Ministre.

madame la présidente. Messieurs les rapporteurs, monsieur le président de la commission des lois, mesdames et messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de présenter devant vous au nom du gouvernement de la République, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, c'est un moment très important pour le ministère de l'Intérieur et l'ensemble des services qui concourent à la sécurité des Français sécurité avec un S sécurité au sens où nous l'entendons évidemment, sécurité, lutte contre la délinquance mais également sécurité civile. On a vu à quel point cet été, les Français étaient de plus en plus inquiets des difficultés qui pouvaient naître évidemment d'un mauvais modèle de sécurité civile sécurité Cyber, on voit bien à quel point l'actualité nous pousse à réfléchir à ces sujets très importants, sécurité et intérieure puisque nous avons aussi des dispositions messieurs les rapporteurs, vous l'avez constaté sur l'organisation territoriale de l'État, le rôle des préfets, des sous-préfets des agents préfecture dans l'action de ce ministère. Le hasard mais pas totalement le hasard veut que le calendrier de ce texte ici arrive en même temps que la loi de finances à l'Assemblée nationale, puisque cette loi de programmation prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires sur les 5 ans à venir, ces 15 milliards d'euros, la programmation de du texte de loi que nous vous présentons va de Pair avec la loi de programmation des finances publiques et la loi de finances pour pour l'année 2023 qui prévoit bien l'augmentation de ces 15 milliards d'euros si j'oserais dire : c'est une loi d'orientation qui est déjà concrète puisque le Parlement votera en même temps, les crédits, nous l'espérons, dans la chambre basse et demain je l'espère, dans la chambre. Pourquoi une loi de programmation du ministère de l'Intérieur, parce que nous avons considéré que les enjeux qui sont devant nous, qui sont devant le peuple français mérite comme pour nos amis militaires, une loi de programmation à une échelle assez longue, 5 ans, qui n'a jamais eu d'expériences précédentes dans l'annal du ministère de l'Intérieur, pourquoi, parce que, auparavant, il y a eu des Loppsi des lois d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure, il n'y a jamais eu de l'autre Lopmi pardon pour ce jeu de mot de programmation de l'ensemble du ministère de l'Intérieur. Et si les Loppsi précédentes ont permis de faire évoluer la pardon, la sécurité intérieure, la première, notamment en faisant venir l'image et la vidéosurveillance surveillance lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, la deuxième en revoyant la façon dont on organisé la sécurité publique, dans le cas de la RGPP lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République, le ministère de l'Intérieur n'a jamais connu sur 5 ans des programmations budgétaires importantes qui lui permet, non pas de répondre au problème, ici et maintenant est évidemment concerne chacune et chacun d'entre nous le ministère et le ministre de l'Intérieur en 1er lieu la délinquance au coin de la rue, le point de stup qu'on arrive pas à résorber la personne qu'il faut accueillir dans le commissariat, hé bien réfléchir à demain, c'est-à-dire aux crises de demain. mesdames et messieurs les sénateurs, je veux ici défendre le texte en évoquant les 5 crises auxquelles ce texte essaye de répondre en y mettant après ce constat, des stratégies et des moyens budgétaires. La première des crises qui est devant nous et qui est toujours persistante, c'est la crise terroriste. Je veux redire ici devant la Haute Assemblée que la menace terroriste est extrêmement prégnante sur le territoire national dans tout le monde et le monde occidental, en particulier, mais en France, bien évidemment, je ne reviendrai pas sur les causes de cette menace terroriste en France, elle a beaucoup de raisons. Oui. Mais nous devons constater que si nous avons déjoué, plus de 39 attentats depuis que le président de la République, il est président de la République, les informations qui nous parviennent les analyses de ce qui se passe dans d'autres pays. Et sans doute la prospective qui doit naître d'un grand ministère, au sud du ministère de l'Intérieur, évoque le fait que cette menace terroriste et d'autant plus prégnante qu'elle se modernise. Que se technologie peut être farfelue devant vous d'évoquer le fait que les attentats de demain. Ne seront pas simplement des attentats commis avec une arme dans une salle de spectacle ou avec un couteau en dehors d'une boulangerie, mais par un drone chargé d'explosifs qui pourrait foncé sur une foule et créer ainsi comme sur les théâtres d'opérations extérieures, la terreur comme nous la connaissons malheureusement sur d'autres armes dites plus traditionnelle. Et c'est le travail du ministère de l'Intérieur, que de prévoir l'acte terroriste de demain. Cet acte terroriste de demain, c'est notamment la façon dont la loi de programmation mais des moyens extrêmement importants. Pour pouvoir répondre à l'intervention des forces de police et de manière générale, de l'État alors que le ces réseaux radio par exemple, sont extrêmement. Monsieur le rapporteur, vous avez accepté que le gouvernement dépose en séance un amendement qui prévoit en dur, si j'ose dire l'ordonnance, ce qui était prévu pour le réseau radio du futur ces 2 milliards d'euros que nous vous demandons dans la programmation du ministère de l'Intérieur pour que demain l'ensemble des forces de sécurité, l'ensemble des administrations qui concourent à la sécurité des Français et un seul et unique réseau radio. Capable d'intervenir en images et en sons partout sur le territoire national et qui indépendamment. Des attaques, quelle qu'elle soit fonctionne et permet à la sécurité civile comme aux politique d'intervention type Red Berry ou gégène d'intervenir avec un seul réseau de communication. Des sociétés françaises ont gagné ce marché je peux désormais le rendre public, notamment la société Airbus qui fait partie de celle qui a gagné ce grand marché public que nous avons lancé que nous espérons concret avec la loi évidemment voter, il est évident que la crise terroriste de de ma fenêtre, évidemment, un travail d'anticipation, la lutte anti-drônes dont nous devons désormais nous prémunir mais également de communication, c'est le cas du réseau radio du futur. La 2ème crise, ce que je voudrais évoquer ici, c'est une crise d'ordre public. Chacun a pu constater, à la faveur de la crise des gilets jaunes que les manifestations de papa était terminé. C'est fini, du temps où les préfets ou le ministre de l'Intérieur se mettaient d'accord éventuellement avec les grandes organisations syndicales, avec un service d'ordre organisé et se mettaient d'accord sur les chemins, même s'il y avait plusieurs millions de personnes qui manifestaient, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, soutenons le, et finalement avec des policiers aguerris puisque l'ordre public est un métier qui n'est pas un métier fait par d'autres policiers que ceux qui sont formés à l'ordre public pouvait répondre à ces manifestations nombreuses sans qu'il y ait des débordements qui soit au-delà de l'acceptable chacun désormais a vu que les manifestations sont spontanés. Numérique difficilement chiffrable sans organisateur ou si peu. Peut déclarer avec bien évidemment une multiplicité de manifestations sur le territoire national. Alors qu'évidemment les villes moyennes ou les villes plus petites ne connaissait pas ce qu'ont connue tous les samedis, DJ, des jaunes, des années précédentes. L'une des difficultés de ces manifestations venait du fait que nous ayons un service de renseignement peut organiser, en tout cas peu organiser pour comprendre ces manifestations nouvelles qui touche d'ailleurs l'ensemble du monde occidental et pas simplement bien sûr la France. Et du nombre de policiers qu'il manquait spécialiste dans l'ordre public pour organiser ses manifestations. Je suis bien malheureux, obligé de constater que 15 escadrons de gendarmerie gendarmerie mobile et de CRS ont été supprimés ces 20 dernières années et lorsque la crise des gilets jaunes est venu les nombres de policiers spécialisés. Dans l'ordre public qui demande un entraînement qui demande un matériel qui demande un nombre et une stratégie particulière été. Peu nombreuses et ont parfois forcé des policiers, dont ce n'était pas le métier, on a parfois vu des policiers municipaux, utilisé par les mairies parce que il fallait bien répondre aux difficultés que nous connaissions des difficultés extrêmement grave pour les policiers eux-mêmes, bien évidemment, mais aussi pour les manifestants et le travail du ministre de l'Intérieur, c'est de permettre aux manifestants, même ceux qui manifestent contre la police, d'être en sécurité le paradoxe démocratique veut qu'il soit ainsi souligné. Prenant en compte cette difficulté d'ordre public, nouvelle et ces manifestations de nouvelles formules, nous vous proposons la recréation de onze. Escadrons de gendarmerie mobile ou de CRS, c'est la première fois dans l'histoire du ministère de l'Intérieur, donc depuis 25 ans, répartis en 7 escadrons de gendarmerie mobile 4 unités de CRS détruite mobile Mobile, on aura l'occasion d'en parler, monsieur le rapporteur, évidemment, sur cette nouvelle stratégie d'ordre public, je voudrais aussi souligner que le choix de recréer cette unité d'escadrons de gendarmerie mobile répond aussi à nos difficultés ultramarines pour vous savez que l'essentiel est gérée par des gendarmes mobiles et non pas par des CRS et qu'il s'agisse des événements potentiels en Nouvelle-Calédonie, des difficultés que nous connaissons à Mayotte et en Guyane, il faut aussi savoir regarder les choses telles qu'elles sont et il est fort à parier que, quel que soit le gouvernement quelle que soit la majorité des assemblées, le gouvernement de la République, la puissance publique aura besoin davantage d'escadrons de gendarmerie et de CRS pour répondre à la fois aux manifestations spontanées numérique et nouvelle et en même temps aux crises ultramarines que nous pouvons connaître. Il s'agit donc de professionnaliser l'Ordre public encore plus que nous avons fait jusqu'à présent, et de s'en donner les moyens et la recréation de ces escadrons à partir de ce constat mérite sans doute une loi de programmation, même si je veux ici souligner que pendant les 2 prochaines années budgétaires nous en créerons l'intégralité de c'est onze escadrons et CRS pour que nous soyons prêts également pour les Jeux olympiques qui est notre grand rendez-vous si j'ose dire et qui va rythmer cette loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Chris terroriste crise d'dans public, nous avons aussi à faire, sans aucun doute à une crise cyber. Mesdames, messieurs, sénateur, la prochaine pandémie que nous allons vivre et sans doute une pandémie cyber. Nous voyons bien les difficultés que tout le monde connaît des grandes entreprises, mais aussi des plus petites, dans chacune, et dans chacun des villages ou des villes que vous connaissez, qui sont vos Terres d'élection des collectivités publiques qui sont attaqués quasiment quotidiennement des hôpitaux publics à qui on demande des rançons et évidemment un certain nombre. Le fonctionnement régulier des service public qui sont évidemment à la. à porter d'attaque cyber, qu'il s'agisse d'un État étranger dans ce qu'on appelle désormais une guerre qui ne dit pas son nom. Ou de groupes terroristes ou du groupe de délinquants cyber qui peuvent ici dévoilé. Le secret de la correspondance l'a empêché le fonctionnement d'un service la demander des rançons qui se joue, qui se chiffrent parfois en milliards d'euros. Le ministère de l'Intérieur étant le ministère de la sécurité dans son côté curatif si dans son côté préventif doit être le ministère de la sécurité de demain. Qui est déjà la sécurité d'aujourd'hui. Mesdames, messieurs les sénateurs, savez-vous que plus de 50 % des escroqueries que vivent les Français sont déjà des attaques cyber. Quand une dame vient vous voir dans votre permanence pour expliquer qu'elle a reçu un mail de que ne connaît pas l'auteur et qui lui demande d'envoyer de l'argent, c'est déjà une attaque cyber. Quant à monsieur vient vous expliquer pour lui fait du chantage à sa messagerie personnelle, c'est une attaque cyber. Et ce qui vaut pour 50 % des escroqueries d'aujourd'hui, ils n'étaient que 15 % il y a encore 2 ans. Va atteindre les quasi 100 % dans les mois, années qui viennent. Songez mesdames, messieurs les sénateurs, que pendant les Jeux de Tokyo, qui pourtant n'ont pas fait venir beaucoup de public pandémie oblige 4 milliards d'attaque cyber. Ont été relevés, alors que nous connaissions encore à passer un peu lointain devant l'étendue désormais des attaques quotidiennes des grandes administrations, des grandes entreprises et il est fort à parier que la Coupe du monde de rugby, mais surtout des Jeux olympiques qui vont faire naître des dizaines sans doute de milliard d'attaque cyber. Soit sur l'organisation elle-même ou tout simplement combiné à une attaque terroriste, le scénario noir que je veux dessiner ici auquel il faut que nous nous préparions c'est à la fois une attaque terroriste par exemple par un drone, imaginons le cas pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, et en même temps une attaque cyber sur les hôpitaux qui prévoirait un plan blanc dans la région parisienne. Ce ne serait pas des dizaines ou des centaines de morts que nous viendrons à a constater mais peut être des milliers. Il faut évidemment nous préparer à cela et c'est pour cela que dans les 15 milliards d'euros que je viens solliciter en plus dans cette loi de programmation, plus de la moitié, 8 milliards sont consacrés. Au service numérique et cyber du ministère de l'Intérieur. Je veux ici donc souligner que c'est pour moi de 15 pour 100 de dépenses de personnel que je sollicite la haute assemblée dans ces crédits et que c'est essentiellement du matériel et pour plus de la moitié de ses crédits pour du cyber ou du numérique que je viens solliciter le vote de la haute assemblée afin que la voix, Numérique au cyber du policier et du gendarme aille aussi vite que la voiture numérique au cyber du voleur, je pense que c'est ce que c'est de faire tous les ministre de l'Intérieur, on cite beaucoup que les morceaux en ce moment au moins depuis Clémenceau, je crois que il faut que nous rendre compte que beaucoup de choses changent et que la police n'est pas tout à fait la même, parce que la délinquance, c'est pas tout à fait la même que depuis Clémenceau. 4ème crise après la crise terroriste que nous attendons, après la crise cyber après la crise d'ordre public, il s'agit évidemment d'une crise. De violence et notamment des atteintes aux personnes que nous voyons remonter continuellement. J'ai pu ce matin des délivrer les premiers chiffres de des violences constatées sur le territoire national et pour une fois qu'il baisse en réjouir notamment en agglomération parisienne ou des baisses à 2 chiffres sont constatées, mais il faut bien voir mesdames et messieurs que la crise de la violence qui touche l'ensemble des pays occidentaux vient de plusieurs raisons politiques sociétales, donc nous pouvons à à Longwy discourir mais aussi d'une crise de l'investigation dans la police nationale est un peu dans la gendarmerie nationale. Nous mettons depuis plusieurs années, beaucoup plus de personnes sur la voie publique. Les interpellations sont plus nombreuses plus 40 % de trafiquants de stupéfiants arrêté par exemple, mais une fois que nous avons mis plus de policiers, de gendarmes sur la voie publique, une fois que nous avons mis plus de moyens pour interpeller les personnes et il faut faire des enquêtes et des procédures judiciaires et pour ça il faut des personnes qualifiées comme telle. Et que nous disent les services de police et de gendarmerie. D'abord, qu'il n'y a pas assez d'OPJ. Les OPJ sont évidemment un maillon extrêmement l'essentiel pour que la procédure soit bonne afin que présenté devant un magistrat, les personnes peuvent être je 17 justement condamné. Et je veux dire ici que lorsque les personnes ne sont pas pour la société, parfois même pour les policiers justement condamné il faut aussi balayer devant la porte du ministère de l'Intérieur et améliorer les procédures judiciaires que nous fournissons. à l'ensemble à l'ensemble des fonctionnaires de la justice, il y a trop d'avocat assez spécialisé pour pas voir que la forme qu'on puisse souvent que le fond et qu'une procédure cassée alors que nous avons mis des mois et des mois pour retrouver telle ou telle délinquants ou criminels ne peut pas l'être, sur la forme, sans que nous soyons partie. Clairement interrogatif sur le contenu de cette procédure, il faut donc augmenter le nombre de pays. Il y a un manque à peu près de 5000 officiers de police judiciaire dans la police nationale c'est amant que structurant et je veux dire, mesdames et messieurs les sénateurs, que lorsque vous m'écrivez pour avoir davantage de policiers dans vos circonscriptions, je suis heureux de vous accorder lorsque je le peux, grâce aux crédits votés ces policiers qui sortent d'écoles, mais le ministre de l'Intérieur n'a pas dans son pouvoir, la possibilité d'affecter de force des OPJ dans vos commissariat ou dans vos services spécialisés nous ouvrons des postes. Mais si les gens n'y viennent pas, nous ne pouvons pas les forcer. Alors nous avons réfléchi à améliorer cette crise de l'investigation, sans lequel il n'y ait pas de réponse pénale forte et il n'y a pas non plus de travail de police à long terme qui vaille,

Et désormais sortie d'école, puisque désormais, les policiers font 12 mois de formation chez les gardiens de la paix au lieu de huit ils passeront le Bloc OPJ une partie d'entre eux le réussiront et pourront donc être affectés directement dans les commissariats, en ayant la qualité d'officier de police judiciaire, premier amélioration. 2ème amélioration vous avez créée dans loi sécurité globale la réserve opérationnelle de la police nationale sur le modèle de la gendarmerie nationale et vous aurez pu constater que désormais un peu partout en France des civils donne quelques jours de leur temps par semaine par mois pour enrichir les effectifs de police, améliorant ainsi le lien police population. Nous avons décidé de leur donner la possibilité de garder leur qualité de PJ quand on part à la retraite, jusqu'à présent un policier pouvait revenir dans son commissariat, la réserve opérationnelle mais ne pouvait pas faire des enquêtes judiciaires alors qu'il ne pouvait la veille lorsqu'il n'était pas partir en retraite 2ème amélioration 3ème amélioration nous créons des assistants d'enquête, je pense que c'est un point qui a 2 occuper un certain temps pendant ce débat, c'est révolutionnaire pour la police nationale, la gendarmerie nationale. Que fait un magistrat notamment au juge d'instruction. Si ce n'est que d'avoir un greffier qui l'aide pour le formalisme de la procédure. Le magistrat se concentre sur son travail de magistrat, pour lequel il a été formé et longuement et bien formés. Mais lorsqu'il s'agit de répondre à l'avocat lorsqu'il s'agit de taper à l'ordinateur lorsqu'il s'agit de pouvoir passer des pièces de faire des photocopies, c'est bien un greffier qui intervient, et qui, d'après, évidemment, des qualifications et des formations, le magistrat se concentrer sur sa procédure. Le policier lui fait tout. Il accueille le gardé à vue, il appelle le médecin, il répond aux sollicitations de l'avocat dès la première heure de garde à vue, il fait les photocopies, il tape à l'ordinateur lorsque l'ordinateur fonctionne et de plus en plus, il fonctionne grâce au crédit que vous ne votez donc c'est une très bonne chose, il répond aux interrogations du procureur de la République ou de son substitut, ce qui est bien logique on peut aussi dire ici que tous les procureurs de la République n'ont pas toujours la même façon de travailler avec tous les OPJ de France et donc on essaye de s'adapter à chaque demande de telle ou telle procureur et donc au lieu de dire telle les démagogues quelques cloisons alléger les droits de la défense pour alléger la procédure pénale, nous préférons dire que nous allons aider les policiers à remplir le formalisme nécessaires dont chacun a besoin, s'il devait être accusé, ce qui est bien logique et laisser les policiers se concentrer sur son travail de policier, ses assistants d'enquête que nous créons, c'est le personnel administratif du ministère de l'Intérieur qui fait un travail formidable qu'on va monter en compétence grâce à des formations, on en rediscutera j'imagine avec le rapporteur de Bresse et qui vont faire tout le travail administratif est formelle que font aujourd'hui les policiers qui demain pourront se concentrer intégralement à leur procédure au service d'enquête aux écoutes téléphoniques aux auditions aux perquisitions mais pas à la photocopie à la copie du dossier à l'appel du médecin, bref au formalisme qui est certes extrêmement nécessaire mais qui est du temps perdu pour l'officier de police judiciaire. Et ce moment la création des assistants d'enquête dont vous nous vous demandons 3000 postes dans la loi de programmation. Du ministère de l'Intérieur va révolutionner, je crois, le travail des OPJ de la police nationale et gendarmerie nationale et ce sera un grand moment, me semble-t-il, d'allégement des procédures pénales. Je voudrais aussi dire que nous avons une disposition dont je sais que le Sénat souhaité suivre l'avis du Conseil d'État et nous suivrons l'avis du Sénat qui a suivi l'avis du Conseil d'État sur les amendes forfaitaires délictuelles, c'est-à-dire ces amendes pénales toujours prises sous le sceau bien sûr du législateur, mais de l'action du procureur de la République qui définit la politique pénale dans son ressort et qui permet d'alléger un certain nombre de procédures. les sénateurs, vous ne m'avez longuement interrogé sur l'amende forfaitaire délictuelle, qui est inscrite otages et qui est une amende pénale, je rappelle, c'est pas une simple amende sur la consommation de stupéfiants. Vous m'avez demandé est-ce que ça marche est-ce que ça a marché : d'un côté, il y a ceux qui disait ça marcherait pas et l'autre, il y a ce qu'qui disait on allait déprécier la réponse pénale du consommateur de cannabis sur la voie publique. Mesdames, messieurs les sénateurs, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été maire. Et lorsque je suis devenu maire d'une première chose que j'ai fait, c'est, je suis allé avec les services de police nationale de ma commune. Pour faire comme fait c'est pas très original, chacun des élus, une tournée avec. Et à 23 heures 30 dans le métro de Tourcoing, monsieur le rapporteur. Je suis avec les effectifs de police et là monsieur sort de la rame de métro avec un joint de cannabis. Et là, le policier qui l'accompagnait, avec le commissaire de police qui ce jour là, était venue quand même accompagné maire j'espère qu'ils le font tous les soirs, sans les maires et son ministres. Il me dit monsieur qu'est-ce qu'on fait et ce qu'on fait comme d'habitude, où est-ce qu'on fait parce que vous êtes là, j'ai fait comme d'habitude, et le commissaire de police a pris le joint la mis par terre. La. Nettoyer d'un pied, il a dit à personne ne s'en aller. J'ai dit : mais pourquoi vous voulez pas interpellé, mais il me dit : Monsieur le maire si on interpelle quelqu'un qui fume un joint dans le métro, ça fait 3 personnes on sort du métro, on l'amène au commissariat, c'est à dix minutes on va appeler le procureur de la République, on va mettre en garde à vue, on va notifier ses droits, il va appeler son avocat, il va appeler son médecin, tout ça est normal et, au bout de qu'elle te heures peut-être quelques dizaines de minutes le coeur de la République va dire cher amis, vous pensez qu'on n'a pas autre chose que de s'inquiéter à enfin des procédures pour des consommateurs de cannabis. Alors il y a 2 réponses à ça, il y a ceux qui disent faut légaliser ce n'est pas la position du gouvernement. Je crois que je l'ai assez répété, c'est pas la position de absolument tout le monde non plus dans tous les partis cher ami. Parfois en cherche et parfois on trouve, c'est ça le problème des chercheurs et la 2ème option, c'est de pouvoir comprendre qu'on ne fait pas des gardes à vue et des peines de prison ferme pour des consommateurs de cannabis, mais qu'on doit faire une réponse pénale qui ne peut pas être que le rappel à la loi. l'amende forfaitaire délictuelle, qui ne concerne que les majeurs et non-récidivistes aujourd'hui fonctionne 260000 amendes ont été mises depuis le mois de septembre 2020. Extrêmement recouverte, puisque c'est votre question, plus que les Allemands de sécurité routière puisque nous avons depuis quelques mois, permis la saisie automatique. Des demande de la direction générale des finances publiques sur les comptes bancaires des personnes, et donc nous avons à la fois une inscription au casier et nous avons à la fois un recouvrement de ces amendes et, par ailleurs, mesdames et messieurs les sénateurs. ça permet surtout aux policiers et aux gendarmes de faire ces contrôles d'identité ou de faire ces contrôles sur la voie publique, puisque chacun sait ici qu'ils ne le font pas d'initiative sans une instruction du procureur de la République, sans être OPJ ou cent effectivement avoir un but de le faire comme l'amende forfaitaire délictuelle, le pire étant que le policier ou le gendarme ne puisse pas faire le contrôle d'identité ou la sanction d'une personne qui est manifestement trouble l'ordre public, d'une manière ou d'une autre, et c'est pour cela qu'une 2ème amende forfaitaire délictuelle est en ce moment en train d'être mis en place et expérimenté la fameuse occupation illicite des halls d'immeubles à Dili, qui avait été inventés par mes augustes prédécesseurs et qui n'avait jamais finalement été appliqué qu'il est très difficile évidemment de pouvoir caractériser ce délit dans une procédure judiciaire complète et qui aujourd'hui fonctionne, je pense notamment dans les Bouches-du-Rhône ou en Seine-Saint-Denis et qui permet aux policiers de mettre fin à ses occupations illicites dans le public, ils doivent désormais être généralisé. Cette amende forfaitaire délictuelle, elle, elle ne vise donc pas à rendre moins durs la sanction pénale, mais à la ronde, plus certaines ce qui compte, mesdames et messieurs les sénateurs, ce n'est pas la dureté de la sanction, mais sa certitude, il ne cherche à rien de condamner les gens à des peines de prison qui ne font jamais des années après leur sanction il sert tout en revanche et notamment la force de la loi que d'avoir la certitude de cette sanction, qu'elle soit effectivement appliquée immédiatement et pour ça, nous devons nous reposer sur les policiers sur les gendarmes qui sont des auxiliaires de justice et qui agissent au nom de la justice française et donc j'ai proposé dans ce texte une simplification de grande envergure de la procédure pénale en faisant et c'était la volonté du gouvernement dans un 1er temps que toutes les peines de prison inférieures à un an et dont nous savions qu'elle est. T'es pas appliquée parce que nous considérions tous qu'effectivement, à force de regarder les jurisprudences, elle ne l'était pas, et sans récidive depuis les patients l'amende forfaitaire délictuelle, le Conseil d'État a 10 juin cette disposition là considéré que nous étions trop large. Le Sénat avait finalement mais monsieur le rapporteur ne dira 2 possibilités : soit mettent des critères. Soit à faire une liste de délits. Monsieur le rapporteur Hervé nous nous rangeons à la position du rapporteur Hervé nous discuterons sans doute de la Coupe du nombre de ces délits mais nous pensons effectivement que ces amendes forfaitaires délictuelles par exemple faire un tag. Est ce qu'on est vraiment certain que ce texte mérite pas une amende, une inscription au casier judiciaire plutôt qu'une procédure pénale qui ne verra pas son aboutissement et qui permettra, je l'espère, d'avoir une meilleure réponse assez désagréable action du quotidien et donc nous aurons un débat très important et il s'en va, évidemment, avec la simplification de la prof Nous avons constaté également que le Sénat vous souhaitez enrichir sur un certain nombre de délits, je pense au rodéo ou à l'atteinte aux élus et le gouvernement sera avec sagesse à l'écoute de la haute assemblée sur cette question, je veux dire à ceux qui attendent le grand soir de l'échelle des peines que désolé de décevoir, je ne suis qu'un 1er rideau, c'est monsieur le garde des sceaux qui viendra vous présenter les états généraux de la justice le plus rapidement sera le mieux, je sais qu'il y travaille ardemment, mais je ne me permettrais pas de me substituer à Éric Dupond-Moretti, d'une part, ce ne serait pas logique dans les institutions, d'autre part, vous seriez déçu. Crise terroriste crise dans le public. Crise cyber, crise de la délinquance qui fait naître la crise de l'investigation. Crise climatique. Le texte ne parle pas que de sécurité, ou alors il parle de sécurité, quand j'ai dit dans mon introduction au sens large, notre modèle de sécurité civile qui est résiliant qui est fondé sur des pompiers valeureux, qui est fondé sur un système de volontariat original qui est fondé sur des départements et un état et une Europe qui aide fortement le fonctionnement de notre pays se trouve face à de grands problèmes. Le 1er c'est que vous le savez, les sapeurs pompiers interviennent de plus en plus dans des domaines qui ne relèvent pas de leur compétence absolument propre et ils remplace de plus en plus de médecins, absent du désert médical ou le système de santé difficilement organisés pour répondre aujourd'hui à la difficulté des Français, je sais que le ministre de santé il travaille. Nous avons essayé de répondre à cette question dans la loi, ma ce que vous allez dire voter, on aura l'occasion d'y revenir, mais surtout les crises climatiques ne font que commencer, on pense tous au méga feu ce qu'ont touché la Gironde et d'autres départements bien évidemment. Je veux ici dire que il y a eu plus de feu au nord de la Loire qu'au sud de la Loire cet été avec des départements comme le Jura, les Vosges, le Maine-et-Loire, le Finistère, dont les pompiers n'étaient évidemment ni les SDIS pas habitué à intervenir pour des feux de forêt de plus de 1000 hectares. Et de l'autre côté il des crises climatiques extrêmement fortes en outre-mer, mais aussi en en métropole je peux penser évidemment au début du quinquennat ce qui s'est passé à Saint-Martin avec Irma, mais je peux penser aussi à la vallée de la Vésubie, il n'y a pas si longtemps que ça, où nous avons été certes au rendez-vous avec l'action de la sécurité civile et des collectivités locales, mais très en deçà de ce qu'il faudrait préparer dans un réchauffement climatique généralisé et donc nous avons décidé de mettre un certain nombre de dispositions dans ce texte à la fois de renouvellement de la flotte, je pense aux hélicoptères à la fois de pouvoirs du préfet en cas de crise il n'a pas tous les mains aujourd'hui pour travailler avec toutes les agences et toutes les administrations et vous savez que c'est un drame dans la gestion des crises. Mais aussi dans le travail que nous souhaitons sans doute enrichir avec vous des modèles de sécurité civile, parce qu'il faut désormais se rendent compte que le réchauffement climatique étant au rendez-vous et même s'il ne feux sur 10 sont d'origine humaine, aujourd'hui les taux d'hydrométrie font que les forêts qui brûle, brûle très largement moins de 10 pour 100 de taux d'eau dans la forêt de Gironde on imagine même que l'incendie soit d'origine criminelle ou involontaire disposition de grandes dispositions sur la sécurité civile, notre modèle de sécurité civile dans dans ce texte. Alors je terminerai par dire que j'aussi l'honneur de présenter en janvier prochain après un débat au mois d'octobre et novembre ici un texte sur l'immigration, donc une absente de ce texte, mais pas absent de la politique gouvernementale, je crois que le Sénat lui-même souhaité des textes resserrer, on essaie de faire le plus resserrées possible avec un rapport annexé certes assez long, mais qui n'est pas législatif et je t'par vous dire, mesdames et messieurs les parlementaires que nous sommes dans la continuité du réarmement du ministère de l'Intérieur des 200 brigades de gendarmerie que nous allons recréer dans l'ensemble de vos territoires lorsque le gouvernement successifs, on a supprimé plus de 500 depuis 30 ans dans l'augmentation des effectifs de police que nous continuons à faire dans l'ensemble des commissariats de France bien évidemment dans les deux sens former ce que que nous créerons pour la sécurité civile, dans l'agence du numérique, puisqu'il faut créer l'impôt à la source au ministère de l'Intérieur qui est un ministère un peu arriérés sur le numérique et qu'il faut donc sans doute que nous modernisons comme nous l'avons fait à Bercy précédemment, ça demande aussi évidemment des moyens avec une agence unique du numérique et puis, avec pour la première fois, et le président de la République l'a évoqué, hier, pour la première fois depuis 17 ans, mais des messieurs les sénateurs, la recréation de sous-préfecture et la recréation d'agents de préfecture dans les préfectures, puisque nous vous proposons : la création d'à peu près 400 postes peut être pas encore assez, mais pour la première fois la reprise. Démographique du nombre d'agents préfecture si important pour notre territoire est au rendez-vous, je crois qu'à la fois le grand débat présidé par le président de la République avec les maires de France, mais aussi ce que nous avons vécu pendant la pandémie et le plan de relance ont montré à quel point les agents des préfectures était important en lien avec les collectivités locales pour les aider en ingénierie et de manière générale en action publique de l'État voilà Mesdames et messieurs les sénateurs, l'honneur que j'ai de présenter un texte qui je crois est très important pour le ministère de l'Intérieur en le disant je veux ici dans son remercier l'ensemble du Parlement qui, dans sa quasi-unanimité a toujours soutenu les forces de l'ordre, où les forces de sécurité civile qui, vous le savez, chaque jour, chaque nuit, risquent leur vie pour nous protéger. J'ai la grande responsabilité de diriger en votre nom, les femmes et les hommes qui est toujours très de ces risques. Et je ne peux pas terminé mon discours sans penser au 17 enterrement. Que j'ai eu à présider et je pense aussi aux 3400 blessés du plus depuis le 1er janvier par exemple dans les forces de l'ordre puisque notre action collective, derrière des chiffres derrière des milliards derrière des pourcentages derrière des textes réglementaires ou logiciel. Derrière des réformes, c'est surtout l'action des femmes et des hommes de terrain qui, dans aucun autre ministère. OK, d'autres ministères ne connaissent autant le risque de la vie et en terminant ce discours, je veux leur dire que si nous aurons des discussions politiques, je n'ignore pas que nous faisons tous selon nos opinions et selon nos convictions le mieux pour les protéger, je vous remercie. Avant de laisser la parole à notre collègue rapporteur Marc-Philippe Daubresse, permettez-moi, Monsieur le Ministre, de vous souhaiter, en y associant, bien sûr, mes collègues sénateurs, hein, très heureux anniversaire au moment où vous changez de décennies. Alors, mes chers collègues, il est 15 heures six je déclare clos le scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République. Monsieur Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des lois, vous êtes invités à prendre la parole. Merci madame la présidente, je voudrais à mon tour remercier le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer d'être ici avec nous cet après-midi ne il fête ses 40 ans, aujourd'hui nous sommes sensibles à cette marque de considération, puisqu'il nous a déposé un texte il, il vient de le dire qui est très important pour lui, pour son ministère pour les forces de sécurité et l'hommage que vous venez de leur rendent évidemment que nous nous y associons pleinement et nous sommes très sensibles à ce au sacrifices qu'ils font au jour le jour, mais vous avez décidé de passer l'après-midi à asseoir avec nous, Monsieur le Ministre, soyez rassurée, votre rapport fait 80 à 90 pages, mais nos collègues ont déposé 115 amendements sur l'article, hein, donc nous allons passer une bonne soirée d'anniversaire en votre compagnie. Mes chers collègues, madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la genèse du projet de loi, le ministre vient de le dire, qui nous rassemble aujourd'hui est longue, il fait suite à la publication du Livre blanc de la sécurité et du Beauvau de la sécurité qui a été suivi avec beaucoup de d'efficacité et de compétence par notre collègue Henri Leroy que je voudrais remercier à nouveau et au dépôt, vous l'avez dit, par le gouvernement d'une loi d'un 1er projet le 16 mars dernier qui a été raccourcie et resserrée, puisqu'il ne fait plus que 16 Arctique 2 programmatique, mais non des moines, puisque c'est une loi de programmation et d'orientation, j'ai eu l'honneur dans ma vie politique d'être ministre délégué auprès de Monsieur Borloo et de présenter, moi aussi, une partie d'une loi de programmation et d'orientation, c'est une loi très importante puisqu'un langage, elle donne une vision, un horizon et qu'langage sur 5 années, des crédits budgétaires dont on espère, puisque vous y avait été, je vous en parle qu'ils ne seront pas détricoter au jour le jour par Bercy, s'agissant justement en 1er lieu de cette programmation budgétaire le projet de loi prévoit dans son article, d'une progression chaque année du montant des crédits de paiement et plafonds des taxes affectées à votre ministère au total 15 milliards d'euros supplémentaires seraient budgété sur 5 ans par rapport aux crédits affectés au ministère de l'Intérieur en 2022 ces crédits supplémentaires, vous l'avez dit vont permettent de financer des mesures de modernisation et dans de nombreux investissements et vous y avez consacré, vous ne l'avez souligné vous avez, vous avez raison, beaucoup de moyens, surtout ce qui est digitalisation numérisation nouvelles techniques à l'utilisation de l'Intelligence artificielle, concernant le rapport annexé, nous avons adopté en commission des amendements sur plusieurs thématiques importantes d'abord de préciser dans le rapport annexé que la réforme de la police nationale devra prendre en compte les spécificités de la police judiciaire dans le cadre de ces enquêtes, celle-ci doit rester sous l'autorité fonctionnelle du procureur continue à traiter seule des affaires sensibles, enfin, au vu du développement exponentiel d'une délinquance organisée qui dépasse les frontières départementales, il pourrait être utile de prévoir des structures zonal, la commission des lois à l'initiative de notre président, François Noël Buffet a créé en son sein de mission d'information qui va faire des préconisations et qui soulignera les garanties apportées, nul doute, Monsieur le Ministre, que je pense de tiendrait compte, à l'initiative du groupe socialiste, nous avons également réaffirmé l'importance de l'accessibilité des démarches dématérialisées, notamment pour les personnes en situation de handicap sur les articles 3 et 4 du projet de loi qui vise à adapter les prérogatives dont disposent les forces de sécurité dans la lutte contre les nouvelles menaces et en particulier les cybermenaces nous avons, pour l'essentiel, soutenu la position du gouvernement et soutenu aussi toutes les crédits qui permettront d'investir dans ces technologies nouvelles, s'agissant de l'article 6 vous y avez fait allusion, Monsieur le Ministre, qui vise à permettre la prise de plainte et la déposition par le recours à la visio-conférence, il s'inscrit dans le développement du recours à ces dispositifs en matière de procédure pénale depuis les années, les années 2000, je rappelle que ces dispositions sont une simple faculté et non une obligation, nous avions prévu qu'il ne concernerait que les biens, vous m'avez longuement expliqué parce que nous avons tous des préventions sur certaines atteintes aux personnes que vous pensiez qu'on pouvait aller dans d'élargir ce Champ ce matin, la Commission a fait appel à la sagesse de l'Assemblée, je solliciterai donc votre point de vue, mais à titre personnel, je dois dire, vous m'avez convaincu enfin nos auditions ont montré l'urgence améliorer la réponse pénale sur 3 enjeux essentiels: les violences faites aux élus, vous l'avez dit vous-même plus 57 % en un an, les refus d'obtempérer, vous y avez fait allusion, malheureusement quand vous êtes obligé de, de, d'être aux côtés des familles dans les funérailles, plus 17 % depuis un an et les rodéos urbains dont chacun vu le feuilleton cet été, la commission a donc prévu un amendement pour protéger que nos concitoyens et renforcer les sanctions pour la discussion générale, je dis à nos collègues des groupes écologistes, communistes et sociale est-ce qu'on présentait de nombreux amendements qui tendent à réécrire la loi d'orientation que nous avons essayé de trouver une cohérence dans nos réponses : d'une part parce qu'il y a eu beaucoup de débats et en commission et dans cet hémicycle, sur la sécurité, le dernier sur la sécurité globale et et le terrorisme et donc nous sommes en cohérence par rapport à nos jurisprudence précédente et les positions que nous avions prise sans surprise et puis le président buffet à créer de mission d'information une s'est fait allusion sur la police judiciaire, l'autre sur la formation des forces de police et de gendarmerie et nous pensons qu'il faut attendre les préconisations de ces missions d'information avant de nous prononcer sur des amendements de nos collègues qui veulent toujours enrichir les formations donc ma position sera constante, ce qui fait que Monsieur le Ministre, ce dans les 115 amendements que nous allons examiner ce soir il y aura fort peu d'avis favorable, mais parce que la commission avait élaboré un très bon texte d'ailleurs mon ami Loïc Hervé va vous le démontrer, à l'instant, merci de votre écoute mes collègues. Si monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Loïc Hervé, rapporteur de la commission des lois. Madame la présidente, monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, mon cher collègue, co-rapporteur, mes chers collègues, il me revient maintenant après Marc Philippe Daubresse d'évoquer devant vous, l'article 5 relatif aux réseaux radio du futur, puis les articles, c'est à seize du projet de loi la plupart de ces articles ont été approuvé par la commission des lois, nous avons considéré qu'il contribuerait à simplifier la procédure pénale et qu'il donnerait aux forces de sécurité intérieure, de nouveaux outils juridiques leur permettant de mieux remplir leur mission, la Commission a toutefois réécrit les dispositions relatives à l'amende forfaitaire délictuelle, Monsieur le Ministre, vous l'avez évoqué, elle a enrichi le texte, on y a serrant certaines mesures qui ne figuraient dans la première version de la Lopmi, mais pas dans le texte, déposé par le gouvernement sur le bureau du Sénat concernant tout d'abord le le réseau radio du futur, la commission n'est bien sûr pas opposé à ce projet qui vise à doter nos forces de sécurité, nos services de secours d'un réseau de communication plus moderne et plus résiliant, la commission a cependant supprimer l'article 5 qui tendait à habiliter le gouvernement à prendre par ordonnances, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet, nous préférions que ces dispositions soient inscrites en dur directement dans la loi, à l'occasion de l'examen du texte en séance publique, le gouvernement a donc déposé un amendement en ce sens qu'nous donne satisfaction, qui a pris en compte nos observations et sur lequel nous reviendrons lors de la discussion des articles. Un ensemble de mesures a pour ambition de renforcer la filière en charge de l'investigation au sein de la police et de la gendarmerie nationale afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes, compte tenu de la désaffection dont souffrent depuis trop longtemps, la police judiciaire, ces mesures nous paraissent aller dans le bon sens, je citerai en particulier, la proposition de recruter 5500 assistant d'enquête chargée de veiller au respect de la procédure, ce qui libérera du temps pour les enquêteurs, qui pourront ainsi se concentrer sur leur coeur de métier, la commission a souhaité qu'une évaluation soit réalisée dans 3 ans de la plus-Value apportée par ce nouveau cadre d'emploi, elle a également adopté un amendement de notre collègue Alain Richard tendant à mieux ton encadrer la compétence accordée aux futurs assistants d'enquêtes en matière de transcriptions des enregistrements, ce qui répond à une inquiétude exprimée par le Conseil d'État pour renforcer les effectifs de la police judiciaire, il est prévu que les policiers et gendarmes puisse passer l'examen pour devenir OPJ officiers de police judiciaire dès la fin de leur formation, la commission a adopté de mesures complémentaires : premièrement, les élèves officiers de la gendarmerie recevrait la qualité d'agent de police judiciaire, ce qui est déjà le cas pour les élèves. Officier de la police et les prérogatives d'agent de police judiciaire sera étendu sous le contrôle permanent d'un OPJ. La commission n'a en revanche pas été convaincu par la proposition de généraliser la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, à tous les délits de moins d'un an d'emprisonnement puni par mois d'un an d'emprisonnement, ce qui correspondrait dans notre pays, à 3400 infraction pénale, la procédure de l'amende forfaitaire, a fait ses preuves pour réprimer certains délits qui peuvent être aisément constater par les forces de l'Ordre je pense à la consommation des stupéfiants et je me range à la démonstration faite tout à l'heure par monsieur le Ministre,

c'est pourquoi la commission a refusé cette généralisation au profit d'une extension limitée à quelques délits pour lesquels l'amende forfaitaire nous paraît plus adaptée, je pense aux tags au délit d'entrave à la circulation encore la décence des tensions sans permis d'un chien d'attaque, je terminerai, madame la présidente, mon exposé en évoquant 2 autres mesures notables qui figure dans ce texte, d'abord, la proposition de réprimer plus Armand l'outrage sexiste qui deviendrait un délit en cas de circonstances aggravantes, la commission il y est favorable et elle ont ça enverrait un signal de fermeté aux auteurs de cette infraction, encore trop peu réprimé sur le terrain. Ensuite, à l'article 15 la proposition d'accroître les prérogatives des des préfets de département en cas de de crise d'une partie culinaire gravité, l'objectif est qu'il puisse exercer pleinement leur autorité sur tous les services déconcentrés pour faire face à des événements exceptionnels tels que nous en avons d'ailleurs connu ces derniers mois sur notre proposition, la Commission a souhaité étendre ce dispositif aux agences régionales de santé-les ARS, qu'il ne nous paraît pas justifiée à la lumière notamment de ce que nous avons observé pendant la crise du Covid de maintenir à l'écart de cette unité de commandement à l'échelle départementale la Commission espère que ces mesures législatives qui pourront être enrichi au cours de notre discussion, combinée à l'accroissement des moyens des effectifs contribueront à améliorer la sécurité des Français, beaucoup reste à faire, mais il s'agit d'un pas dans la bonne direction, qui nous conduit à soutenir l'adoption de ce texte, merci beaucoup. Merci, monsieur le rapporteur, la parole est à monsieur Philippe Paul, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans un long processus entamé il y a déjà plusieurs années, on se souviendra particulièrement de la commission d'enquête du Sénat sur l'état des forces de sécurité intérieure, sous l'égide de François Grosdidier et Michel Boutant, qui avait déjà attiré l'attention sur les causes du malaise policier en 2018 la proposition numéro 10 du rapport de la commission d'enquête était la suivante : élaborer un Livre blanc de la sécurité intérieure, puis adopté une loi de programmation permettant de fixer un cadre budgétaire opérationnel et stratégiques stable et crédible. nous vous savons donc gré aujourd'hui, Monsieur le Ministre d'avoir mené à bien ses travaux du Livre blanc, puis le Beauvau de la sécurité qui a permis de prendre d'importantes mesures en faveur des policiers, des gendarmes, ainsi les grandes orientations du rapport annexé nous vous apparaissent pertinente et nécessaire transformation numérique, augmentation de la présence sur la voie publique, lutte contre les violences intrafamiliales prévention des crises telles sont, effectivement, les grands défis que nous avons affrontées pour que nos forces de sécurité soient plus efficace et plus crédible contre la délinquance en constante évolution, en outre, les 15 milliards prévus pour mener à bien l'ensemble de ces transformations et celle qui concerne les autres missions du ministère de l'Intérieur, représente un effort important, sans doute à la hauteur de l'enjeu, en revanche, nous restons un peu sur notre faim sur le lien qui existe entre ses grandes orientations et sa programmation des moyens, en effet, ce texte c'est trop centrée sur la sécurité pour être une véritable loi d'orientation de l'ensemble du ministère de l'Intérieur, mais en même temps, il est trop imprécis sur les moyens accordés aux missions des policiers et des gendarmes pour être une véritable loi de programmation de la sécurité ainsi, Monsieur le Ministre, vous savez que nous sommes, nous nous sommes inquiétés a plus âme à plusieurs reprises de l'État, indigne d'une grande partie du parc immobilier domaniale de la gendarmerie nationale sur ce sujet rien de précis dans le texte, il nous faudra si l'on en croit le rapport annexé attendra encore la mise en place d'un nouveau service chargé des habits d'établir un tendanciel de dépenses pourtant ne considérez-vous pas les que les moyens sont déjà bien, a eu notifié et qu'il est urgent d'agir, c'est en tout cas, notre conviction, d'où les amendements apportés par notre commission enfin nous regrettons une certaine précipitation dans la mise en place des 200 nouvelles brigades de gendarmerie, nous craignons que les collectivités soient sollicités alors que certains ne peuvent pas se permettre un tel investissement, ce qui a motivé notre amendement commun avec la commission des lois, pour finir, je voudrais encore une fois saluer l'engagement contre la délinquance, de l'ensemble de nos forces de sécurité et en particulier pour ce qui concerne notre commission de la gendarmerie nationale, dont le statut militaire, reste pour nous la meilleure garantie d'efficacité partout où elle exerce sa compétence, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, la parole est à Madame Gisèle Jourda. Rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées. madame la présidente, monsieur le Ministre, chers collègues, une des grandes orientations de cette loi revêt une importance particulière, il s'agit de ça le qui prévoit de faire du renforcement de la présence dans la ruralité, une nouvelle au politique à part entière, la relocalisation de certains services du ministère dans les territoires ruraux et les villes moyennes ou encore l'objectif de doubler la présence des forces de sécurité sur le terrain vont assurément dans le bon sens, tout comme le recours accru aux réserves opérationnelles de la police et gendarmerie nationale qui se sont rendus indispensables dans de nombreux territoires encore faut-il que l'augmentation de leurs effectifs aille de Pair avec démission suffisamment nombreuses sur l'amener, c'est ce dont nous avons voulu nous assurer par l'heure d'par l'un de nos amendements, il s'agit ainsi de permettre un réel processus d'acquisition de compétences et une fidélisation de des réservistes qui se rendent, disponible pour des missions au profit de la collectivité, à notre sens, le chapitre consacré au renforcement du maillage des forces de sécurité dans les territoires ruraux et péri-urbaines ah un peu trop maigri, Monsieur le Ministre, par rapport au livre blanc les développements sur la répartition territoriale des 2 forces s'étant évanouie chemin seule annonce concrète, la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, sans autre précision, mon expérience locale m'incline à penser que cette question de la répartition des forces n'est pas pas secondaire les deux forces ne sont pas interchangeables, la polyvalence de la gendarmerie avec l'unité entre les enquêteurs judiciaires et gendarmerie départementale enraciné dans le territoire s'opposant à la spécialisation policière, il serait donc préférable d'élaborer des critères objectifs, prenant en compte la réalité de la délinquance, afin d'effectuer des ajustements, enfin plutôt que d'un rester aux critères simpliste en ce qui concerne la coopération entre les 2 forces sur un même territoire en cas d'urgence ou des phénomènes particuliers de délinquance, il est également nécessaire de généraliser les bonnes pratiques autour des protocoles départementaux, police, gendarmerie, d'où 2 amendements sur ces sujets connexes offert les modalités de la création des 200 brigade nous préoccupe notamment en ce qui concerne la participation des collectivités territoriales, l'audition du président de la commission sécurité de l'AMF, nous a confirmé, dans ses haines dans autre surprise, les annonces sur le terrain, qui se sont succédé ces derniers jours, avant que nous commencions l'examen du texte, je souhaite vraiment et nous souhaitons que les débats d'aujourd'hui permettront de dissiper tous ces août je vous remercie. Merci madame la rapporteure dans la suite de la discussion générale là. Parole est à monsieur Alain Richard pour le groupe RDPI. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, voici un texte de grande importance qui fait bien commencé de façon tonique notre session et cette partie du du mandat gouvernemental et présidentiel, ce texte va définir le cadre des moyens humains et matériels de nos forces de sécurité pour les 5 années qui viennent de façon ample puisqu'il y a une forte augmentation des crédits et le rapport prévoit aussi de façon cohérente, les grandes orientations d'emploi les grandes finalités de ses moyens, donc nous avons là un document cohérent qui qui réutilise en effet les débats qui ont eu lieu et qui ont été très pluraliste très partagés dans le livre blanc et dans le bobo de la sécurité, il me semble donc que c'est une un un bon débouché de débats qui ont été approfondi, je veux souligner aussi que la programmation à part elle-même des vertus, elle ne peut s'appliquer évidemment à tous les ministères, parce que sinon ça deviendrait très compliqué de faire un un, une loi de finance annuelles mais sur un sujet comme la sécurité intérieure, il me semble que c'était une bonne option que le ministre a bien fait de dépenser de l'énergie et de la persuasion pour arriver à une programmation qui nous servira de de comment dire de balises en quelque sorte à chaque loi de finances pour vérifier que la continuité et la l'organisation cohérente de ces moyens se développent. Et comme le ministre l'a dit, je ne vais pas prolonger cette partie-là, ces moyens bénéficie naturellement aux deux grandes forces de sécurité intérieure, police nationale et gendarmerie nationale avec une meilleure diffusion territoriale mais bénéficie aussi de façon très substantielle à la sécurité civile et donc à tous les moyens de lutte contre les catastrophes qui nous qui cette loi de programmation bénéficie aussi à tout le l'environnement numérique ou plutôt le support numérique du ministère qui, qui va mettre en cohérence. Toutes les fonctions opérationnelles de sécurité intérieure et, comme le ministre l'a reconnu lui-même qu'il va faire sortir le ministère d'une phase où il n'était pas particulièrement en avance sur ce sujet-là, on nous voyons des gains de, de, de, d'efficacité opérationnelle qui vont se se poursuivre et, enfin, le ministre-là aussi noté je voulais absolument faire mention pour une pour la première fois des récréations d'emplois dans les préfectures, alors que c'est vrai que les personnels des préfectures, les cadres de ces, de ces administrations ont dû faire face à beaucoup de réduction de moyens humains au cours des 15 20 dernières années, et était dans des conditions de travail qui a été souvent très tendu et je crois que c'est ça sera excellent pour motiver les les cadres et les préfectures, ajoutons que tout ça va comporter des enjeux de recrutement et de formation sur lesquelles le ministère devra bien sûr se mobiliser je voudrais aussi mentionné, puisque les 2 rapporteurs se sont bien réparti le travail : les principales dispositions concrètes puisqu'il y a 2 articles de programmation sur lesquels on peut commenter mais qui, qui ne sont qu'une approbation d'un programme global et ensuite des articles qui sont des articles législatifs, je crois que nous faisons un bon choix la la majorité de la commission, en ne suis en pas la preuve le 1er projet du gouvernement et en faisant plutôt une liste fermée pour l'instant des infractions pour lesquelles pourraient s'appliquer la l'amende forfaitaire délictuelle, je crois que c'est important pour une raison bien sûr, il y a une raison juridique que le Conseil d'État a soulevé, mais il y a aussi une raison pratique, c'est que toutes vos équipes, monsieur le ministre, qui seront en déplacement sur la voie publique et qui auront la faculté d'utiliser l'amende forfaitaire. Délictuel auront un problème de capacité mémorielle, si on leur dit : vous avez le droit de le faire pour 500 des pour 500 délit différents et il me semble donc il vaut mieux se concentrer sur une dizaine pour l'instant de délits qui sont ni limitativement énumérées et sur lesquels ils auront le savoir-faire, l'aide à la rédaction tout simplement de l'amende de de la la le procès verbal d'un mode de manière que ce soit efficace rapidement et si comme on peut le supposer, ça se révèle efficace, on pourra faire une deuxième vague entre guillemets de catégorie d'infractions qui pourront en être redevable. Je crois aussi que la le développement des assistants d'enquête est une une bonne mesure que ça complète en effet le la capacité des officiers de police judiciaire et que d'ailleurs les autres mesures qui simplifie le travail des OPJ ne sont vraiment pas du luxe notamment les habilitations, plus rapides et la possibilité de demander des actes de police scientifique sans passer par une procédure formaliste, donc il me semble que c'est un texte sur lequel la Commission a très bien travaillé, je crois, en en très forte convergence avec le l'esprit du gouvernement. Ce qui prouve que c'était un très beau choix d'amener ce projet de loi au Sénat en premier, donc nous la pression beaucoup, je voulais terminer en soulignant que nous sommes dans une situation de tension à l'heure actuelle, sur le plan du moral dans les effectifs de la police judiciaire que vous y attacher une grande importance, Monsieur le Ministre, mais nous nous suivons toute cette affaire, il me semble qu'il y a d'abord une une recommandation à faire, qui est que ça ne traîne plus trop et que la décision formelle de réorganisation soit prise et qu'elle soit bien concentré sur une refonte des moyens et une centralisation des soutiens, mais qui n'affecte pas la liberté professionnelle et la responsabilité des agents, mais le malaise, il y a aussi, il faut bien le dire, d'une situation de surcharge, que vous avez décrite, mais aussi d'un sentiment d'un succès assez fréquent du fait de la complexification de la du code de procédure pénale, qui entraîne un certain nombre, il faut bien dire de pas, pardonnez-moi l'expression, mais de plantage parce que les pièges de procédures qui sont dans ce code sont vraiment trop nombreux, je si j'ai une recommandation à faire au gouvernement dans son ensemble et pas seulement à vous, Monsieur le Ministre, c'est que la la refonte complète du code de procédure pénale soit mené à bien le plus vite possible, par des autorités jury juridique indiscutable de manière que les officiers de police judiciaire puisse travailler avec un bon outil donc encore notre approbation. Merci, Monsieur Richard, la parole est à monsieur Jérôme Durain pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur que nous examinons aujourd'hui est en quelque sorte un texte 2,0, je ne l'affublent pas de ce qualificatif par rapport à son volet numérique qui est conséquent, mais bien parce qu'il s'agit de la 2ème version de ce texte après celle qui nous avait été présenté en pleine campagne présidentielle cette 2ème version amaigrie de moitié m'apparaît dans l'ensemble plus sage, elle a été expurgé de ses dispositions relatives à l'immigration par exemple si l'immigration fait bien partie des prérogatives du ministère de l'Intérieur, je remercie la première Ministre d'avoir choisi de ne pas confondre causalité et corrélation en ce qui concerne les thèmes de l'immigration et de la délinquance, mais Monsieur le Ministre et je vais peut-être en surprendre certains, ce n'est-ce pas à ce stade, le texte de sécurité le plus déséquilibré que nous ayons eu à étudier au Parlement ces dernières années, cela tient à son architecture 7 Lopmi comprend 3 parties : la partie budgétaire la partie orientation avec le rapport annexé et la partie normative avec le reste du projet de loi en ce qui concerne la partie budgétaire, le groupe socialiste se félicite des moyens accordés au ministère de l'Intérieur dans une période où nos forces de l'ordre sont soumises à une pression quotidienne dans une société, souvent décrite comme confrontée à davantage de violence. Notre groupe veut profiter de ce débat pour exprimer à nouveau un soutien sans réserve à nos forces de l'ordre, police, gendarmerie, police municipale, qui ne compte bien souvent ni leurs heures, ni leurs efforts pour assurer la tranquillité de nos concitoyens Nantes au Creusot, à Saint-Denis, Dijon, Besançon ou ailleurs, la plupart des candidats à l'élection présidentielle, s'était engagé à accorder davantage de moyens à la lutte contre l'insécurité, les 15 milliards annoncés dans ce texte constitue donc une bonne nouvelle et nous ne ferons pas la fine bouche, même si nous serons vigilants sur l'application de cette Lopmi dans les années qui viennent, dans un contexte économique toujours incertain. En ce qui concerne la partie orientation qui constitue en quelque sorte le mode d'emploi de ces 15 milliards il y a une cohérence dans le rapport annexé qui nous est fournie, on comprend la filiation avec le livre blanc de la sécurité et le bureau de la sécurité, la place octroyée au numérique, même si nous comprenons les inquiétudes de certains agents, échaudés par les échecs passés nous semble légitime, si nous ne croyons pas dans le solutionner isme technologique, nous sommes convaincus qu'il faut donner à la police, les moyens d'affronter la criminalité à armes égales sur les moyens plus classiques, nous attendons d'être rassurés sur la méthode, notamment en ce qui concerne les déploiements des brigades de gendarmerie, nous avons pris bonne note des orientations annoncées en ce qui concerne les rapports police-population comme sur la formation, mais nous pensons qu'il pourrait être fait davantage, nous avons en outre quelques interrogations sur le caractère exact du continuum de sécurité, les associations, les associations d'élus aiment à rappeler que les collectivités doivent agir en complémentarité avec les forces de l'ordre et non en substitution, mon collègue Hussein Bourgi reviendra sur ce point dans quelques instants, comme beaucoup de groupes, nous profiterons du rapport annexé pour proposer des amendements sans surprise, ce sera pour nous l'occasion d'aborder la question de la réforme de la police et de la place de la police judiciaire qui suscite une levée de boucliers, massive, n'en déplaise au DGPN en ce qui concerne maintenant la partie normative, je tiens en 1er lieu à saluer le travail des rapporteurs, j'ai lu ici ou là, que le Sénat avait durci le texte, cela ne me semble pas correspondre à la réalité sur plusieurs articles messieurs les rapporteurs ont tenté d'apporter des éléments de cadrage je pense ici au dépôt de plainte par Visio à l'abandon des ordonnances pour la radio prévisions apporter aux précisions apportées pour l'amende forfaitaire délictuelle, par exemple, notre groupe comprend et partage par ailleurs la volonté d'a rapporté des rapporteurs d'aligner les sanctions pour violences sur les élus sur celle risqué pour des violences sur d'autres, dépositaire de l'autorité publique, pour autant, le groupe socialiste, écologiste, plus qu'un, ne se satisfait pas de ce projet de loi telle que sorti de la commission des lois, nous défendrons dans ce débat, nos exigences sur plusieurs points qui nous paraissent essentiels : il s'agit des amendes forfaitaires délictuelles de la réponse au rançongiciel, nous formulerons aussi la proposition d'une juridiction spécialisée dans les violences sexuelles et que c'est sexiste infligés aux femmes et aux enfants, nous proposerons également de revenir sur des articles ou la commission a effectivement durci le texte, je pense ici au refus d'obtempérer et oh rodéo urbain, je ne crois pas, nous ne croyons pas que sur ces sujets difficiles la réponse réside dans un simple durcissement de la punition sur ce point comme sur l'ensemble de la loi, je pense que nous aurons une discussion parlementaire sereine si notre chambre n'a pas été renouvelé au mois de juin soyez assuré, Monsieur le Ministre, qui avait parfaitement consciente de l'état du pays et de la nécessité d'avoir un dialogue, un dialogue parlementaire constructif le Sénat était déjà partisan du parlementarisme, de fait, avant la majorité introuvable, sortie des urnes en 2022 nous ne doutons pas que vous saurez y contribuer avec nous, nous aurons en tout cas cette nécessaire prise en compte du Parlement dans sa diversité, au moment de décider de notre vote. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Éliane Assassi. Pour le groupe CRCE. Madame la présidente.

madame la présidente, monsieur le le ministre, mes chers collègues, le projet de Love a été annoncée donc lors des conclusions du Beauvau de la sécurité en 2021, il s'inscrit dans la logique de la loi dite de sécurité globale de mars 2021 nous dont nous demandons l'abrogation, s'appuyant sur le Livre blanc de la sécurité intérieure publié en novembre 2020, près de la moitié des moyens prévus par le projet de l'opinion est dédié à la transformation numérique alors loin de moi l'idée de rejeter cette transformation Yves, il me semble que l'équilibre n'est pas respectée au sens où la formation de nos policiers auraient dû être elle aussi aurait dû elle aussi par donc faire l'objet d'un effort conséquent en terme de moyens alors je sais bien que certains ici ne veulent pas l'entendre, mais mon groupe, c'est toujours, toujours refusé à stigmatiser nos forces de l'ordre et il a toujours reconnu les difficultés dans l'accomplissement de leur mission, mais nous portons l'idée selon laquelle les dispositifs de maintien de l'ordre doivent reposer le plus souvent possible sur la négociation, le dialogue et la pédagogie et non sur la répression au risque d'aggraver le sentiment de défiance envers la police et une partie de la population, malgré vos affirmations, Monsieur le Ministre, selon laquelle la Lopmi est un levier de rapprochement avec les citoyens, force est de constater que c'est le contraire d'une part, les victimes seront mises à distance par cette loi ainsi les dépôts de plainte devrait se faire en présentiel et non en ligne chacune et chacun ici peut en comprendre les raisons d'autre part, le projet de l'autre mis s'éloigne de la coordination entre police et justice en prenant le tout répressif par la systématisation et la simplification de la procédure en simplifiant la procédure pénale, sans vouloir l'expliquer n'est-ce pas considérer que nos agents sont un cas seraient incapables de les comprendre, de la comprendre, on ne cesse de nous répéter qu'il ne s'agit pas d'un texte sur la justice, mais au regard de ces dispositions, nous pouvons sérieusement en douter, La Lopmi, en généralisant l'amende forfaitaire forfaitaire délictuelle à certains délits prive les justiciables des garanties fondamentales coffre la procédure pénale, elle délègue aux agents de police, une fonction qui relèvent en principe de l'autorité judiciaire, comme l'a souligné la Cncdh mais également le Conseil d'État dans son avis du 10 mars dernier La Lopmi envisage également que les OPJ puisse procéder à des constatations et des examens techniques ou scientifiques sans réquisition préalable éloignant alors les enquêteurs du contrôle en temps réel du parquet ou du juge d'instruction, or il est difficile d'accepter l'idée que la police technique et scientifique puisse s'autosaisir en outre un abaissement des exigences dans le recrutement des OPJ n'est pas souhaitable, un officier de police judiciaire dispose de pouvoirs coercitifs dont ne disposent pas un agent de police judiciaire la responsabilité nécessite l'expérience de même mettre en place la fonction d'assistant de police et de gendarmerie n'est pas un gage d'efficacité, la procédure pénale, même son aspect le plus infime nécessite vigilance et rigueur mais chers collègues avec cette ni nous sommes face à une excusez-moi l'expression, Mac Donald isolation de la procédure pénale, or servir le citoyen et sa sécurité, voilà le coeur battant du métier de policier, le projet de l'autre mis l'ignore pour nous proposer une vision un peu fantasmer à savoir une police hyper récup'équipés, c'est le Label Robocop qui nous est proposé des exosquelettes ou encore des policiers, des gendarmes et des pompiers augmenter ne font pas de nos agents de police de meilleurs professionnels ce texte passe à côté des véritables enjeux des métiers de la sécurité publique, nous souhaitons une police qui met qui met en oeuvre le triptyque : prévention, dissuasion, répression, une police non pas coupé du citoyen mais une police de proximité exemplaire et digne, ce qui est l'ambition portée par des milliers de policières et de policiers votre tâche au gouvernement, notre tâche au Parlement, c'est d'aider à restaurer une confiance trop souvent perdues, quelle politique, mettez-vous en place pour parler à la jeunesse des quartiers populaires, nous dénonçons par ailleurs les partenariats privilégiés avec des sociétés privées, dans la droite ligne du projet de sécurité globale que La Lopmi envisage traduit la volonté de l'exécutif, de se couper de la police républicaine au profit de sécurité de sécurité mercantile bien éloignée de fonctions régaliennes de l'État enfin La Lopmi et l'antichambre de la réforme à venir portant là dès la départementalisation de la police judiciaire une départementalisation synonyme d'intrusion du pouvoir exécutif dans les procédures pénales, la colère s'exprime fortement au sein de la magistrature chez les avocats et comme nous l'avons vu la semaine dernière chez les enquêteurs de police judiciaire, Monsieur le Ministre, notre société est sous tension à la crise sociale se sont ajoutés les cris sanitaire et la guerre sur notre continent la réalité de la crise climatique et écologique est incontournable : l'insécurité globale et la police, ce doit être une force d'apaisement et non pas rajouter de l'anxiété à l'anxiété cette difficile équation je veux bien le reconnaître, entre prévention, accompagnement et protection est un défi, votre loi et votre approche ne peuvent en l'état le relevé, nous voterons donc contre ce projet de loi de de l'eau qui et proposeront au Sénat des voies alternatives, même si j'ai bien compris qu'elle risque d'être rejeté par nos rapporteurs Merci madame la présidente. La parole est à Madame Dominique veut rien pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je tiens tout d'abord à vous dire que j'apprécie particulièrement les développements de votre rapport annexé à l'article 1 cas nous demandons beaucoup à nos policiers et à nos gendarmes, mais ils ont besoin de soutien et d'accueil et d'accompagnement, et dans ce rapport, nous trouvons tout ce dont nous rêvons pour un meilleur fonctionnement de la police de la gendarmerie et la meilleure prise en charge des victimes mais pardonnez-moi, je ne suis pas sûr que tout soit applicable sans avoir recours à des modifications de la loi modifications que l'on ne trouve pas forcément dans le texte que nous examinons, aujourd'hui, je pense par exemple aux évolutions nécessaires pour assurer notre sécurité lors des grands événements sportifs à venir ce n'est pas grave, l'intention est louable et cela nous donnera la l'occasion de nous revoir prochainement revenons donc au texte sur la police judiciaire d'abord un syndicat bien connu communiquent souvent en disant que le problème de la police, c'est la justice, mais c'est oublier que parfois le problème de la justice, c'est la police, et je n'incrimine bien sûr pas les policiers mais force est de constater que la filière d'investigation n'attire plus autant qu'avant et ces difficultés de recrutement, avec de nombreuses équipes en sous-effectif, ont des conséquences directes sur la qualité des enquêtes et le délai de mise en oeuvre de la réponse pénale et les stocks qui se constituent dans les commissariats sont autant d'affaires non traitées, donc de justice non rendue qui vont se terminer trop souvent en déclaration sans suite, faute d'avoir les moyens de les poursuivre les un sentiment d'injustice au plaignant mais est-ce un sentiment. En réponse, ce texte prévoit une facilitation de l'exercice des missions d'investigation, un renforcement de l'efficacité de leur action, une formation initiale, plus orienté vers les métiers de l'investigation, ainsi que la création d'agent de police judiciaire, je salue également la proposition de nos rapporteurs Loïc Hervé et Marc Philippe Daubresse, d'attribuer la qualité d'agent de police judiciaire aux élèves officiers de la gendarmerie nationale durant leur scolarité afin qu'il puisse constituer un renfort appréciable durant leur stage en unité territoriale. Ces apports de outre permettre à plus de dossiers d'être traité de mieux accompagner les victimes, mais attention à certaines propositions du rapport annexé car permettre à chacun et chacune de déposer une plainte et d'en effectuer le suivi en ligne avec un contact Direct par Chat avec un policier ou un gendarme, ce sont de formidables eux idée mais est-ce bien réaliste tant ces propositions représentent un bond de géant par rapport à la situation actuelle et je crains quelques déceptions j'espère cependant me tromper sur le cas particulier des violences intra-familiales qui sont devenus un contentieux de masse avec la libération de la parole, le rapport prévoit un doublement du nombre d'enquêteurs dédiés et le financement de 200 postes d'intervenants sociaux en en police et en gendarmerie ces intervenants sociaux sont très utiles, hein, et il est vrai que leur financement poser trop souvent un problème que vous proposez donc de régler, je salue aussi la création d'un fichier de prévention des violences intrafamiliales afin de mesurer pour un jour, empêcher la réitération de faits de violence et de prendre en compte les signaux de dangerosité là aussi son efficacité dépendra de la formation des forces de l'ordre et de leur capacité à distinguer des signaux faibles et à prendre les bonnes décisions rapidement un gendarme ne doit plus hésiter à demander le retrait d'une arme à feu d'un ami chasseur dans un contexte de violences intra-familiales. Enfin, les associations pourront accompagner plus efficacement les femmes victimes de violences en organisant le dépôt de plainte dans leurs locaux et en signalant les faits dont elles ont connaissance aux forces de l'ordre, j'imagine que ce dépôt de plainte à se fera par déplacement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, d'où l'utilité de la création de ces derniers. Toutes ces mesures vont dans le bon sens et sont les bienvenus si elles sont réellement appliquée, je ne manquerai pas de faire un suivi particulièrement attentif de la mise en oeuvre de ces mesures, après avoir fait un état des lieux dans le cadre de la mission que m'a faut confier la première ministre sur le sujet des violences intrafamiliales sur le numérique, enfin j'ai eu souvent l'occasion de me pencher sur la situation du numérique pour la justice, bien moins pour la police, hein, mais heureusement, je ne suis pas dépaysé, tant les problèmes sont similaires d'ailleurs, justice et police ont tout intérêt à travailler et à concevoir ensemble les outils transversaux Cassiopée, par exemple, qui pénalise tant de magistrats temps magistrats que policiers et gendarmes dans le cadre de la procédure pénale numérique est un bon exemple de cette nécessité d'un travail concerté, l'idée d'une grande agence du numérique pour le ministère de l'Intérieur, avec une double tête, gendarmerie, police paraît donc pertinente, mais seulement si les leçons de l'échec du projet scribes en partie due à une divergence de vision sur le numérique entre police et et gendarmerie ont bien été tirés. Enfin, cela ne relève pas de la loi, mais peut être faudrait-il aussi se concentrer sur le plus urgent et sur ce qui peut être réglé rapidement, par exemple, certaines gendarmeries au hasard dans l'Yonne, ne sont toujours pas fibrer et ne le seront pas avant, dans le meilleur des cas, 2023, il est sans doute possible d'accélérer les choses, hasard toujours je vous ai alerté sur ce sujet par une récente question écrite restée sans réponse à ce jour, cet exemple ben souligné l'importance du maillage territorial maillage que vous venez renforcer avec les nouvelles brigades de gendarmerie et les gendarmes mobiles, mieux équipées en plus grand nombre, ainsi que par le développement des maisons France service sur ce sujet d'ailleurs Monsieur le midi Monsieur le Ministre, ça me fait toujours tiquer quand j'entends vos services parler de création de Maisons France service alors oui, c'est bien une création de non, oui, mais j'entends beaucoup notre préfet notamment parler de création, alors qu'en fait il, c'est souvent une montée en compétence, c'est vrai, mais de structures de maisons de service au public déjà existantes, je pense qu'il y a suffisamment à faire et que vous en fait déjà beaucoup pour ne pas gommer ce que vos prédécesseurs ont pu déjà créé, je le dis d'autant plus facilement que ça n'était pas ma famille politique mais seulement que les maisons de services public existait déjà en définitive ce texte enrichi par le travail de nos rapporteurs que je tiens à saluer une nouvelle fois, constitue une bonne réponse aux problématiques que nous connaissons sous réserve de sa juste application mais vous pouvez compter Monsieur le Ministre, sur la vigilance du Sénat à ce sujet en conséquence le groupe Union centriste votera ce texte. Merci, cher collègue. Mes chers collègues. Si le résultat du scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République, nombre de votants 288 suffrages exprimés, 261 majorité absolue des suffrages exprimés 131 bulletins blancs 27 bulletin nul 0,

Ce candidat ayant. Tenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est proclamé juge suppléant à la Cour de justice de la République Monsieur Gilbert Favreau va être appelé à prêter devant le Sénat le serment prévue par l'article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, je vais donner lecture de la formule du serment, je vous prie de bien vouloir vous lever. à l'appel de votre nom et de répondre, en levant la main droite par les mots, je le jure, voici la formule du serment. Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions de garder le secret des délibérations et des votes et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. magistrat. Acte est donné par le Sénat du serment qui vient d'être prêté devant lui. Et nous reprenons le fil de la discussion avec l'intervention de monsieur Stéphane Ravier.

cela n'a malheureusement pas été le sort va y arriver, réservé à Éric Arella directeur zonal de la police judiciaire de Marseille limogé, ce vendredi, connu chez nous pour son professionnalisme et son intégrité, vous avez coupé la tête d'un géant et cela ne vous a pas grandi et vous persistez puisque dans la presse vous menacer de sanctions des policiers manifestants vous ne réformez pas vous détruisez un monument avec des méthodes expéditives, que des observateurs étrangers n'aurait pas tort de qualifier d'autoritaire et peu démocratique mais revenons à ce projet de loi vous n'éradiquer pas les causes de l'insécurité, vous vous contentez d'en gérer les conséquences, on ne lit rien de la nouvelle stratégie en vue de rompre avec le délitement de l'autorité et l'augmentation de l'insécurité, le contexte est pourtant très dégradé, nous restons sous la menace terroriste incapables : incapables de localiser et d'expulser un imam islamiste, au point qu'il a dû s'expulser lui-même et impuissant devant la recrudescence des rodéos urbains et des refus d'obtempérer mortel pour les agents et les passants et l'on entend monter une détestable petite musique venue d'Hugo qui stands dont les paroles affirme que la police tue sans que ce texte n'instaure de nouveaux grands principes pour la protéger la présomption de légitime défense pour toutes les forces de l'ordre, faisant usage de leur arme dans l'exercice de leurs fonctions eut été un symbole fort, vous l'avez refusé de plus, la police municipale n'a semble-t-il pas sa place dans votre continueront de sécurité, elles sont pourtant les dernières garante de l'ordre dans les communes reculé et quasi systématiquement les les primo-intervenante sur le terrain, c'est totalement anachronique de parcourir ce texte sans aucune mention, ses agents municipaux il conviendrait pourtant de leur accorder des compétences de police judiciaire et de généraliser le port d'arme de catégorie B enfin vous avez évoqué en août, la représentation des étrangers dans les statistiques de la police et de la justice, avec notamment 55 pour 100 des délinquants interpellés à Marseille qui sont étrangers, nous n'avons aucune traduction dans ce texte du commencement d'un début de solution pour y remédier, vous qui aimez décloisonner je pensais naïvement que vous comprendriez l'utilité de ne pas légiférer avec des oeillères, ce n'est pas pour rien que le classement des villes les plus sûres du monde donne, Marseille et Nice derrière Bagdad et Tripoli qui représentent respectivement les villes d'Al-Qaïda et de Daesh, après que l'insécurité aura gagné l'ensemble du territoire urbain à la répartition de l'immigration dans les campagnes, voulue par Emmanuel Macron général se généralisera à n'en pas douter, le grand ensauvagement à évoluer, à évaluer le coût financier de cette insécurité française à 69 milliards d'euros par an, un Torrent de larmes et de sang dans un gouffre financier, ce phénomène national menacé les Français dans leur intégrité physique dans leur prospérité dans leur cohésion sachez à l'avenir, Monsieur le Ministre, vous en souvenir, et de ne plus vous trompez de cible en limogeant plutôt que ceux qui la combattent. Merci Monsieur Ravier, la parole est à Madame Maryse Carrère pour le groupe RDSE. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, notre pays va être le lieu de nombreux événements ces prochaines années, jeux olympiques et Coupe du monde de rugby qui s'ajouteront aux défis habituel de la sécurité publique, nous ne voulons pas revivre les polémiques de mai dernier, autour de l'organisation de la finale de Ligue des Champions au Stade de France, c'est pour cela qu'il faut impérativement prévenir tout risque de fiasco aussi je rejoins la position ne non rapporteur pour l'essentiel, ce texte va dans la bonne direction et répond à un certain nombres d'atteinte du ministère de l'Intérieur et des besoins de sécurité publique, nous saluons les annonces et les ambitions du rapport et de la perspective budgétaire, outre l'adaptation au monde numérique, il est tenu compte des problématiques de l'ancrage local des forces de sécurité, cela nécessite évidemment des moyennes du point de vue du personnel et du matériel, nous y serons vigilants lors de l'examen des prochains Budgets et surtout ces nouvelles ressources devront tenir compte de la spécificité des enjeux locaux, on parle ce souvent en zone urbanisée, lorsqu'il est question de sécurité publique, mais le milieu rural ne doit pas être oubliée, nous saluons également les apports de notre commission concernant l'accessibilité des personnes en situation de handicap, d'autant que la France accuse toujours un retard en matière d'accessibilité universelle en revanche un autre point nous préoccupe très particulièrement celui de la formation des personnels concourant à la sécurité intérieure du pays si la formation initiale est relativement étoffé, il n'a, n'est pas toujours de même pour la formation continue, qui est trop souvent délaissée au cours de la carrière il y a encore à faire si nous souhaitons améliorer la performance des divers des différents services, les travaux en cours de la mission de d'information sur les moyens d'action et les méthodes d'intervention de la police et la gendarmerie nous révèle une marge importante de progression de ce point de vue nous émettons quelques réserves quant à la disposition de l'article 9 qui assouplit les conditions requises, hein, pour exercer les attributions attachés à la qualité d'officier de police judiciaire, notamment en supprimant la condition des 3 années de service, bien sûr, cela ne retirera rien à la formation initiale de l'argent, mais 3 années de pratique lui seront enlevés alors que chacun sait combien ces postes sont exigeants et que l'expérience et le PAM d'armes de la formation des agents un policier ou un gendarme doté de responsabilités, notamment en matière d'investigation doit être expérimentée, nous nous interrogeons aussi sur la simplification de la procédure pénale, le rapport annexe le souligne, il y a un sujet autour de la complexité procédurale de l'action pénale pour autant nous croyons aussi que la simplification ne doit pas s'accompagner d'une dégradation de certains principes fondamentaux, l'encadrement procédural donne sa légitimité à l'action de l'État en matière de répression, c'est un moyen pour écarter l'arbitraire et de ce point de vue, il ne saurait être question de renoncer à des éléments de procédure seulement parce que les policiers et les gendarmes ne sont plus en capacité de les respecter en revanche simplifier notre droit jusqu'à renoncer à l'intervention d'un juge ne saurait être une réponse : manque de moyens et de formation d'un au service, la généralisation de l'amende forfaitaire délictuelle nous apparaissait comme une fausse bonne idée, dans la mesure où elle participait à marquer un Net recul de l'action des juges comme du principe fondamental d'individualisation des peines je veux donc saluer la position retenue par notre commission des lois, sur cette question en limitant très fortement ce dispositif je rajouterai un élément sur la récente polémique déclenchée suite à la proposition de réforme de la PJ, les inquiétudes sont légitimes, les experts des expérimentations ont été menées, quels sont les résultats de ces expérimentations, nous aurions souhaité à Alain avoir connaissance afin de mieux nous prononcer sur ce projet de loi si sur le fond, on pourrait y être favorable sur la forme, le manque de concertation aura été pénalisant, mais Monsieur le Ministre, vous avez fait, pas plus tard qu'hier, hein, pas dans ce sens je conclurai en évoquant un dernier sujet qui s'est invité dans ce projet de loi suite à l'adoption d'un article par notre commission visant notamment au renforcement de la réponse pénale quant aux violences faites aux élus, ce sujet est très préoccupant, nous observons ces dernières, ces derniers mois une forte recrudescence des incivilités et surtout des agressions envers les élus locaux, nous avions déposé plusieurs amendements reprenant différentes propositions de loi déposées par mes collègues du groupe RDSE Nathalie Delattre : Éric Gold je regrette qu'ils aient été pour la plupart déclarée irrecevable en raison d'une approche restrictive du périmètre de ce projet de loi nous voulons redire notre mobilisation sur ce sujet, toutes ces remarques n'enlève pas l'intérêt de ce projet de loi que notre groupe votera dans sa quasi-majorité, je vous remercie. Merci madame Carrère, la parole est à monsieur le président, Roger Karoutchi pour le groupe Les Républicains. madame la présidente, monsieur le Ministre, puisque la présidente Assassi a fait tout à l'heure référence cinéma cinématographique sur Robocop moi je pensais plutôt 40ème rugissants oui, Monsieur le Ministre le le film le 40ème Rugissants ah exactement 40 ans, il y a 2 82 comme vous, si je puis me permettre et et et il est filmé avec un acteur formidable Jacques Perrin, qui avait 40 ans au moment du film et cet acteur affronte des lames de fond. Bah, vous ministre de l'Intérieur, vous affrontez des lames de fond. La lame de fond, c'est la course poursuite entre l'État, les collectivités qui essayent d'assurer la sécurité. Et d'autre part, la délinquance qui se renforce. Qu'il y a de plus en plus violentes, c'est de plus en plus technique, qui est de plus en plus difficile à maîtriser et on a l'impression, depuis plusieurs années, nous avons ici voté beaucoup de textes sur la sécurité, on a l'impression qu'il y a une course dont on est jamais vainqueur parce que les délinquants toujours plus de moyens, parce que les délinquants toujours plus de technique et parce que nous, respectant les règles et les lois, nous avons du mal à la contrecarrer. Et nous n'avons jamais réussi dans ce pays à faire de la sécurité, un droit fondamental, la sécurité n'est pas un droit fondamental en France, elle n'est pas et elle n'a pas de qualité de critères supra législatif en réalité aucun citoyen ne peut opposer son droit à la sécurité, il y a une obligation de moyens, il y a pas une obligation de résultat. Et c'est en soi-même, quelque chose d'extrêmement difficile, alors je ne vais pas revenir sur les excellents rapports des excellents rapporteurs je ne vous cacherai pas que, naturellement, bien entendu, et vous le savez, nous allons voter ce texte amendé par la commission des lois, parce que je pense que peut être, pour la première fois. L'État reprend la course et l'état peut peut être se donner si naturellement de budget en budget on respecte cette loi d'orientation peut peut-être se donner les moyens de gagner contre les délinquants à partir de là, je n'ai pas grand chose à vous dire à part. Vous avez de la chance, à 40 ans ministre de l'Intérieur, vous avez un texte qui pourra, après tout, est quand même un texte qui fait fait large majorité et un texte qui va marquer, je pense que ça va marquer parce que vous avez cranté un certain nombre de sujets qui vont être déterminante dans la lutte contre l'insécurité et à partir de là, je n'ai plus grand chose à vous dire, sinon peut-être deux 3 observations : premières observations Monsieur le Ministre, vous ne le prendrez pas mal, je pense que. Vous aviez changé l'image. Du ministre de l'Intérieur auprès des policiers. Beaucoup de policiers, beaucoup de syndicats de police, il y a six mois me disait. ça bouge. On est content, ça marche, on a plus de moyens, plus d'équipements, on est reconnu et il faut reconnaître, et j'en ai parlé avec Philippe, il faut reconnaître que cette affaire de de la police judiciaire il faut trouver une solution, vous avez fait des propositions, ces derniers jours, je pense que le rapporteur, en fait, il faut que vous trouviez sincèrement une solution parce que c'est pas seulement l'affaire de la police judiciaire. C'est l'affaire de la police en général et nous avons besoin de la police de la République et vous avez besoin de la police de la République, il n'y a pas d'état, il n'y a pas de république sans police, sans police reconnu par les citoyens comme étant leur police, la police du peuple, la police de la République et c'est pour cela que très naturellement dans mon camp politique, jamais personne ne se permettrait de critiquer l'action de la police ou de tenir des propos qu'on a pu entendre dans certains temps et j'admets bien volontiers que ça n'est pas dans le groupe communiste qui l'a dit tout à l'heure et c'est pas de ce côté-là que les choses se disent : il faut que l'action de la police soit soutenue, si nous voulons avoir une chance que cette sécurité qui est un droit premier pour les citoyens soient aussi quelque chose que chacun des citoyens s'approprient et là vous avez un rôle essentiel à jouer le 2ème élément et dans le temps qui m'est imparti, j'arrêterai là, Monsieur le Ministre, vous avez dit vous-même tout à l'heure, il y aura Monsieur Dupond-Moretti à qui je ne doute pas vous parler régulièrement, qui viendra avec un texte sur les mises sur les états généraux de la justice, et cetera franchement depuis des années, j'entends dire, police, justice, les policiers disent les magistrats ne nous suivent pas donc c'est décourageant les magistrats disent oui mais la police parfois, et on a un côté, on a un côté un peu, on peut se parler, à quand des états généraux de la police et de la justice, pas seulement entre les 2 ministres d'entre tous les syndicats, tous les acteurs, par pitié, les Français méritent bien ça.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mais si le rapporteur, mes chers collègues. Notre pays, les homicides sont en hausse, les coups et blessures volontaires, ainsi que les violences sexuelles connaissent une très forte augmentation. Ce constat dressé par le ministère de l'Intérieur pour l'an 2020 doivent nous alarmer délinquance du quotidien ou grande criminalité, l'enjeu, la cité dans notre pays et majeur pour nos concitoyens, le président Macron avait promis lors de sa réélection de renforcer la présence des forces de l'ordre sur le terrain, le projet de loi qui trace le chemin pour y parvenir d'ici à 2027, il met les moyens, budget, la voiture de 20 pour 100 de plus de 20 %. Bien que cette trajectoire soit pour crédible par le Conseil d'État, il est indispensable de juguler la progression de la sécurité. Elle brise la vie de certains de nos concitoyens et empoisonne les autres l'insécurité met en péril le pacte républicain, elle nuit également au développement de notre économie et au rayonnement de notre pays, la France s'apprête en outre à accueillir de grands événements. C'est 2 raisons supplémentaires pour que les forces de l'ordre disposent de moyens d'assurer lors de public. Notre groupe est en faveur de cette augmentation de budget. Parallèlement à celui de la justice, l'État doit être en mesure d'assurer ses missions régaliennes, il s'agit, en effet, en effet, de ses missions les plus essentielles, les fonds prévus pour les forces de l'ordre serviront notamment à augmenter les effectifs, c'est une très bonne chose. Je souhaiterais plus partisans évoquer 2 sujets concernant les effectifs, le 1er est celui du zonage, les interventions en zone gendarmerie, il me semble très important que les forces de l'ordre connaissent le terrain, les habitants pour agir au mieux, au plus près de leur caserne, le second concerne la police judiciaire, une réforme est sans doute nécessaire, mais il semble indispensable que ces en conservent leur capacité d'enquêtes très spécifique et nous y serons attentifs. La problématique des effectifs ne doit pas par ailleurs masqué, celle des équipements et des installations vétustes, il est grand temps d'inverser cette tendance et de là, nous, je sais que c'est le cas, c'est parti pour le rapport annexé au projet de loi prend en compte cette problématique, nous soutenons également attentifs à la mise en oeuvre des mesures annoncées au des aspects pragmatique du rapport et de 2 premiers articles, le projet de loi contient plusieurs dispositions de procédure pénale. Il était notamment question de généraliser la procédure d'amende forfaitaire à toutes les infractions punies dans d'un emprisonnement d'au moins d'un an maximum, le Conseil d'État a indiqué dans son avis qu'une telle disposition, ce rentrer dans ce périmètre, plus de 3400 infractions, la solution retenue par la commission nous paraît plus sage, une dizaine d'infractions supplémentaires pourront désormais faire l'objet de cette procédure, notre groupe est satisfait de ce ciblage beaucoup plus précis, nous sommes inquiets de constater que les taux de groupements de ces amendes forfaitaires et pour usage de stupéfiants, fer de lance de cette procédure, le taux et qui est inférieur à 50 % en 2021, dans ces conditions, il nous paraît important d'améliorer sur comment de cette amende le texte prévoit également la création de la fondation d'enquête ce personnel sera chargé de réaliser leurs tâches administratives qui éloigne les policiers du terrain. Amende forfaitaire et d'enquête sont donc de des symptômes d'un mal plus profond de 2008 à 2022 le code de procédure pénale est passé de 1700 Arctique, à 2014 articles la complexification des procédures plus difficile le travail des policiers, des magistrats et des professeurs du droit. Cette complexification est également porteuse de risques pour nos concitoyens, qu'ils soient mises en cause aux victimes. l'inflation normative de juguler les procédures doit de ce que veut le Mans simplifier la fusion des quatre d'enquête pourrait y contribuer, les états généraux de la justice ont rappelé la nécessité de conduire une telle étude d'impact sur la faisabilité et le portier une telle fusion il faut-il procéder sans attendre les mesures contenues dans ce projet de loi sont nécessaires, notre groupe comme beaucoup dans cet hémicycle, soutiendra son adoption ne reçoit demande une action forte de l'État pour lutter contre l'insécurité, ce texte y contribue, mais il faudra continuer à agir. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Guy Bénard Roche. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires.

Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, l'avenir le rôle du ministère de l'Intérieur, son organisation, ses moyens sur des sujets au coeur de notre pacte républicain de notre organisation sociale, de la protection des citoyens du respect des droits du justiciable je ne surprendrai personne si j'exprime ici au nom de mon groupe, les craintes que les dispositions présentes dans ce projet suscite un mélange de Big Mother is watching You et les meilleurs passages de 84 d'Orwell et du pire de Robocop Mystery Shoppers policiers augmenter robot d'accueil drone aux frontières numérisation à outrance, là à l'heure où l'électronique tous une immense partie de nos citoyens et où les territoires se sentent de plus en plus éloignés de l'accès à un humain du service public. Nous nous devant vous tous, chers collègues, mon groupe et moi, de mettre en action 100 sobriété notre énergie et nos retraites et licence collective pour ce projet de loi, nous avons donc voulu être une force de proposition, puisque le ministre le rappeler, hier, dans sa lettre envoyée à l'ensemble de la PJ sa porte est ouverte à toutes les propositions, nos propositions, notre vision sont issus d'une réelle réflexion d'équilibre et pourrait se décliner en 2 éléments principaux : le 1er ne vous étonnera pas, Monsieur le Ministre, nous n'avons pas la même vision de la police de la sécurité de la protection du Mathias, de l'ordre de la tranquillité publique que celle que vous exposez et défendez dans cette loi et ce rapport, mais nous ne partageons pas non plus la position que nous trouvons attentiste des rapporteurs et de la majorité, un exemple frappant est celui de l'amende forfaitaire à laquelle nous sommes opposés, non seulement ça connaît jusqu'à présent une application territoriale disparates et hétérogènes, oserais-je dire éminemment concentré sur certains quartiers, mais surtout de plus en plus cette rupture de traitement territorial, la volonté du gouvernement de l'État légèrement resterait par la commission sans aucune réelle étude de son efficacité de son efficience actuel est un pas de plus dans l'éloignement du juge ce texte assis, se fait l'écho des pires positionnement qui voudrait que la justice, garante de l'application du droit soit un frein aux forces de l'ordre. Cela nous amène au second élément essentiel dont je parlais, c'est que nous demandons que les femmes et les hommes, dont le rôle est d'assurer notre sécurité et notre tranquillité soit traités avec humanité, avec respect, avec considération. Clairement, nous considérons que les conditions de travail de nos forces de l'Ordre ne sont pas au niveau des services que nous attendons de nous devons veiller à diminuer leur souffrance au travail à leur métier, le sens qu'ils ont perdu notre soutien aux agents de l'État doit reposer sur la réalité retrouvée d'exercer un métier avec et pour leurs concitoyens. Le besoin de sécurité des citoyens portent aussi sur la transparence de l'action de la police, une meilleure gestion des dérives parfois violentes, une nouvelle vision de l'IGPN mais aussi sur la transparence des données de la police de leur publication de leur transmission aux élus, entre autres, le besoin de sécurité des citoyens portent aussi sur la gestion des risques incendie amplifiée par l'inaction climatique du gouvernement, condamné à plusieurs reprises nous proposera des améliorations sur ce sujet des services incendie le besoin de sécurité des citoyens portent aussi sur leur environnement, c'est pour cela, nous tracera aussi des pistes pour le développement d'une police environnementale le besoin des citoyens, c'est aussi que le rapport annexe, ce que le rapport annexe appelle pudiquement la transparence et l'exemplarité des forces de l'ordre, nous ferons de nombreuses propositions sur le sujet a fait renouer la confiance que les citoyens doivent avoir dans leurs forces de l'ordre nouveau remercie d'avance de ne pas faire d'amalgame à des fins purement politique de nos positions avec des supposés positionnement Antipolis ou anti-républicain, tout au contraire, nous prétendra et nous chercherons à vous démontrer que nos propositions sont plus protectrice, non seulement pour les citoyens, mais aussi pour tous les personnels des forces de l'ordre, tant physiquement que mentalement, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, nous ne voulons pas de droit à nos frontières et du tout surveillance dans la politique migratoire y compris à l'intérieur de nos frontières européennes, nous voulons une réelle réflexion sur des mouvements migratoires au niveau européen, mais aussi une refonte de nos politiques d'accueil, nous ne voulons pas d'une réforme de la police judiciaire qui déstabiliserait la dépendance du travail des magistrats de projets qui entraîne le risque d'un affaiblissement de la lutte contre le grand banditisme, refusant perdent à la PJ sa spécialisation attachant les services de la PJ des des PN en établissement Liens forts entre ceci et les préfets, ce projet génère une confusion entre le pouvoir judiciaire, administratif, nous voulons une sanctuarisation des moyens prof de la PJ de sa spécificité, une sanctuarisation de l'accès à la qualification d'OPJ loi de sa dilution dans les autres formes de sécurité loi d'une marginalisation des parquets dans la définition de la politique pénale. Nous ne voulons pas vider les commissariats juste pour mettre du bleu dans la rue et faire du chiffre, il y a des amendes forfaitaires, nous voulons une réelle police de proximité pacificatrice liée à son territoire, nous ne voulons pas de LBD de drônes de lacrymo de la tactique de Lana sous d'autres techniques d'interpellation dangereuses dans les doctrines de maintien de l'ordre et le contrôle de la population depuis l'action j'observe parfois avec surprise, souvent avec effroi la dérive autoritaire de certains textes, la sécurité, l'enjeu de tous, mais les dérives sécuritaires sont toujours venir des même Monsieur le Ministre, c'est pourquoi nous proposons l'expression de notre vision par un grand nombre d'amendements que nous allons discuter et dont le sort Celera notre position finale vis-à-vis de ce texte. Merci monsieur Bénard Roche, la parole est à monsieur Hussein Bourgi pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, monsieur le Ministre. Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est proposé à au moins 2 vertus la première, c'est celle de répondre à une demande ancienne visant à doter nos services de police et de gendarmerie, des moyens humains et matériels à la hauteur des missions qui leur sont confiées, la seconde vertu de ce projet d'être ambitieux avec l'annonce de moyens et d'objectifs conséquent ces 2 vertus étant relevée et saluer je veux monsieur le Ministre, me focaliser sur les sujets qui méritent un peu plus d'engagement et de précision, de votre part, si votre projet de loi et le rapport annexé liste les grandes orientations et les grandes trajectoires cela manque parfois de précision et de précisions chiffrées, en particulier, nous formons le voeu que le débat parlementaire nous permettent de répondre à ces attentes pour sortir des indications parfois vague et floues, vous avez élaboré votre doctrine en matière de sécurité à partir du Livre blanc de la sécurité intérieure et du Beauvau de la sécurité à l'occasion de l'élaboration de ce continuant de sécurité, vous avez voulu établir un partenariat renforcé avec les communes en matière de lutte contre l'insécurité, or, Monsieur le Ministre, les maires sont de plus en plus nombreux à déchanter, en effet, lorsqu'ils souhaitent s'équiper en caméras de surveillance par exemple et qu'il sollicite la préfecture pour obtenir un cofinancement, il leur aurait répondu que l'enveloppe n'a pas évolué depuis le dernières élections municipales, il y a de plus en plus de communes qui souhaitent s'équiper de caméras de vidéosurveillance l'enveloppe allouée aux préfectures n'a pas augmenté lorsque ces mêmes maires prennent à leur compte les travaux d'aménagement de locaux de gendarmerie et de police, c'est le cas dans l'Hérault par exemple à Frontignan ses bureaux se trouve au bout de quelques années, malheureusement déserté avec les policiers qui sont transférés dans la commune voisine, celle de cette en particulier dès lors, les maires sont de plus en plus nombreux à s'interroger à nous interroger sur ces réalités qu'ils vivent, ils ont le sentiment que le partenariat que vous leur avait proposé et parfois déséquilibré en leur défaveur, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux ont accueilli avec circonspection et même prudence l'annonce de la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, ils craignent une mise en concurrence entre les territoires, ceux qui ont les moyens de mettre à disposition des locaux et les autres, ils craignent de financer de locaux et de ne pas avoir le service attendu par les administrés à l'arrivée, qu'avez-vous à leur dire, monsieur le Ministre, car ils ont le sentiment d'avoir parfois conclu avec l'État un contrat léonin, en matière de sécurité, beaucoup de maires sont confrontés à la multiplication des infractions en matière de sécurité, de circulation, de stationnement dans les grands centres urbains, les moyens techniques sont désormais disponibles, ça s'appelle la. Lecture automatisée des plaques d'immatriculation, ces outils permettent un contrôle efficace et régulier des flux important de véhicules, néanmoins, en raison du cadre réglementaire, vous le savez, Monsieur le Ministre, le Champ d'utilisation des systèmes reste limitée, c'est pourquoi, dans le respect des règles de protection des données personnelles, il est impératif de faire évoluer à la réglementation pour lutter plus efficacement, permettre aux maire prêtre présidents d'intercommunalité de lutter plus efficacement contre le stationnement gênant sur les places réservées aux PMR contre le stationnement gênant sur les plateformes de tramway contre le stationnement gênant sur les pistes cyclables qui malheureusement occasionne souvent des accidents corporels et parfois des accidents mortels, plusieurs maires de grandes villes vous ont écrit en ce sens, c'est le cas de Michaël Delafosse, maire de la ville de Montpellier, ils attendent une réponse de votre part, concernant l'évolution réglementaire, ce n'est pas du domaine législatif, mais je me permets de le préciser ici monsieur le Ministre, vous avez annoncé votre volonté de doubler les effectifs en matière de police et de gendarmerie sur le terrain nous souscrivons tous à cet objectif, mais si l'objectif est atteint, il restera néanmoins la question du traitement là Christian du traitement des procédures d'infraction qui seront constatées dès lors le risque est réel pour ne pas dire certains, Monsieur le Ministre, de voir le stock de procédure en souffrance augmenter, comment appréhendez-vous cette situation et comment comptez-vous faire pour endiguer cette probabilité, vous souhaitez enfin permettre à la prise de plainte et la déposition par le recours à la visio-conférence, pourquoi pas, ce qui compte, ce n'est pas la manière dont on dépose plainte pré-plainte visioconférence, ce qui compte, c'est que le plaignant soit informé tout au long de la procédure et en la marche les Miles on a hier là les marges de projection de progression et de projections sont réelles et sérieuses bon de conclure mon intervention le ministre je voudrais réitérer au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain, l'intérêt que nous portons aux juridictions spécialisées en matière de violences conjugales et intrafamiliales, peut-être que le débat, vous permettra de nous dire votre sentiment à la question ce projet étant expurgé des éléments clivant, Monsieur le Ministre, nous formons le voeu et que vous puissiez faire un pas envers nous, afin de témoigner la considération que nous avons tous pour les gendarmes et les policiers et l'intérêt que nous portons à la sécurité des Françaises et des Français, je vous remercie. La parole est à monsieur Philippe Dominati pour le groupe des Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, après avoir écouté mais diffère rend collègue de cette assemblée, Monsieur le Ministre, je peux vous dire qu'il y a un 1er succès, c'est que rarement une loi a été aussi attendue et à apporter aussi d'intérêts sont toutes les bancs de cette assemblée, et pourtant la gestion n'a pas été facile parce que dans le premier quinquennat nous avons eu le sentiment que la mission sécurité n'était pas une priorité du gouvernement et du président de la République, la mission n'a pas été facile parce que, en réalité, vous avez évoqué la crise du terrorisme dans cette horrible année de 2015 mais vous êtes le 7ème ministre de l'Intérieur en 7 ans, ce sur une période où je prends le dernier quinquennat et l'avant- dernier quinquennat et le dernier quinquennat dont vous êtes le 7ème Ministre de l'Intérieur en ces temps, c'est pour dire que, pour les pouvoirs publics, malgré la crise du terrorisme ce ministère mérité des réformes méritait une attention particulière et en réalité on a géré de crises, une succession de crises qui se sont manifestées par les agents de l'État à des fréquences de plus en plus régulières, ça nous amenait évidemment normalement à la au Livre blanc qui a été suivi par les rencontres de Beauvau une première version de la de Lopmi en mars 2022, et une seconde version aujourd'hui et cette seconde version effectivement c'est un intérêt particulier parce que nous sommes au début d'une mandature et que vous avez su probablement attirer l'attention du chef de l'État sur la nécessité de recentrer la mission sécurité au coeur du débat en ce début de mandature ans quel quel quel est l'effort pour ma part, je m'arrêterai, surtout à l'article 2 de cette loi d'orientation, c'est-à-dire l'effort financier, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a une OPCI l'objet en 2009 2 milliards 500 dans la Lopmi, c'est 6 fois plus, j'ai essayé de faire, c'est pas tout à fait simple le périmètre et périmètre constants sur les 2 dernières sur 2 séquences de 5 ans, c'est-à-dire 2013, 2017 l'effort financier, les crédits de paiement avaient augmenté

effectivement l'effort financier pour les 5 ans à venir, d'autant que la principale et le principal effort sera fait au cours du budget 2023 et plus que satisfaisante puisque ce sera de l'ordre de 22 ça c'est pour l'aspect financier, l'enveloppe puis financière cette l'obtenir répond à deux principales. Repas revendications mais nécessité : la première, c'est celle de répondre à la révolution numérique, l'effort est important, c'est une véritable modernisation du ministère et des agents de sécurité sur le terrain, la 2ème réforme c'est de doubler les effectifs sur le terrain, effectivement, comme ça a été dit par de nombreux collègues, le doublement des effectifs sur le terrain ne doit pas se faire évidemment au détriment du fonctionnement et de l'investissement, c'est la dérive que nous avons constaté au Sénat au cours de ces dernières années, qui a été redressée, notamment grâce au crédit de relance du Covid et que vous avez sécurisé dans cette loi de programmation du ministère de l'Intérieur, c'est un ministère où il n'est pas simple de faire des réformes. En réalité, il n'y en a pas eu de pluie, la crise du terrorisme en aurait si il y en a une, celle du temps de travail, celle du temps de travail, le vendredi, fort ça occupé le ministère pendant 5 ans à peu près, vous avez annoncé à la fin du quinquennat précédent qu'effectivement ça avait été abandonné mais ça avait été initiée par Bernard Cazeneuve, c'était normalement une bombe destinée à l'alternance qui devait exploser et puis finalement ça ne s'est pas produit comme prévu donc, c'était la seule réforme qu'il y a eu ces dernières années concernant ce ministère, il est en ce moment, la réforme de la PJ, réforme de la PJ, elle est pas simple à appréhender parce qu'effectivement, comme tout le monde on écoute les inquiétudes il y a des inquiétudes sur la départementalisation il y a des inquiétudes sur le quantitatif par rapport au qualitatif, mais pour autant elle est initiée par le directeur général de la police judiciaire, qui a passé je crois 29 ans dans cette institution et elle semble en partie répondre effectivement la nécessité d'incarner à nouveau par une seule personne dans un lieu précis la fonction policière et enfin il y a une réforme qui a pas du tout été abordés qui annoncé gouvernement par gouvernement régulièrement mais si la disparité qu'il y a entre la police nationale et la préfecture de police, le coeur je dirais du du pays, ça a été annoncé, nous avons eu Monsieur Kastec Bernard et Monsieur N'uñez, devant le Parlement, qui avait dit que ce serait l'une des réformes clés et puis finalement au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a ces disparités, il n'y a rien dans cette loi d'orientation concernant le coeur du pays, coeur du pays, où toutes les sensibilités politiques, il y a quelques années en tant qu'élu parisien, je tiens à le souligner, était plutôt pour la défense de la police nationale, Bertrand Delanoë avait annoncé qu'il souhaitait que ça reste comme ça, et maintenant toutes les sensibilités politiques sont pour une police municipale, on en a beaucoup parlé, mais il n'y a strictement rien sur ce sujet, monsieur le Ministre, c'est un début, continuer dans les réformes de ce ministère, puisque c'est une nécessité beaucoup trop de retard a été pris. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Henri Leroy pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le Président, buffet, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Voilà une réforme qui va dans le bon sens. En tant que partie prenante comme parlementaires très engagés pour la sécurité de nos con pitreries de nos compatriotes, c'est naturellement que je voterai cette 7 cette 7 Lopmi et c'est suffisamment rare pour être souligné, correspond aux espoirs des forces de sécurité intérieure, aux attentes des élus locaux et nationaux, qui avait eu l'occasion de s'exprimer, notamment lors des nombreuses séances du Beauvau de la sécurité. Je vous le dis, en connaissance de cause, pour avoir participé activement au titre du sénat avec notre collègue Jérôme Bureau. Notre mission consiste à contrôler l'action du gouvernement à participer à l'amélioration de la loi, vous me permettrez monsieur le Ministre, donc de formuler de réserves à première relève de la prudence, cette loi est le fruit d'un long travail d'analyse et de concertation, nous en convenons tous mais je vous demande ici, solennellement, de veiller à son application trop de textes votés reste lettre morte faute de décret d'application pris dans un délai raisonnable, mais surtout de suivi concret sur le terrain et vous êtes un homme de terrain. Ma 2ème réserve porte sur le contenu du texte lors de nos échanges en audition par la commission des lois, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet, certes vous engagez judicieusement. La départementalisation de la police nationale, mais vous oubliez l'idée qui était pourtant présente dans le propos de la sécurité, de revoir la répartition territoriale des forces de sécurité intérieure, c'est pourtant une attente forte qui relève de la logique temporelle tant de certains élus que de nombreux acteurs silencieux du terrain. La répartition actuelle date du siècle dernier, depuis la délinquance et la criminalité ne sont plus du tout les mêmes, et dans tous les domaines d'appréciation concrètement cela consiste en une nouvelle répartition optimale des forces de sécurité intérieure, sur le territoire en étroite collaboration avec les maires, en vue de faire face à l'hydre du XXIe siècle qui est devenue la délinquance dans notre pays, mais alors, pourquoi un tel renoncement. Pour des raisons qui ne peuvent qu'être à contre-pied de l'intérêt général. Pour semblerait-il apaiser des craintes corporative d'intérêt plutôt particulier, voire sectorielles. Vous avez renoncé parce que, comme le font trop souvent de nombreux décideurs vous avez vrai simplement cédé et c'est mon opinion à la pression syndicale, monsieur le Ministre, notre devoir à tous est d'assurer la sécurité des Français de projeter des forces de sécurité intérieure dans l'avenir, la situation est grave, très grave, trop du territoire sont des territoires perdus des territoires délaissés des territoires sacrifiés de la République dorénavant l'incivilité, la délinquance, le crime, la barbarie frappe partout, y compris dans cette France rurale et périphériques cette ou Douce France, autrefois épargnées. Prendre des mesures justes, efficaces s'avère parfois difficile, car cela implique de combattre les lobbies et les habitudes et vous y êtes en plein dedans, mais c'est aussi à ceux-là qu'on mesure la pertinence et l'importance d'une réforme montrer Monsieur le Ministre que comme vos illustres prédécesseurs, Pierre Joxe et Charles Pasqua votre détermination ne s'arrête pas des attributions matériels techniques, logistiques et humaines, elle intègre aussi la notion de stratégie organisationnelle et fonctionnelle, vous le savez parfaitement, monsieur le Ministre, la répartition territoriale et vraisemblablement l'une des clés clés essentielles de cette très attendue Lopmi la repousser, c'est peut-être renoncer à l'espoir de voir les forces de sécurité intérieure prendre le dessus définitivement sur la délinquance sur la criminalité en France, nous restons pas dans le fond du panier derrière le Mexique ou la Malaisie dans le classement des pays basé sur l'indice de sécurité moyenne un BO cette loi est un 1er grand pas, ne vous arrêtait pas, nous le devons à nos concitoyens, nous le devons à nos forces de sécurité, comme nous le devons à nos élus de première ligne ou nos valeurs, je vous remercie. La discussion générale est Close, monsieur le Ministre, vous avez la parole pour répondre aux orateurs. Les. Merci madame la la présidente je vais et si on essaye de répondre aux orateurs en les remercions très sincèrement de de leurs critiques aussi leur encouragements j'ai j'ai donc noté un soutien si j'ose dire, de la majorité sénatoriale du du Sénat y compris de de ces groupes, comme le RDSE, si j'ai bien compris, le groupe de Monsieur Maluret, j'ai compris que le groupe socialiste interrogatif et souhaité que nous allions vers un sens d'écoute, je voudrais vous dire était vraiment la position du gouvernement et on aura l'occasion d'avoir un débat, je l'espère, le plus intéressant possible et j'ai compris que c'était un

Alors beaucoup de choses ont été dites. Soulignant notamment, soit des interrogations des amendements Véronique permettront d'y revenir plus largement, soit des manques que vous avez évoqués dans ce texte. aurait essayer de résoudre un paradoxe puisque le Parlement demande des textes de plus en plus courts et puis évidemment compte on traite pas l'intégralité du Champ politique publique, on dit : mais c'est pas assez long, ouais, très bien, je veux bien répondre à ces interrogations, tout en ayant pas de baguette de de de magicien. Peut-être aux 2 rapporteurs d'abord dont je voudrais remercier le le travail mais c'est un travail si je veux dire d'un continuum puisqu'ils ont travaillé ensemble sur la loi sécurité globale, finalement j'entends 2 interrogations de la part des rapporteurs, le 1er du du rapporteur de Bresse sur la la plainte en visio qui recoupe un certain nombre de de questions sur le numérique, la distance. Il est bien évident d'abord que pour le ministre de l'Intérieur, que je suis n'est pas question de remplacer à 100 pour 100 le réel par le visio-ou par le numérique, je suis très attentif et je voudrais oui aux amendements du groupe, notamment socialiste me semble-t-il, qui évoquait la possibilité de toujours laisser une possibilité papier concret, il sera adopté avec enthousiasme du ministre de l'Intérieur, c'est ce que j'ai fait, lorsqu'on a fait l'impôt à la source, ensemble, c'est ce que nous faisons quand nous faisons la y'procuration il y a toujours évidemment un accès en même temps au monde papier au monde réel pour l'utiliser comme vous l'avez dit, disons que je veux dire au rapporteur de Bresse pour l'avoir évoqué avec lui en étant un peu surpris de son amendement pour faire très vite, nous permettons aujourd'hui par la loi que vous voterez que demain, nous pourrons faire des plaintes en visio vous prendrez un rendez-vous avec un officier de police judiciaire qui soit gendarme qui soient policiers et vous pourrez déposer votre plainte de votre ordinateur. Et ainsi ne pas vous déplacer au commissariat, la brigade de gendarmerie, c'est quelque chose de très important parce que, aujourd'hui, plus personne ne comprend qu'il doit passer 2 à 3 ans dans un commissariat pour déposer une plainte que l'on peut qualifier de véniel, je me suis fait très dégradée ma ma mon véhicule. Je dois le faire absolument pour les assurances, parce que c'était un véhicule professionnel si nous allons ensemble dans un commissariat, que vous connaissez toutes et tous pour le visiter plein de fois en en allant voir les services de police ont donc ce sont des gens qui attendent depuis une heure et demie deux heures parce qu'il faut absolument qu'avant qu'repartent demain matin, parfois c'est des commerciaux, parfois c'est des gens qu'ont les horaires atypiques et donc très courageux, datant de 2 heures d'avoir un un policier en face de soi, c'est pas une police moderne. Pardon de de le dire au moment où on paye ses impôts à son numérique ou on peut commander, y compris on fait parfois de la médecine, de toute façon numérique, la police sera donc le seul endroit au monde où le papier serait toujours imprimer et le commissariat ressemblant à Gérard Jugnot dans Pinot simple flic, je, je pense que il faut que nous acceptions la modernisation d'une grande administration parce que le mystère, l'intérieur, c'est avant tout une grande administration. à vendre une illustration de Force républicaine alors. Aujourd'hui il y a déjà des pré-plaintes en ligne. Elles ne sont possibles que pour les atteintes aux biens. La peinte en ligne, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est 50 % des plaintes que va évoquer le policier ou le gendarme et notamment le policier dans les zones les plus urbaine, ça marche. On n'est pas obligé dans une organisation normal de pouvoir se dire que tout le monde doit passer encore physiquement au commissariat ou à la brigade de gendarmerie. Il faut passer de la pré-plainte en ligne à la plainte en ligne en laissant le choix à l'interlocuteur s'il veut venir physiquement évoquer son sujet ou si il veut le faire de manière numérique et personne ne comprend, encore une fois qu'on demande une demi-journée de congé à quelqu'un pour aller déposer une plainte lorsque son vélo. Non. Je prends l'exemple d'un commissariat parisien que j'ai visité il y a pas plus tard que quelques jours ou la dame qui a à la grippe, me dit : je me suis fait voler mon Vélib attendre une faire une demi demi-journée de congés, c'était le cas de la dame pour aller déposer plainte pour son Vélib ou du réclamer l'administration parisienne, ce qui est bien logique. Donc chacun comprend l'intérêt quand même sur certaines plantes de ne pas encombrer les pouvoirs. Les services de police, mais en même temps, de libérer la vie de nos citoyens. Et de concentrer les plaintes les plus graves, notamment les atteintes aux personnes notamment les violences intrafamiliales qui demande beaucoup de temps, évidemment et d'écoute. Pour pas se dire que, il y a un travail si j'ose dire, plus rapide à faire : que sont les dépôts de plainte lambda, on va dire ça comme ça, vous recevez des un mail hein, phishing qui vous demande, se faisant passer pour un petit cousine de l'argent envoyé dans un pays étranger, faut il avait passé 3 heures au commissariat de Tourcoing pour faire cela, alors qu'on pourrait très bien le faire de façon numérique alors la disposition dans lequel, pour lequel heures Daubresse ma. Mais interrogé c'est que lui il encadrer la vision qu'plaintes pour les biens. Et nous disons, nous discutons de l'ensemble des plaintes parce que. Il appartient sans doute peut-être au législateur de regarder davantage mais que les plaintes qui méritent des examens médicaux des questionnements plus intime des accompagnement psychologique méritent évidemment de se faire en physique. D'ailleurs, je voudrais dire ici pas en physique seulement dans le commissariat, nous faisons, nous expérimentons, on n'a pas besoin de mesures législatives pour ça le aller vers comme de la vaccination aujourd'hui les policiers gendarmes dans 10 départements de France vont chez l'avocat vont chez la maman vont chez la cousine vont CCAS vont dans la commune pour pour pas recevoir la dame notamment si c'est une violence intrafamiliale une agression sexuelle dans le commissariat, mais dont dont dans l'association venir prendre la plainte grâce au moyen qu'ont les policiers gendarmes pour faire des choses désormais à distance, mais il y a un certain nombre de plaintes, y compris qui touche physiquement les personnes qui peuvent être totalement déposé effectivement de manière visio à la condition qu'un certain nombre d'éléments soient réunis, notamment l'identité numérique pour qu'on soit certain que cette personne soit la bonne personne qui dépose plainte, donc on aura l'occasion d'en d'en parler, mais ça me paraîtrait absurde. Que seule l'administration de la police nationale et du et et la gendarmerie ne puisse pas utiliser le numérique pour simplifier la vie de nos concitoyens. Je dirais que dans l'absurdité parfois Center et le dernier, nous avons été les derniers à pouvoir faire voler des drônes en France, tout, tout le monde pouvait faire voler des drônes, sauf les policiers et les gendarmes. Grâce à la

le sénateur Hervé R RF, je veux dire que d'abord, le gouvernement a essayé de déposer le moins d'amendements possible et été parlementaire moi même je sors, je reviendrai sans doute un jour Ministre c'est très bien, mais, mais c'est pas un CDI, je voudrais dire, Monsieur le Ministre, Daubresse, monsieur le rapporteur Hervé que nous déposons 2 amendements gouvernementaux je voudrais non mais je veux dire que c'est quand même, je crois aussi, ah si positif vis-à-vis du travail parlementaire et notamment l'un des deux c'est la demande de la commission du Sénat que de transformer l'ordonnance en nous l'avons fait vous avouerez que c'était pas facile, nous l'avons fait et donc, c'est aussi pour ça que c'est un moment sera certes long mais respectueux, je crois, des droits parlementaires puisque nous renvoyons pas ça à une ordonnance alors beaucoup de questions ont été posées ensuite par les orateurs, j'ai essayé de les sérier, madame la présidente, mais gageons que ça fasse gagner du temps dans la discussion d'amendements si. Les parlementaires se sentent éclairée Madame Jourda et monsieur le roi à l'instant que je remercie de sa participation pour vous, la sécurité, comme le sénateur du évoqué la question de la répartition, police, gendarmerie, je sais que ça passionne absolument tout le monde et notamment les sénateurs particulièrement, il a encore plus que les sénateurs sont parfois en campagne électorale, ça peut arriver mon département et renouvelable je voudrais constater d'ailleurs qu'il y a quatre députés, 4 sénateurs du Nord

au sénateur le roi, j'ai dit à la rapporteure Jourdain se pose. Alors, elle n'est pas, à mon avis. Si difficile à faire, a priori, parce que, en fait, peu de textes législatifs. Viennent convoqué la répartition entre la police et la gendarmerie, si c'était un article, j'ai un article du code général des collectivités territoriales qui prévoit que, au sud, un certain nombre d'habitants, 20000, me semble-t-il, de mémoire en dessous, c'est une zone gendarmerie aussi, c'est une zone police et désormais, il y a quelques exceptions qui ne confirme pas la règle puisque par exemple si je prends le cas de Libourne est en zone gendarmerie, alors que l'augmentation de la population a été beaucoup plus forte. à votre argumentation et c'est. Pas les lobbies, monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur, pardon, qui m'ont poussé à ne pas proposer cette nouvelle répartition et donc je n'ai pas repris cette proposition, pas tellement du bobo si vous remettez mais plutôt du Livre blanc de la sécurité d'abord, si je rentre aujourd'hui dans une répartition, police, gendarmerie. Je fais naître à mon administration une discussion sociale extrêmement forte. Puisque c'est pas si simple que ça, les gendarmes dorment dans leur caserne, avec leur famille, les policiers ne vivent pas dans leur commissariat, donc c'est c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, et donc il faut des projets immobiliers, il faut un accompagnement social et nous allons passer des mois et des mois, et c'est bien normal à l'accompagner. Et deuxièmement, nous aurons donc une discussion avec les collectivités locales sur cette question un peu long et c'est bien logique. Je pense qu'au moment où la délinquance est forte, où nous devons organiser face aux crises que j'ai évoqué le ministère donateurs qui a pris beaucoup de retard sur le cyber n'a eu ton le terrorisme et organiser les Jeux olympiques, je ne suis pas certain que l'énergie du ministre de l'intérieur et de tous ces services doit être aujourd'hui se concentrer sur la répartition, police, gendarmerie, au niveau territorial, je ne dis pas que, ici ou là un certain nombre de choses ne le mérite pas, notamment en outre-mer, mais pas que je dis que, à choisir ses combats et je crois qu'ils sont nombreux dans ce que j'essaye de mener dans la priorité ce n'est pas la priorité première que j'ai souhaité mettre en place ici la priorité première c'est la lutte contre la délinquance, les premiers chiffre d'ailleurs dévoilé ce matin montre que la stratégie, on y reviendra de présence de voie publique apporte certain solutions 23 % de baisse de de violences aux personnes en moins par rapport à l'année dernière, c'est la première fois en 4 ans, qui ne se personne baisse bon, donc je pense que l'énergie doit se concentrer là-dessus et dans la réussite de Coupe du monde de rugby et des JO, donc plusieurs pour que vous évoquez est pas sur ce sujet qui est certes important, mais qui n'est pas le plus important. 2ème sujet : je me pose la question, Monsieur le Sénateur, madame la sénatrice de savoir si cette répartition territoriale posé la question n'est pas y répondre, je me pose la question en toute sincérité, n'est pas un peu daté. Est ce que la délinquance d'aujourd'hui fonctionne seulement par territoire, telle que nous avons connu, commune par commune. Est ce qu'on se dit pas que le territoire numérique qui fait naître une délinquance territoriale, les points de deal son numérique le dark web fenêtre une monnaie numérique. Des échanges d'armes se font sur un territoire numérique est-ce que ça ne vient pas un peu cassé les réflexions, il y a encore 20 ou 30 ans de la répartition, police, gendarmerie, les lieux de transport aujourd'hui, les zones de transports, si je prends l'agglomération toulousaine qui prend 15000 habitants par an, fait que les lieux de transport c'est un côté police côté zone police un côté gendarmerie côté gendarmerie et ce qu'on doit pas imaginer que la police aujourd'hui, il doit être compétente selon non pas des territoires, de délinquance, mais des thématiques de délinquance pour tu as tout à fait imaginer que la gendarmerie ou la police, ce spécialiste de l'intégralité des transports parce que on s'arrête pas une station de métro ou une station de bus parce que c'est, c'est quand même de la gendarmerie qui vont prendre la suite, je connais des rocades, d'autoroutes qui sont en zone police avec CRS et des et des autoroutes de cette même regarde qui sont gendarmerie zone, gendarmes mobiles et ce qu'on ne dit pas que c'est un peu absurde d'à l'heure où nous parlons d'imaginer en territoire poser la question n'est pas, ils répondent définitivement, mais je crois. Que cette réflexion n'était pas tout à fait, fait et renforcée par le premier argument que ce n'était pas la priorité du moment et ça laissera du travail pour les autres mises l'intérieur parce qu'après tout on ne peut pas tout faire en une seule fois, donc j'en suis, j'en suis très heureux, n'y voyez aucun conservatisme, monsieur le sénateur, ici, à la fois une hiérarchie des priorités et une réflexion sur ce qu'est la délinquance, je voudrais évoquer la question de la méthode sur des brigades de gendarmerie qui intéresse évidemment tout le monde, je suis surpris, Monsieur le Sénateur, Bourgi, mais c'était une invitation au voyage, finalement, vous disiez que les élus étaient inquiets pour leur proposer des brigades en plus j'avoue que. Je n'ai pas encore vu de pétitions des locaux pour me dire moins brigades de gendarmerie, mais dès qu'il y en a, je, je, je m'engagerai à ne pas maître de brigades dans ce département, si tout le monde le monde sans aucun doute, sans aucun problème, nous allons recréer 200 brigades de gendarmerie et je veux aussi souligner que nous c'est pas des promesses en peau de lapin, comme on dit dans le Nord, puisque nous avons la création de 52 % d'effectifs dans la police et 48 % dans la gendarmerie, c'est la première fois qu'a mise à l'intérieur propose à quasi-parité le nombre de policiers, nombre de gendarmes et s'est notamment fait parce que nous recueillons ces deux 200 brigade à peu près 10 militaires par brigade, évidemment, c'est une moyenne un peu technocratique de ça ne veut rien dire, ça nous fait quand même 2000 gendarmes prévu dans la loi de programmation dont une très grande partie des Budgets 2023 donc, dès l'été prochain, je suis capable de réouvrir des brigades de gendarmerie dans vos départements, et donc c'est vraiment extrêmement concret, comment nous allons faire, j'ai commencé dans le dans le Cher, mais je crois que des représentants de de évidemment de la haute assemblée était présente, nous réunirons tous les maires, tous les parlementaires avec le commandant de groupement de la gendarmerie avec le préfet et quand il le pourra, avec le ministre et nous dirons voilà la délinquance dans la zone gendarmerie de votre département, les forces et les faiblesses des difficultés, les brigades qui ont été supprimés, les augmentations de population, les augmentations de délinquance les les nouveaux, les nouveaux projets, voilà où nous pensons qu'il serait bon dans une zone définie où on peut, maître des brigades en plus entre 2 et 4 par département, si dans un département, il faut médecin qu'on en mettra cinq et dans les départements très urbain, je, je leur dis : voilà, dans les Hauts-de-Seine, sachant que c'est pas un département de gendarmes, vous comprenez que il y a pas de brigades de gendarmerie, donc évidemment c'est à la louche, mais centre de 4 ou 5 brigades par département et nous leur disons une chose suivante aux élus, voici ce que nous pensons, nous, comme expert de la sécurité, vous avez 3 ou 4 mois pour réfléchir entre vous, comme vous le souhaitez, notamment nous appuyant sur l'association des maires ruraux et sur l'association des maires de France départemental pour dire. Là c'est bien, mais là c'est pas très bien parce que on a des projets pavillonnaire, on a un projet économique qui arrive, il faut réfléchir pour les 20 ans qui viennent, et pas seulement à délinquance d'aujourd'hui et tout le monde sera consulté à commencer évidemment par les parlementaires et sur la double proposition des élus locaux et du commandant de groupement bah, nous ferons un certain nombre d'arbitrage. évidemment, mais je le dis pour les deniers publics, plus on aura des locaux disponibles, ce n'est pas du tout un chantage, c'est une évocation plus on aura des locaux disponibles, plus on pourra vite implanter ces brigades de gendarmerie mais ça commence par l'État, l'État a des vous locaux vides dans vos départements qui n'utilisent pas ou qui n'a pas rénové, c'est le cas de caserne de militaires. C'est le cas d'anciens endroits du ministère de l'Intérieur, mais c'est le cas aussi peut être d'un certain nombre de bâtiments publics concentration de l'État a fait qu'on a perdu des implantations et nous on est prêt évidemment à payer les rénovations et les aménagements, mais je ne vais pas non plus bouder mon plaisir, c'est une agglomération, département nous dit on a décidé d'aider une commune à avoir une brigade de gendarmerie flambant neufs, voilà donc on en reparlera parce que il y a des amendements, effectivement, moi je suis tout à fait prêt à allez les discuter, je suis évidemment pas d'accord sur le montant, mais j'ai aussi pris comme un comme elle comme un appel à à la discussion, en tout cas, je veux dire que c'est en parfaite discussion collective que nous ferons, c'est 200 brigades qui seront toutes annoncé au mois de mars prochain et, dès l'été prochain pour ceux qui seront prêts ne pourront créer ces brigades de gendarmerie puisque nous avons les effectifs pour Madame Assassi. Bon je, je, madame, j'ai pris votre intervention, d'abord par avec de vraies questions sur la formation, je partage votre opinion, mais c'est un texte formation il aura un peu, un peu plus motivation pour former les policiers et gendarmes, d'abord, nous sommes le gouvernement qui avait augmenté de 4 mois et c'est le cas aujourd'hui dans les écoles de police et les écoles de gendarmerie, la formation initiale des gardiens de la paix et des gendarmes avant il faisait 8 mois maintenant, il faut 12 mois. C'est pas mal, c'est une amélioration substantielle et sur la formation continue Madame il n'y a, nous avons 2 problèmes, un manque de formateurs de un manque de temps pour les forces manque de formateurs dans la programmation, je propose, c'est 250 formateurs recrutés en formation continue pas formation initiale pour la gendarmerie et 500 pour pour la police nationale, nous recrutons dans ce texte, 750 formateurs, encore faut-il former les formateurs et plus nous l'avons nous avons déjà commencé à le faire partir du principe qu'on aura quand même une majorité pour ce texte, il n'y a jamais eu autant de progrès. Pour avoir autant de lieux de formation et de formateurs dans la police et en gendarmerie, parce que je suis bien conscient de ce que vous dites et vous avez parfaitement raison, la formation permet d'aider les policiers et gendarmes à être respectueux des lois de la République et aussi protéger leurs propres actions juridiques oui mais ça, c'était un des quatre du Beauvau de la sécurité, je pense que les dessinateurs sénateurs qui ont participé ont pu traduire cette demande forte des forces. Et puis, ce que nous, on dit aussi les forces et que il y a des moments où ils ont des formations, il y a des moments où ils peuvent le faire selon ils peuvent pas le faire parce qu'ils sont rappelés par leur service au moment où je vous parle, je dois cinq semaines de congés payés aux gendarmes mobiles aux CRS. Là maintenant parce que nous les utilisions tout le temps. Quand c'est pas des matchs de football, c'est la police aux frontières qu'on s'est pas produire ces manifestations du samedi, quand c'est pas les manifestants du samedi, c'est une bassine qui, attaqué par je ne sais quel ultra gauche nous utilisons toujours on utilise on est hyper si personne ici se relève de l'ultragauche j'imagine donc ses renpas une attaque ad hominem. Nous utilisons beaucoup les CRS et gendarmes mobiles et donc pourquoi ils ne sont pas assez formés, c'est pas par manque de formateurs, c'est par manque d'effectifs et chacun sait qu'on rogne sur leurs congés et sur leur formation pour qu'ils aillent presque parer au plus pressé, c'est-à-dire l'ordre public qui font du coup un peu moins bien parce qu'ils sont fatigués parce qu'ils ne sont pas assez formés, le chat se mord la queue, donc la recréation dès 11 unités de forces mobiles après la suppression des 15 unités de forces mobiles, c'est aussi non pas maître forcément plus de policiers, de gendarmes sur le terrain mais permettez 3 tiers. Un tiers de repos, un tiers de formation, un tiers d'actions et donc là, je crois vraiment madame peut-être que c'était un mot d'explication de la part, mais je pense vous avoir convaincu, je ne vois pas sur la la victime à distance parce que je pense que je l'ai évoqué, à votre collègue rapporteur et vous même vous savez sans doute qu'il y a du bon sens à avoir sans doute dans l'utilisation de l'outil numérique pour ministère de l'Intérieur. Vous m'évoquez les BTS, mais c'est un très bon exemple, la police technique et scientifique, la police technique et scientifique aujourd'hui

il faut faire confiance aux agents. Technique, administratif et scientifique du ministère de l'Intérieur, les services de police ne peuvent pas été seul. De tous les services à faire des protocoles entre avant d'intervenir,

les gardiens de la paix, les, les, les gendarmes. Dans une école, ils vont, ils ont 19 20 21 22 ans, c'est les enfants du peuple, c'est pas les enfants du CAC 40 en général qui font, gardien de la paix, on peut le regretter, peut être, mais enfin c'est une vérité moi je ne veux pas opposer les forces de l'ordre à la jeunesse, puisque ce sont des jeunes. Qui rentre dans la police nationale et dans la gendarmerie et puis ce débat soit société on aura évidemment d'autres moments pour le faire, j'imagine, le remercier de, de, de, ses, de ses encouragements, si je veux dire comprendre évidemment ces interrogations, j'ai vu qu'il avait déposé des amendements, je regarderais bien volontiers, dire que par, par nature, j'ai du rapporteur, je suis très favorable à un moment qui a déposé avec l'autre rapporteur de votre mission d'information sur judiciaire, je viendrai sur la filière judiciaire, aucun sujet avec ça, oui, juste le corriger si il ne le permet, l'immigration n'a jamais été dans la première version de la Lopmi voilà, donc ça n'a jamais été le cas d'ailleurs, ça m'est parfois reproché mais la Lopmi était sans l'immigration il y aura un texte immigration et donc même dans la version initiale je ne sais pas quelle version vous avez eu en tout cas pas celle qui a été rédigé par le ministère de l'Intérieur, donc c'est une, c'est une bonne chose aussi ma madame veut rien, j'espère que je prononce bien vous évoquez

assistant ou assistante sociale, psychologique, je voudrais seulement faire remarquer 2 choses d'abord oui Monsieur Bourgi, je crois, et vous-même, je suis personnellement favorable à la juridiction spécialisée pour les violences intrafamiliales, comme le font les espagnols donc vous y voyez un soutien très fort du ministère de l'Intérieur, même si cela relève du ministre de la Justice, j'ai constaté quand même le 1er ministre avait évoqué ce sujet, et personnellement je m'en félicite et j'en suis je crois très heureux parce que ça aidera également les policiers et les gendarmes à agir avec des gens devant un contentieux spécialisé même si ils ont fait beaucoup d'efforts, il faut continuer à faire ses efforts de formation de continuité, donc j'y suis favorable 2ème question je voudrais qu'remarque avec vous que 30 % seulement c'est évidemment beaucoup 30 % de trop et qu'on se mettre méprenne pas sur mes propos des femmes ou des hommes, mais majoritairement des femmes qui sont tombés sous le coup de leur conjoint avait déposé une plainte ou vous avez fait un signalement aux services de police ou de justice ça veut donc dire quand même, bien sûr qu'on a très large encore amélioration à faire dans les services pour mieux accueillir la parole mais que ce n'est pas simplement au mieux former les policiers et les gendarmes que vous arriverez à résoudre le problème, vous, vous savez bien des violences intrafamiliales et surtout des féminicides comme nous disons aujourd'hui, il y a donc dans d'autres pans de la société, je pense, personnellement au monde associatif, au monde médical également des devoirs d'alerte qui ne sont pas forcément au rendez-vous, donc il faudra qu'on en parle, si vous le souhaitez, dans le cas de votre rapport, mais ne ne n'ayons pas aussi comme l'une de penser que seuls les policiers et les gendarmes pourrait résoudre par une meilleure formation 100 % des féministes, si bien sûr ils pourront réduire au maximum le le et je pense qu'on peut toujours faire mieux, vous le savez, j'ai pris moi-même des dispositions extrêmement forte, pour qui il est meilleur, même pas de de doute sur les policiers, les gendarmes qui prennent les plaintes, mais ce n'est pas l'Alpha et l'oméga bien évidemment de la lutte contre les violences intra-familiales, même si c'est une très important bien sûr, il y a pas de dispositions sur l'ordre public, comme vous avez évoqué, mais je crois que nous aurons une loi JO très bientôt, on aura l'occasion sans doute d'en d'en reparler Monsieur Ravier, je ne sais pas s'il est encore là.

ce qu'on l'avait mis dans la loi sécurité globale et et que le le Conseil constitutionnel nous a dit une chose très simple si vous allez plus loin dans les pouvoirs donnés aux polices municipales, il faut mettre les polices municipales sous l'autorité du procureur de la République. Bon, je ne connais pas beaucoup de maires qui souhaitent le faire s'il y en a qui qui soit, qui soit volontaire, qui n'hésite pas, ou alors il faut changer la Constitution, ce qui n'est pas l'objet de notre loi ordinaire aujourd'hui ce qui leur permet, dire monsieur ravi qu'il ait légèrement antinomiques puisque il voudrait donner plus de pouvoir judiciaire, la police municipale mais refuse que la police judiciaire se réforme. à mon avis un paradoxe sont actuel complexe et sur l'immigration Monsieur Ravier mais d'une autre manière que de Monsieur dur à dire que il y aura un autre discussion un autre moment, j'espère qu'on pourra en discuter avec avec Karoutchi a parlé comme d'autres de la réforme de la police nationale et je veux donc lui répondre comme au d'autres intervenants, d'abord, je veux dire, mesdames et messieurs les sénateurs, que j'ai évidemment conscience des difficultés des dérogation qui se pose. Comme toute réforme importante et c'est une réforme très importante, c'est une réforme tellement importante qu'elle a été pour la première fois demandé par mon prédécesseur monsieur Joxe. Alors ça ne rajeunir à personne mais Monsieur Jo s'était mis à l'intérieur en tout cas, au moment où il a fait sa réforme au lendemain de son 2ème passage à Beauvau, c'est-à-dire au lendemain de 1988. Et le 1er qui évoquait le fait quelqu'un ici a cité le grand migrateur, qu'il était, je suis tout à fait d'accord avec le sénateur, le roi en disant que la police nationale, travailler en silos. Alors, mais dans messieurs les sénateurs, il y a des moments où vous me dites vous n'écoutez pas assez le Sénat. Alors une fois qu'on écoute au Sénat, vous dites, vous allez trop vite pourquoi au fait cette réforme monsieur le Ministre, Karoutchi a eu 7 rapports depuis 25 ans, fait par des majorité sénatoriale différentes et, selon le consensus du Sénat avec un président et rapporteur de couleurs politiques différentes qui préconisait les 7 rapports les 7 derniers rapports sur la police, la réforme de la police nationale que nous mettons en place.

La police nationale de points, c'est le titre. Une institution fortement divisé, tandis que la gendarmerie nationale je ne dit pas autre chose, bénéficie d'une structure unifiée de commandement et d'un esprit de corps affirmé la police nationale souffrent de sa forte segmentation et d'un manque pas tant de cohésion qui pèse au quotidien sur des agents comme sur l'efficacité des services, une organisation peu centraliser éclatée entre plusieurs centres de commandement au niveau national comme au niveau territorial. Mesdames et messieurs les sénateurs, c'est ce que nous faisons. Que fait la gendarmerie nationale, si c'est d'avoir un commandement hé oui, bien sûr, une filière spécialisée qu'on appelle les. Si on les sections de recherche, pardon, je suis un peu fatigué, c'est pas encore la fête de mon anniversaire. Que de rendre rapport au général qui commande la région ah oui, non c'est pas départemental parce que la gendarmerie il peut pas toujours du sur une départementale de par son organisation. Mais la section spécialisée de police judiciaire, elle est saisie par les magistrats et ça fait 2 siècles que ça dure, les magistrats n'ont jamais évoqué le fait que c'était attentatoire à la séparation des pouvoirs que de saisir les gendarmes et les saisissent bien volontiers, que fait la préfecture de police, monsieur le sénateur Dominati que si c'était de fonctionner avec. un fonctionnement d'ensemble de commandement, le préfet de police il préfet de tous les services de police dans un, dans une zone de police pouvez le regretter mais qui fait 35 % de la délinquance et l'essentiel des affaires, ce que vous disiez le coeur de notre pays, c'est comme ça que ça fonctionne, il y a la direction, directeur de la police judiciaire qui rend compte au PP, mais qui, bien sûr, pour ce qui est de l'enquête répond aux magistrats et pas au préfet de police, c'est la police nationale que l'exception à la règle et non pas l'inverse. Alors bien sûr, il y a des interrogations, on peut toujours en discuter mais moi j'ai tendance à écouter les 7 rapports sénatoriaux. Alors Monsieur le Ministre, Karoutchi quand on dit que les rapports sont faits et que jamais le gouvernement applique une fois qu'ils les appliquent, on dit parce qu'il y a des gens et c'est normal qu'il pose des interrogations auxquelles il faut répondre, ils sont, ils sont pas forcément tous content je vous réponds : travaillons aussi ensemble si vous le permettez, alors pour répondre aux. Ministre Richard le calendrier est clair : il y a des élections professionnelles début décembre, moi je vais pas discuter de réformes en attendant que les syndicats sont en campagne, donc j'attends et c'est normal, donc j'attends que les policiers élisent leurs représentants syndicaux le 15 décembre quelqu'un parler des expérimentations puisque ça déjà c'est déjà passé en outre-mer, je regarde le sénateur de Mayotte, il pourrait peut-être témoigner du fait que la DTP malgré les difficultés de Mayotte, qui sont grandes et plus efficace en Guyane, même le procureur général en convient en Martinique et en Guadeloupe, c'est pareil, je reviens de la Savoie ou un un syndicat de police a fait son son congrès dans ce département, tout le monde considère que ça se passe bien dans ce département, il y a 2 difficultés dans d'autres départements, j'en conviens bien volontiers, je dis qu'on a, on a attendre ces expérimentations j'aimerais me recommande un rapport de l'IGA de l'IGPN et j'ai demandé que l'Inspection de la justice, il soit il y a 2 rapports sénatoriaux, un rapport sénatorial, un rapport de l'Assemblée nationale le 15 décembre j'aurais ce rapport, je demanderai aux syndicats de venir me voir nous discuteront de la réforme à ce moment-là on a Mendras ce qui doit être amendé. Mais ici, je peux vous dire qu'on ne peut pas rester dans un monde où on se réfère qu'à Clémenceau, qui était un grand personnage, dont bien sûr, je ne serais pas à la hauteur du petit doigt de l'orteil, je veux bien le dire, bien volontiers, mais même la Moussa, je ne vais pas à la hauteur, monsieur le monsieur le sénateur, Karoutchi mais depuis Clémenceau depuis Clémenceau, on a inventé la mondialisation aujourd'hui celui qui est à Dubaï, commande la drogue qui arrive dans le port du Havre de Marseille qui descend dans les points près de chez vous, on a abaissé malheureusement les taux d'élucidation et on ne peut pas se satisfaire de ce constat que tout le monde fait la Cour des comptes, les 2 chambres parlementaires les anciens directeurs généraux de la police nationale et se dire bon ben c'est comme ça, puis c'est tout. Ne changeons pas les organisations parce que Clémenceau inventé mais Clémenceau quand il a créé la police judiciaire qu'est-ce qu'il a fait, il a constaté qu'il y a un truc qui fonctionnait pas puisque la criminalité organisée, il a retiré la police aux pouvoirs municipaux mesdames et messieurs les sénateurs, voilà ce qu'a fait Clémenceau. Les les villes, les communes, les maires et les polices municipales ou alors vous avez beaucoup de manifestations, il a forcé. C'était le moins démocratique sans doute à l'époque, il a forcé à s'organiser, d'où la criminelle et il a dit devant une criminalité organisée, je fais une police organisée. Hé ben devant une criminalité numérique internationale multiforme qui demande désormais à ce que. La police des étrangers sont rien que la police judiciaire qui sont rien que la police de sécurité publique, qui sont bien que les renseignements pour pouvoir lutter contre les délinquances très forte que nous connaissons et que vous dénoncez à juste raison, il faut réformer la police nationale, par contre, tout le monde, pas de manière autoritaire, ça fait 30 ans qu'on parle de cette réforme, on en a parlé depuis Joxe, on en a parlé dans le livre blanc de la sécurité, je voudrais leur dire que ceux qui siégeait à l'époque, recommandé de faire cette réforme, on en a parlé au Beauvau de la sécurité, hé oui, au bout de trente ans, on se dit : ce serait peut-être bien de l'affaire, alors je veux rassurer ici les magistrats, ils auront évidemment toujours l'immense et entière responsabilité des enquêtes. Seuls eux peuvent donner des des aux policiers, aux gendarmes dans le cadre de leurs enquêtes, personne d'autre, pas le préfet par le directeur départemental de la police nationale, par le directeur général de la police nationale, ils ont le libre choix du service, selon l'article 12 du code de procédure pénale et évidemment les questions qui sont posées, notamment de probité, on fera monter les affaires d'un niveau local au niveau national puisqu'il paraît que les préfets et les élus par le sous-souvent de questions de cet ordre, je ne le crois pas, mais je veux bien prendre l'abondement et donc toutes les affaires de probité de la crise financière seront montés un niveau qui n'est pas départemental alors nous ce que nous allons continuer à discuter évidemment. Mais je veux vous dire que ce que nous faisons là n'est pas sorti des idées simples, du ministre de l'Intérieur, mais de 30 ans de réflexion sur pourquoi la police nationale doit se réformer, je le ferais évidemment concertation mais je voudrais dire aussi aux parlementaires, renier le débat que nous pourrons avoir, que ce ne sont pas des dispositions législatives. Et que nous changeront 176 textes réglementaires que nous l'avons mis par honnêteté dans le rapport annexé nous discuterons évidemment des amendements d'ailleurs en acceptant je crois la quasi-intégralité d'entre eux, mais il faut aussi savoir réformer lorsque réformer, je pense que c'est un ministre de l'Intérieur et merci d'avoir souligné qu'a jamais trouvé autant de moyens et qui défend je crois hormis étourdi les forces de l'ordre qui peut permet de leur dire parfois qu'il faut aussi se réformer en respectant profondément leur métier, leur filière et et leur action parce que la police a été créé pour les gens. Et pas pour nous-mêmes 2ème intervention sans doute plus critique, celle de monsieur alors ben Haroche, c'est bien ça. Voilà. Vous me dites, monsieur le sénateur, de ne pas faire d'amalgame politique facile. Ou quelque part en en mettant le vaccin ou l'antidote à, à ce que je pourrai pour vous répondent, c'est-à-dire effectivement pour améliorer, j'ai bien noté la souffrance au travail, le sens des métiers de la police, vaut mieux pas trop les insultez pas trop dire que la police tue ça aide aux policiers à aller mieux, je pense, dans leur action, mais vous dites, ne fais pas de politique d'amalgame. Je vais vous dire vous me traitez d'Orwell à la tribune de l'Assemblée s'est légèrement excessif, bon, d'abord parce que j'ai pas son talent littéraire et ensuite parce que je suis né en 82 et pas en 84 Oui, merci, monsieur le rapporteur. Mais je veux essayer de répondre à votre à vos critiques plus sur le fond d'abord, vous me dites : il faut créer une police environnementale, mais vous allez voter le texte, monsieur le sénateur, nous créons la première gendarmerie verte parce que la politique environnementale et sans doute une police de l'environnement en zone gendarmerie, la police, la gendarmerie verte première fois qu'on le traite. Et nous allons renforcer de manière très importante le Kleist l'office concerné donc nous félicitons-nous de de cette avancée très importante. Vous nous dites : il faut dénoncer le le le côté disparate des des AFD. Alors ça c'est un point très important, parce que dans votre intervention, vous avez dit, vous mettez en cause finalement, voici un peu la la réforme de la police nationale, vous nous dites

vu, dès que l'on mais c'est vrai qu'il y a des endroits dans le Val-d Oise monsieur le ministre Richard le nombre de grammes de cannabis qui fait naître l'AFD n'est pas le même qu'en Savoie parce que vous savez quoi, il y a un procureur qui le définit. Et c'est bien, non pas le ministre de l'Intérieur qui définit la politique pénale mais les procureurs de la République c'est pour ça, l'AFD respecte profondément l'indépendance des magistrats, une fois que vous aurez voté telle législation imaginons l'amende forfaitaire délictuelle pour la consommation de cannabis, une fois que nous l'avons voté c'est les procureurs de la République qui prennent une circulaire dans le ressort et qui dit aux services de police, la loi a dit ça, mais moi je dis que 15 grammes de cannabis, c'est très grave, et donc je faire et je demande qu'on interpelle, je monte la garde à vue, je vois la procédure et puis il y a des départements comment va doivent, on pense que 15 grammes de cannabis, bon, on en voit beaucoup, donc on préfère se concentrer à faire plus de 30 grammes en dessous de 30 grammes bah, on fait l'AFD, au sud de 30 grammes on on défaire mais c'est procureur qui décide, c'est pas le commissaire de police, le ministre de l'Intérieur, ou le gardien de la paix, alors parfois ça peut apparaît disparates les faut accepter que les procureurs ne répondent effectivement pas tous au milieu, la justice au ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, non il ne recommande pas évidemment les ordres de la place Beauvau, donc vous arrivez à défendre avant démonstration, monsieur le sénateur, à la fois qu'on doit laisser tout liberté aux magistrats et quand ce disparate selon les ressorts, vous dites il y a trop disparaît de de trop différence entre les ressorts la politique pénale, monsieur le sénateur n'est pas défini par le ministre de l'Intérieur, elle est définie. Par le garde des sceaux, mais surtout par les circulaires pénales parce que nous vous demandons, c'est rien d'autre que de permettre à à la sanction que de s'appliquer puisque les listes de délit que nous allons évoquer ne connaissent pas de sanctions, sauf le rappel, la loi qui n'est pas une sanction, au sens de nos concitoyens et quand quelqu'un fait un tag, personne ne peut accepter, bien sûr, qu'il aille en prison, ce serait absurde et même le code pénal prévoit malheureusement qu'il aille en prison, si j'ose dire, mais il faut qu'il ait une sanction. Parce que si y a pas de sanction quand on commet un tag, on aura, on appelle à la Halle recommencer. Donc le débat que nous aurons, monsieur le sénateur, c'est pas est-ce qu'on se substitue pas aux juges : franchement, je pense que c'est pas le sujet, le débat que nous aurons c'est et ce que nous considérons que les délits que nous évoquons mérite la contravention avec inscription au casier judiciaire sous l'autorité du procureur ou une procédure pénale, c'est d'autant plus vrai que celui qui a crée les AFD par sécurité routière ce sont des gouvernements de gauche. Si, si vous parce que les avis avant d'être créée sur le délit pénal tout court érotique très sur les délits qui était auparavant du délit pénal soit sécurité routière si vous n'aviez pas de permis de conduire, par exemple, vous pouvez-vous prendre une AFD naïve de sécurité routière, donc c'est pas un débat d'attente à la à la justice de notre pays, c'est un débat d'efficacité, de simplicité, je pense qu'il ne faut pas mettre des des bovidés bah si vous permettez, ce ce point de vue là où ils ne sont pas. Monsieur Bourgi alors évoqué les la les FIP et d'ailleurs, j'étais très étonné de votre intervention, je sais pas ce qui se passe dans l'Hérault, j'ai demandé au préfet Moutou rapidement, ce qui fait de son argent parce que, en 2022 il y avait 5 millions de plus

Et dans le budget 2003, c'est 5 millions de plus et sera 5 millions chaque année de plus donc je vais regarder ce qui se passe dans l'Hérault et et je, je, je vais donc m'étonner auprès du préfet moto que vous ne soyez qu'on ne vous répondent que il y a plus d'argent, parce que malheureusement si j'ose dire. De ce point de vue, l'argent il y en a, et je demande plutôt aux élus de le dépenser,

je crois que vous les connaissez très bien, vous qui êtes du département du Rhône, hein ça bon, donc je suis très heureux que dans le groupe socialiste des gens me demandent des caméras de vidéoprotection donc ce que je je trouverai de l'argent évidemment pour tous ceux, socialistes qui demandent des caméras de vidéo-protection. C'est normal. Sur les Lapie là, puis vous avez parfaitement raison, alors c'est tout à fait réglementaire, moi je m'engage à ce que les maires puissent obtenir la compétence sur les tapis, c'est un tout petit peu plus complexe regarde monsieur votre représentant la CNIL Monsieur Hervé ce que je pense que c'est plutôt s'il me permet de lui qu'il faut comprendre que moi, mais évidemment c'est réglementaire ont, je vais essayer, je vais essayer, c'était une interpellation sympathique que monsieur le rapporteur, je vais essayer de vous répondent ici la 2ème la 2ème 2ème retour, vous m'avez évoqué des brigades de gendarmerie mais je pense que je vous ai répondu également vous avez pas les effectifs, je crois que, à Montpellier, ils peuvent pas se plaindre des effectifs que le ministre de l'Intérieur accorde ne semble-t-il parce que, effectivement, il faut travailler pour lutter contre contre la délinquance, je terminerai, madame la présidente, puisque je je je vous imagine impatiente, c'est sur les propositions, en tout cas les interventions de Monsieur Wade et de monsieur Dominati. Pour Monsieur Mohamed, il a dit quelque chose de très juste parmi toutes les choses qu'il l'a dit et je reviens pas sur la PJ puisque j'en ai parlé, il dit voilà les conditions matérielles, c'est très important, et jusqu'à présent c'était pas super.

et je me doutais que ça pouvait pas bien marché parce que si vous augmentez ses effectifs et des moyens humains. Y compris d'ailleurs en rémunération, mais vous ne l'accompagnait pas ça de moyens technologiques matériel le commissariat de brigades de gendarmerie de véhicules évidemment qui qui est, qui a une distorsion et on a tous fait des tours avec les policiers ou les gendarmes avec la voiture qui avait quasiment là le fil de fer qui sortait aujourd'hui, je ne dis pas que c'est pas que c'est le cas partout, mais je pense qu'ils ont vu l'énorme effort que nous avons tous consentir grâce à vous, en mettant dans le plan de relance, la police, gendarmerie, ce qui était pas évident au début des cinq mille huit ans sont je crois la plus belle vitrine mais c'est pas vrai que pour les 5008, c'est vrai pour l'ensemble du matériel, je peux faire le détail du bilan du quinquennat précédent mais ce que nous essayons de faire, et la loi que nous présentons. Une stratégie budgétaire ce qu'il faut que le T2 augmente autant voire moins que le haut et de et je veux redire ici. Ah la. Représentation nationale que c'est le 1er, texte qui prévoit plus de crédit. Qui n'est pas de personnel et qu'il y ait de matériels et technologies c'est la première fois que nous osons dire aux policiers, aux gendarmes, bien sûr, on crée des postes, bien sûr, on peut imaginer un certain nombre d'augmentations de rémunération, ce que nous faisons, mais ce qui est important pour vous, c'est le rattrapage technologique matériel et les les casernes, les brigades les commissariats que nous devons rénover recréer mutualiser plutôt que toujours de donner un chèque de plus voilà et ça je pense que c'est très important parce que c'est la stratégie budgétaire qui est d'ailleurs, c'est 15 milliards. et vous devez être convaincu, Monsieur le Sénateur que quand je vous dis que sur les 15 milliards, il y en a 7 à 8 qui sont sur le numérique et le cyber ça paraît pas évident pour nos concitoyens, parce que ce qu'ils veulent, c'est ici et maintenant, des policiers et des moyens matériels, les policiers veulent ici et maintenant des moyens matériels, mais nous, nous pensons que pour les aider à gagner demain la bataille contre délinquance, c'est ce qu'évoquait le sénateur Karoutchi nous devons éviter de prendre un train de retard comme d'habitude. Rattraper simplement par le numéraire, ce qu'on n'arrivait pas à leur donner comme matériel et moi je, je souhaite que cette loi marque aussi un changement dans la politique budgétaire du ministère de l'Intérieur et qui prévoit, comme dans l'armée que le matériel est aussi important que les moyens humains, c'est pour ça que nous essayons de faire notre programmation enfin monsieur le sénateur Dominati je terminerai par là parce que je crois que Monsieur Le Roi a eu, a eu sa réponse. D'abord, ce sénateur Dominati, vous avez eu la gentillesse de rappeler qu'on était peu de chose puisque je suis le 7ème ministre en 7 ans. Bon, alors quand je suis arrivée au ministre, l'intérieur, les syndicats de police m'ont dit : vous savez, les ministres pas ces syndicalistes reste. C'était un mot vraiment très sympathique, j'ai déjà vu 4 départs de responsables syndicaux depuis que je suis là, donc je commence à faire des congrès syndicaux pour dire : vous savez, les syndicalistes des ministres, il se trouve que sur 7 ans je, je, je suis quasiment fait 2 ans et demi. Donc votre formule était belle mais mais peu juste. Dans trois mois et demi, me semble-t-il, j'aurai atteint le niveau de vie de monsieur Cazeneuve. Si je termine l'année 2023 j'aurai dépassé celui de monsieur Et si je vais jusqu'aux Jeux olympiques, j'aurais été au niveau juste en dessous de monsieur Marcelin. Qui a très bien connu, le sénateur de Brest, je crois, c'est la tendance quoi. Tout ça pour vous dire que je suis d'accord avec vous qu'il faut durer et endurer sans doute au ministère, l'intérieur et durer pour faire des des réformes en profondeur. Et moi je suis très heureux que le président de la République n'est pas confirmée au ministère de l'Intérieur pour le principe d'être ministre, mais pour enfin mettre du temps long au ministère de l'Intérieur, parce que la moyenne et mis intérieur pendant ces 7 dernières années, ça a été moins d'un an, vous ne pouvez pas faire des réformes structurelles, vu l'actualité vue d'urgence que traite un ministre de l'Intérieur, si vos directeurs votre personnel Bercy dans son éducation est persuadé que vous allez passer vite, donc moi je souhaite je ne je ne dépends et je ne suis pas propriétaire de mon poste mais plus longtemps, je resterai plus autant j'essaierai de porter des réformes qui permettent de voir loin et de transformer fondamentalement la police, alors je sais que vous évoquez de grandes réformes, l'une que nous mettons en Une de notre programmation et l'autre que nous mettons pas le doublement de la présence. Policière et gendarmes sur le terrain, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est très important parce que je crois que c'est le coeur de notre discussion aujourd'hui si on sort le cyber. Ce n'est pas le doublement de la présence du nombre de policiers ou gendarmes. C'est le doublement de la présence policière. Il y a des effectifs en plus, on vous en a demandé 10000 dans le quinquennat précédent dont 4000 sont partis au service de renseignement. donc, à peu près 6000 seulement si j'ose dire, dans les forces de police et gendarmerie, nous vous en demandons 8500 pour le quinquennat suivant, il est sûr que plus de policiers, gendarmes, c'est plus de présence sur la voie publique, mais ce n'est pas suffisant. Comment nous allons doubler la présence de voie publique d'abord, nous allons faire faire des efforts aux policiers et gendarmes sur leur taux horaire. Et c'est ce que vous avez souligné monsieur le sénateur, nous avons mis fin au cycle dispendieux de la police nationale, où les policiers étaient moins présents sur la voie publique, parce que finalement il y avait une sorte. D'accord, on n'arrive pas à régler vos problèmes matériels, on n'arrive pas à régler pour la délinquance du coup on accepte que vous soyez moins présent sur le terrain, sorte de deal social qui était négatif pour tout le monde, nous avons mis en place un système qui fait que là où il fallait hein 8 policiers pour, qu'en est un, sur la voie publique, maintenant il faut 7 policiers pour qu'on sur la voie publique, ça vous paraît peut-être déjà trop peu, mais on a fait un effort dans tous les commissariats de France désormais, nous sommes passés. à ce qu'on appelle le rythme binaire. Améliorer par tel ou tel endroit dans quelques commissariats. La 3ème des choses, c'est les réserves. Ce qui marche admirablement bien pour la gendarmerie nationale n'existait pas pour la police nationale. C'est un excellent sujet police-population. Que des boulangers, des ouvriers, des. Encadre des petits patrons, des grands patrons, des moyens patrons aillent passer quelques jours sous l'uniforme, après une formation pour travailler dans la police nationale et de temps en temps aussi ben leur apportent expérience de la vie professionnelle de la société civile. C'est la réserve, soit la création de la réserve de la police nationale qui est une énorme avancée pour la police nationale soit et ça a été dit tout à l'heure à la tribune par la commission de la défense, je le dis devant le rapporteur de la commission de la défense qui s'est exprimé tout à l'heure, nous allons sanctifier les crédits de réserve. Qui, par manque de bonne cohésion budgétaire faisait qu'au mois d'août septembre vous commandant de groupement, on n'avait plus les moyens d'avoir de la réserve, puisque c'était des crédits les plus facilement annulables et c'est ce qu'on faisait votées dans le PLFR désormais grâce à la loi que je propose 100 % des crédits de réserves seront gelés au sens où ils ne pourront pas être justement dégeler et ça contribuera évidemment à la présence au doublement de la présence quatrièmement la simplification de la procédure pénale, mesdames, messieurs les sénateurs, en 2 ans, on a fait une réforme sans doute que vous ne voyez pas de manière considérable, on ne fait pas la une des 20 heures mais c'est ce genre de téléphone, ceci est un iPhone, j'en suis désolé mais d'une d'un Tél néo-cons désormais tous les policiers tous les gendarmes sur eux fabriqué d'ailleurs par une entreprise française, une PME d'Aix-en-Provence que je que je vous demande de de promouvoir grâce à cet outil, ce qui n'était pas le cas lorsque je suis arrivée au ministère de l'Intérieur, il ne l'avait pas tout c'est pas dans ces conditions, les policiers gendarmes ne retourne pas à la caserne ne retourne pas au commissariat pour regarder le fichier.

désormais, ils font tout grâce tous grâce à leur téléphone individualisé et le réseau radio du futur, mesdames, messieurs, ce sera la radio sur ce téléphone là où vous voyez les gens qui ont une grosse radio quand ils vous accompagnent pour ceux qui sont en filature, c'est très pratique dans une grosse radio quand on fait une filature en civil dans un an, c'est fini et tout sera sur ce téléphone et on y verra des images de radio en même temps que le son de radio et l'ensemble de la police et de gendarmerie et peut-être demain des pompiers et peut-être demain des douanes ou admiration pénitentiaire aura le même réseau donc en faisant ce genre de simplification qui ne sont certes pas la une de tous les journaux nous permettons plus de présence de voie publique pendant qu'ils sont pas au commissariat en train de vérifier les fichiers, ils sont sur la voie publique évidemment la procédure pénale a son importance et je veux dire à l'ensemble des sénateurs qui vont interpeller sur la procédure pénale, nous faisons-nous de la petite procédures pénales simplifiées va venir au moment du garde des Sceaux, le président de la République, il l'a dit pendant le cadre du Beauvau de la sécurité va a demandé qu'on simplifie, par exemple, l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance en seul cadeau d'enquête, c'est un travail de temps gagner considérable pour les services de police dont je voudrais vous convaincre monsieur le sénateur que le doublement de la présence policière, elle est fondée sur une vraie stratégie budgétaire de la programmation et de transformation du ministère de de de l'Intérieur, alors pourquoi nous ne réformons pas la préfecture de police, bon, faut-il réformer la préfecture de police pour, je sais que vous vous dites : oui, la préfecture de police, vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, date de son histoire, sans faire de mauvais jeu de mots tautologique, à Paris, le maire n'a pas le pouvoir de police, quand les autres maires, faut-il lui donner, c'est une réflexion que le Parlement doit avoir, mais Paris ce n'est pas n'importe quelle ville d'abord c'est une ville où il y a tous les lieux de pouvoir, à commencer par votre assemblée et c'est une ville qui connaît rien que la Ville de Paris, 23 % de la délinquance de toute la France, quand vous tenez la délinquance à Paris, vous tenez une grande partie de la délinquance, faut-il donc des moyens exceptionnels pour un endroit exceptionnel, j'ai plutôt tendance à répondre oui, bon 2ème sujet : faut-il, mais j'ai répondu à une question d'actualité de votre à votre demande, monsieur le sénateur, faut-il entamer la réforme difficile de la préfecture de police, au moment où nous devons gagner la victoire contre la délinquance qui est très forte à Paris, songez que cet été au 14 juillet il y a eu plus de voitures brûlées à Paris qu'il y en a eu, en Seine-Saint-Denis, ce qui montre, c'est un changement, me semble-t-il, de l'urbanisme et de la politique parisienne, mais je ne fais que constater moi qui regarde les choses de manière non politique au sens électoral du terme et ça doit poser des questions à un certain nombre de, de, un moment, nous allons organiser les Jeux olympiques. Je ne suis pas certain qu'il faut bousculer le fonctionnement certes originale, mais quand même, performant, la préfecture de police pendant le moment où nous allons organiser les Jeux olympiques 600000 personnes pour la installer une ouverture ah vous me direz, il y a toujours un moment où faut pas réformer bon

Je survis. à la Haute Assemblée. Ah ces rapporteurs. Aux chiffres de la délinquance aux aléas que le ministre de l'Intérieur peut connaître qui tous les jours s'accumulent sur son bureau. à la dissolution de l'Assemblée nationale. à la réussite de Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques et qu'en septembre 2024. Monsieur le sénateur Dominati, vous me dites, Monsieur le Ministre, après la Loki après la baisse de la délinquance, après la réussite de la Coupe du monde et les JO, quel chantier ouvrez-vous peut-être que j'aurai une réponse différente. Merci, monsieur le Ministre. Je vais suspendre la séance pour quelques minutes, la séance est suspendue.

La séance est reprise alors à l'article 1er nous avons plusieurs de de demandes de parole, à commencer par monsieur Laurent Burgo a, pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous abordons ici un sujet qui m'est cher et qui peut désormais concerner un grand nombre d'entre vous, l'été dernier, a une nouvelle fois démontré que le réchauffement climatique est bien une réalité et que l'intensité du risque de feu s'accroît d'année un année partout en France et en Europe par le haut niveau de technicité de ses hommes comme par la qualité de ses équipements et superstructures, la base aérienne de sécurité civile de Nîmes-devrait naturellement s'inscrire comme le Centre d'expertise et opérationnel européen Monsieur le Ministre, ce européen positivement gravé dans votre texte sera la possibilité d'accélérer les synergies, les coopérations entre elles différents acteurs : c'est un signal fort pour notre pays et pour notre continent, c'est aussi un signal attendu par le territoire Denis métropole très investie par le projet européen Nemo ZUS cette échelle continentale inscrite dans votre texte trouverait Avantage à l'évolution du mécanisme européen de protection civile vers la création d'une véritable agence européenne sur notre base nationale dans les semaines qui viennent, ni métropole recevra du ministère des Armées la propriété de l'aéroport pour mieux porter encore cette dimension continentale dont a besoin l'oeuvre de sécurité civile, Monsieur le Ministre, il faut continuer à défendre ce projet, la France en a besoin l'Europe en a besoin et le Gard sera y apporter une réponse positive, je vous remercie. Si Monsieur Burgot, hein, la parole est à monsieur Philippe Tabarot pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le Ministre, messieurs les rapporteurs cet article 1er sur l'approbation du rapport annexé décrit les projets qui seront conduites par votre ministère, à partir de 2023 on peut saluer les avancées de cette loi de moyens notamment grâce aux apports du Sénat en commission, ça a été largement dit, tout comme je souhaite tout de même décrié les habits de cette loi d'absents cette carence sur le sujet de la sécurité dans les transports, en effet, elle n'apporte que trop peu de réponses aux 122170 victimes dans les transports en commun en 2021, un cap a été franchi, non seulement dans le degré de violence mais aussi dans leur périmètre, il y a bel et bien une violence dans les transports en commun, comment comprendre que rien de tangible ne figure dans cette loi sur la sûreté dans les transports, j'ai déposé des amendements, co-signée par plus de 70 collègue avec des propositions qui n'ont malheureusement pas passer le filtre de la recevabilité, signe d'une loi beaucoup trop restrictive pour éviter des discussions interminables, et je vous cite concernant la fraude, comment expliquer, par exemple, à nos concitoyens qu'un voyageur contrôlé pour absence de titre de transport dans un TER pour la 30ème fois puisse continuer à narguer en toute impunité, les agents de sûreté dans les transports, comment expliquer à nos concitoyens que pour la surveillance des vols à la tire dans un métro, les agents de sûreté ne puisse réaliser des palpations préventive que dans certaines stations, et pas dans d'autres, devenus de véritables refuges pour certains délinquants comment enfin expliquer à nos concitoyens que ces mêmes agents de sûreté ne puisse interdire l'accès en gare à une personne ayant il a un comportement dangereux susceptible de menacer leur sécurité, j'avoue ne pas comprendre pourquoi on s'abandonne à cette fatalité véritable preuve d'indifférence ou même pire, de renoncement. Si cher collègue, la parole est à Madame Nathalie Delattre, madame la présidente, vous avez la parole. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, je souhaitais à ce stade, mettre un focus sur 2 sujets, la gendarmerie et la formation, les gendarmeries sont le maintien de l'ordre dans nos territoires et dans nos communes rurales, notamment dans un contexte de montée de l'insécurité des violences aux personnes, aux personnes dépositaires de l'autorité publique et des élus, des tentatives d'implantation de nouveau points de deal en ruralité, l'annonce de la création de 200 brigades de gendarmerie est la bienvenue, tout comme celle de la construction de nouvelles casernes sans oublier la réhabilitation de locaux vétustes en effet un bon équipement valorise et motive les gendarmes dans leur quotidien et les conforte dans leur entourage lorsqu'ils vivent en caserne avec leur famille, j'ai l'exemple de l'inauguration récente de la caserne de Pineuilh en Gironde il faut implanter de nouvelles brigades notamment dans les territoires qui connaissent une poussée démographique comme la Gironde, j'espère qu'en baisse en fera partie de souligner et saluer aussi la possibilité pour les élus de disposer de brigades itinérante qui va dans le bon sens 2ème point la formation continue, qui est encore trop négligé un nombre important d'agents ne font même pas une formation par an, il est nécessaire d'inscrire dans la loi une exigence de périodicité, c'est ce que j'avais rigide, rédigé dans un amendement déclarée irrecevable, malheureusement, car la formation continue peut concourir à garantir l'adaptabilité des forces de sécurité intérieure et l'efficacité de ces interventions, je vous remercie. Merci, cher collègue, et enfin la parole est à monsieur Laménie. Pour le groupe oui merci madame la présidence, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, quelques mots concernant cet article 1 qui suscite beaucoup de d'amendements et notamment sur les priorités qui sont liés à la sécurité intérieure, vous l'avez rappelé monsieur le Ministre, notamment la lutte contre la cybercriminalité, notion de sensibilisation, de prévention et vous, vous avez insisté sur la la proximité au niveau des forces de sécurité, notamment la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie du département des Ardennes, qui a un département frontalier au même titre que le département du Nord, notamment, s'est vu aussi bah c'est des dernières années, malheureusement, avec des suppressions de brigades de gendarmerie, j'ai en mémoire, je suis toujours objectif il y a quelques années, c'était en 2010 et 2011 il y avait la loi Loppsi 1 Loppsi 2 sur lequel aussi il y avait eu des avancées significatives les forces de sécurité aussi mais mérite beaucoup de respect, de reconnaissance, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, le statut militaire, les militaires aussi qui joue aussi un un rôle important et je crois que la notion de proximité est fondamental, rouvrir des brigades, je crois que c'est réellement important avec ce maillage du territoire, les violences intrafamiliales, vous l'avez aussi largement évoqué avec la la nécessité de postes aux créations de postes d'intervenants sociaux, la coopération opérationnelle entre les 2 forces, la place de la réserve opérationnelle au niveau gendarmerie et police sont aussi fondamental, n'oublions pas non plus les revendications légitimes aussi de l'ensemble des forces de sécurité et ma question c'est aussi recruter des des jeunes gendarmes et des policiers n'est pas simple et je crois que c'est aussi un un rôle important de lien avec l'Éducation nationale, mais néanmoins je suivrai le pour voter cet article 1 qui mérite aussi beau qui a mérité beaucoup de réactions mais aussi beaucoup de travail, merci. Merci monsieur Laménie alors, nous passons à l'examen des amendements et nous démarrons par le 174 présenté par Madame, la présidente à. merci madame la présidente, donc c'est un amendement qui demande la suppression de cet article 1er et nous plaidons donc pour cette suppression l'avoir dit, lors de la discussion générale, nous portons une ambition particulière, c'est celle de recréer restaurer le lien de confiance entre la population et la police et de garantir la sécurité des biens et des personnes, mais également celle de nos forces de police, donc nous pensons que cette ce ce, ce rapport s'ne ne répond pas à cette à cette ambition et je voudrais simplement préciser que notre groupe, c'est ne pas s'enfermer dans des postures de Roger et nous l'avons démontré en déposant un certain nombre de propositions de loi et une à laquelle je suis très attaché, c'est celle qui vise à réhabiliter la police de proximité qui, selon nous, pourrait répondre à un certain nombre d'ambitions et particulièrement à à s'installer dans la prévention, la dissuasion et ensuite la répression ce n'est pas ce que nous retrouvons dans ce rapport et c'est la raison pour laquelle, laquelle nous demandons sa suppression. Merci madame Assassi, monsieur le rapporteur, avis de la commission. Alors avis défavorable, c'est un amendement de suppression, contraire à la position de la commission et qui nous priverait de, de, d'un débat très intéressant sur la centaine d'amendements qui suivent défavorable.

Merci madame, c'est une définition, un petit peu de nos doctrine en matière de police de proximité, les objectifs développés dans le rapport annexé au pour but 1er de renforcer la présence des gendarmes, des policiers sur le terrain, remettre du bleu sur la voie publique sur l'expression d'Emmanuel Macron mais quelle sera la réelle mission du policier, le policier sur le terrain sera-t-il un nageur verbalisateur dans la première mission sera de sanctionner de constater les infractions de verbaliser d'écarter les personnes indésirables sur la voie publique, alors même que la relation entre la police et la population des pas apaisé, il y a dans ce rapport, aucune contrepartie aucun contrôle qui permettent de s'assurer d'un équilibre entre l'exercice des missions de sécurité suivi des missions sociales des agents des forces de l'ordre ni aucune perspective d'amélioration des Liens entre la population et la police police crédit très clairement que le ministre Darmanin déploie plus d'officiers sur le terrain, dans une logique exclusivement répressive, le malaise de la police parallèle à celui de l'institution judiciaire s'accroît d'année en année il est il y a plusieurs facteurs qui s'entretiennent et se renforcent mutuellement la dégradation des conditions de travail, à travail axé sur la politique du chiffre et du résultat des locaux de travail vétuste, l'augmentation du nombre d'Alter vention, un management 18 confiance rompue avec les citoyens solide réforme d'ampleur modifiant les prérogatives et missions des polices permettra de revaloriser les métiers, le groupe écologiste appelle de ses voeux une grande réforme pour instaurer une police plus territorialisée, s'appuyant sur la connaissance de son terrain tout en répondant au sentiment d'insécurité des habitants, nous voulons une police au plus près de la population et qui produit de la confiance, une police qui soit en contact permanent avec les bailleurs sociaux, les maires, les associations de résidents et de quartier, comme l'a indiqué la Cncdh dans son rapport sur les Liens entre la police et la population, l'instauration d'un climat de confiance entre les habitants et leurs police notamment dans les quartiers défavorisés s'avère plus efficace sur le long terme qu'une approche exclusivement répressive pour prévenir des incivilités de la petite délinquance en ce qui concerne l'accueil des usagers, le livre blanc de la sécurité intérieure, reconnaissez

Monsieur Bénard Roche c'est le longuement de la CDH pour écrire son amendement, je lui avais dit en commission que sur une partie de ceux qui le souhaitent, c'est tout à fait possible de le prendre, mais il y a des priorités proposées qui sont très problématique, on y reviendra d'ailleurs dans le dans le débat ultérieur, développement de mission sociale par la police, remise de récépissé en cas de contrôle d'identité, interdiction de verbalisation distance donc avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre.

je vous cite. Le gouvernement refusera tout usage du pouvoir de verbalisation à d'autres fins que celles prévues par la loi. Si vous connaissez des verbalisations qu'on ne fait pas selon la loi de la République ou lesquels ça veut raison de dire que les policiers mais des variations alors qu'ils n'ont pas de soutien réglementaire ou législative pour cela, c'est quand même très étonnant. Les pratiques de contrôle une entité des organisations seront évaluées à l'aune de leur impact positif ou négatif sur la confiance, ça serait plus et la population le gouvernement restreindra les possibilités de contrôle identité je veux dire que en fait en France ne contrôle d'identité que sous l'autorité judiciaire. On ne fait pas de contrôles d'identité sans l'autorité judiciaire, soit parce que des réquisitions, soit parce qu'il y a des policiers qui ont des OPJ qui sont habilités par les magistrats donc en fait je pense que votre sujet principal, c'est vous, vous n'avez pas confiance dans les forces de police et les forces de police et gendarmerie, vous savez, ils sont formés, ils n'ont pas la même parole que celle de n'importe quel citoyen parce que leur parole et et supérieur du fait que ce sont effectivement des auxiliaires de justice et je pense que vous parliez de souffrance au travail de conditions vous savez la la Pierre de souffrance au travail, c'est quand on on a beaucoup de suspicion de la part des personnes qui sont sous votre sous votre autorité et moi je pense qu'il y a beaucoup de exigeante qui serait assez blessé de lire votre amendement. Merci, monsieur le Ministre, c'est un avis défavorable, ah pardon, explications de vote. Excusez-moi, ma petite explication de vote d'abord si vous étiez si vous êtes choqué, je suis effectivement très choqué par vos propos, ça ça ne résume absolument pas dans le passé, monsieur Darmanin, je me suis pas permis de résumer la vôtre d'une façon aussi caricaturale, je me permets de vous le dire, donc je je précise qu'en fait que la solution que nous présentons avec nous proposant ça qui consiste dans la création de. Programme local permettant d'identifier les besoins et les attentes des usagers établie entre les habitants et les forces de l'ordre ayant comme aussi critères la satisfaction des usagers concernant leur accueil avec une évaluation, c'est pas une défiance monsieur Darmanin c'est une manière de sens au travail et de faciliter ensuite la confiance et le bien-être au travail des policiers également moi je ne le vois pas comme une défiance et beaucoup de policiers ne le voit pas comme ça non plus, il est essentiel que le gouvernement reporte les missions de la police et les pratiques actuelles décrié, entre autres, par des associations, pas que la Cncdh nous le fait penser la police et le représentant le plus accessible de l'État et des pouvoirs publics, monsieur Darmanin il se doit, elle se doit d'être le reflet des valeurs de notre République, d'autres sont en que je peux vous rappeler, mais que vous connaissez aussi bien que moi si c'est mieux l'évaluation de l'impact des pratiques policières dont vous venez de parler sur la qualité de la relation police-population est est un angle mort, et un impensé de votre politique, monsieur le ministre de l'Intérieur, dès lors, les membres de notre groupe, appellent de leurs voeux une véritable prise en code des choix politiques du ministre de l'Intérieur, au regard de leurs conséquences sur la relation entre la police et la population, nous vous rappelons également que le renforcement de cette confiance n'est pas seulement au service des citoyens mais qui va permettre d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie, certaines pratiques policières ne font que renforcer la dimension répressive du travail des agents et pour ta tête à cette relation entre la police et la population, entre autres, les contrôles d'identité ou les verbalisation systématique dont vous venez de parler les les contrôles d'identité représente une des principales occasions d'interaction entre les forces de l'ordre et certaines catégories de la population à la source de ces tensions, voilà je pourrai prolonger mais je. Alors, je vais mettre aux voix, explications de vote. vote. La présidente, monsieur le Ministre, donc tout simplement pour vous dire, moi je m'étonne toujours de ce genre de, de, de, de propos parce que en fait il s'agit de quoi, de mettre en accusation de jeter la suspicion permanente quand on voit à certaines occasions, des groupes très organisés qui ne cesse de prôner la violence, de mettre en cause la police ou à l'autre niveau de demander des récépissés à tout va pour le contrôle, une cité alors qu'on sait ce que cela alourdirait les procédures et ça compliquerait la tâche je me, je m'étonne si vous voulez de de fait d'un autre côté, de dénoncer les violences policières sous toutes ses formes, avec le propos de sur le terme violences systémique et dans le même temps d'alimenter ce ce, ce sentiment de suspicion, donc là il y a là un comportement qui me semble complètement contradictoire et je crois qu'au contraire, alors quand même on peut le dire ici, calmement,

de ce qu'elle fait et elle a, elle, s'est à répondre quand il y a lieu, elle s'être sanctionné donc cette ce discours global, je veux dire, je ne le comprends pas et je trouve que tout ça finalement, finit par avoir l'effet inverse et après on a beau déplorer les effets de ses propres inconséquences au niveau des discours. Merci, cher collègue, alors je mets aux voix. Sauf s'il y a encore des demandes d'explications de vote non, je n'en vois plus donc je mets aux voix l'amendement 90 qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté, nous passons à l'amendement 137, il est présenté par Monsieur dessus. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, donc j'ai appris aujourd'hui qu'on avait le même âge et quelques semaines d'avance, on a vécu les mêmes évolutions technologiques, les mêmes progrès qu'elles ont apporté, mais aussi les mêmes, on a pu constater les mêmes dérives je pense et et ce rapport fait la part belle aux nouvelles technologies avec une fascination qui est presque naïve, avec toujours le même argument ces solutions permettront devant les policiers, plus efficace sur le terrain, mais dans ce domaine, beau comme dans beaucoup d'autres, c'est toujours la même logique, donc, le ministère qui a rédigé ce rapport appelle à plus de moyens plus investissements sans jamais questionner les finalités, les effets induits ou les limites de technologie on a on a j'ici dans un techno solutionner isme donc naïve, je l'ai dit, mais presque béat qui peut très rapidement dériver vers des réels dangers techno sécuritaire, voire à l'arbitraire, c'est donc notre rôle de législateur de borner cet enthousiasme qui peut se révéler dangereux, puisque dans ce rapport annexé, on parle beaucoup de principe et de grands objectifs, je propose d'en ajouter, hein, à savoir que l'usage du numérique doit se faire dans le respect absolu de la vie privée et des libertés individuelles, collectives et politiques tels que reconnus par la loi et la constitution et nous connaissons tous ici les dérives que l'usage de la technologie au service de leur peut amener fichages, surveillance généralisée reconnaissance faciale logiciels intrusifs, ce n'est pas de la science-fiction, la Chine nous offre en ce moment le parfaite exemple la parfaite démonstration d'une politique techno sécuritaire autour d'un État sans garde-fou et donc, au vu des enjeux au vu des dangers qui pèsent sur l'usage, c'est que notre technologie, nous estimons que ce rappel est loin d'être anecdotique et qui le fait qu'il est même fondamental. Si cher collègue, monsieur le rapporteur, avis de la commission.

les principales que les principales avancées qui ont été faites lors du de du dernier débat sur la sécurité globale sur le respect des libertés individuelles ont été à l'initiative du Sénat et avec l'accord du gouvernement, je, je, je vous ai dit si vous rectifiez votre amendement, on peut prendre la première phrase, vous avez décidé de ne pas le rectifier parce qu'on voit bien que l'intention va au-delà : avis défavorable. Même avis, merci monsieur le Ministre. Pas de demande d'explications de vote, je mets aux voix l'amendement 137 qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté à un moment 71 monsieur Bena Roche. Si madame la présidente, le rapport annexé prévoit la dématérialisation de la procuration de vote qui permettra à terme de, je cite : supprimer le nécessaire passage devant une autorité habilité officier de police judiciaire ou Adjoua de police judiciaire. Personnellement, je l'ai souvent dit, c'est souvent exprimé dans un certain nombre de de projet de loi autre proposition de loi très clairement la procuration et la modalité de vote la plus à ça sert qui est rouge, c'est pas là il il dirait la même chose que moi, c'est la seule été le Ventoux, on n'est pas sûr de l'effectivité ou de la véracité de ce vote là paix à personne, surtout sur les bancs de cette assemblée, les risques que fait courir l'absence de l'OPJ de cette procédure de procuration j'oserais ajouter que les procurations simplifié, entre guillemets, on en a vu pas mal chez moi quand je parle de chez moi, je parle des Bouches-du-Rhône et de Marseille, l'usager n'aura plus à se déplacer au commissariat de police en brigade de gendarmerie ou dans sa tiers-lieux autorisés par arrêté du préfet pour établir sa procuration, le gouvernement prévoit donc implicitement à la fermeture des guichets, tandis que, en dehors de cette insécurité ansi que 13 millions de personnes en France sont touchés par l'électronicien ou ne sont pas à l'aise pour mener des démarches dématérialisées, personnes âgées, fragiles, seront mis en mal par les envies de Take du gouvernement ou, pire, on pourrait abusé de leur confiance, avec ce système et les faire voter à leur insu. La fermeture des guichets dématérialisation d'une démarche administrative pour toujours à tête au principe d'égal accès au service public, les usagers doivent conserver le choix de leurs relations avec les forces de sécurité, les agents du service public afin de pas être enfermé dans une relation exclusivement numérique. Si cher collègue, monsieur le rapporteur, avis de la commission. Encore une fois, on part d'un postulat on aboutit à une mauvaise conclusion : on nous dit qu'on va les les guichets, mais le ministre, il vient de dire exactement le contraire dans sa réponse générale aux interventions générales et et pour la plainte en ligne, c'est une faculté ça permet justement d'éviter pour des personnes qui travaillent de devoir se déplacer d'attendre longtemps mais ça ça ça ne n'empêche en rien de pouvoir aller au commissariat et et les guichets vont rester ouverts votre amendement est satisfait, tels que le texte est écrit donc : avis défavorable. Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, d'abord, le monsieur le rapporteur a raison c'est une faculté, c'est pas 100 % donc bien évidemment, on pourra toujours continuer à aller passer en physique, si j'ose dire, si l'envie vous en prend, dans un site qui fera des procurations, deuxièmement la y'procuration en tout cas l'après-procuration a quand même démontré sa popularité, on a eu 170000 de mémoire mais je ne me rappelle plus exactement procurations en ligne qui ont permis, je crois à des. Citoyens d'exercer leur droit de vote alors après on peut être contre, on peut être contre la procuration mais là je pense qu'on dépasse le texte qu'on propose qu'on propose ici, troisièmement, il faut bien sûr pouvoir s'occuper de l'identité de la personne, à ce titre aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que l'OPJ. Mais ça prend aussi beaucoup de tâches indues des policiers, des gendarmes qui n'ont pas quand même pas que ça à faire, si j'ose dire que de passer un temps à vérifier l'identité de de la personne toilettes des moyens plus moderne aujourd'hui au moment où vous payez vos impôts sont passés devant un percepteur il y a peut-être moyen de vérifier, entité de quelqu'un sans passer devant un OPJ. Et c'est pour cela que la phrase du projet de loi dit à terme puisque nous allons travailler en peut-être qu'il y aura discussion sur ce sujet sur l'identité numérique aujourd'hui, mesdames et messieurs les les. Parlementaire, vous faites des virements bancaires, c'est quand même des choses importantes, sans passer par votre banque, parce qu'on est certain de votre. Identité numérique et donc identité numérique telle que l'imagine le gouvernement, et singulièrement l'intérieur en lien parfait évidemment avec la CNIL et le Conseil d'État permettra de vérifier d'identité de la personne, mais le contrôle de la procuration, il se fait également au moment du vote, il met au moment du vote voilà donc je pense que Monsieur le le le sénateur que sauf si vous êtes contre la procuration par principe et dans ces cas-là, évidemment, on ne peut pas faire grand chose dans ce texte, je crois qu'pouvait être à la fois rassurer et en même temps modernes ça me permet de dire ici Monsieur le sénateur, que ce n'est pas qu'un texte comme vous l'aurez constaté de police, il s'agit non de tous leurs que l'action du ministère de l'Intérieur a commencé par un grand service que le service des élections puisque nous modernisons aussi beaucoup les procédures de vote dans ce texte. Merci Monsieur Bénard Roche pour explication de vote.

on voit bien dans la réalité des faits, la difficulté, on voit bien qu'on aboutit finalement toujours à la faire à la disparition d'un certain nombre de personnels de guichet à la difficulté de plus en plus croissante pour des millions de personnes pas les personnes dont parle monsieur le ministre de l'Intérieur, bien entendu que pour ceux qui ont une maîtrise totale de tous les outils, ça ne pose aucun problème, voilà, mais par contre pour 13 millions de personnes, je suis désolé, c'est pas j'ai pas inventé le Siffre ça pose des problèmes, et comme on aboutit toujours avec ses procédures là à une disparition de l'humain et à une disparition de l'accueil public, je suis désolé de vous dire que la réalité prouve que j'ai raison et que mon raisonnement et bien et abouti bien à la conclusion à laquelle il doit aboutir, qui n'est pas une conclusion virtuel en l'occurrence mais conclusion de la réalité de la vie. Merci, je vais donc mettre aux voix l'amendement 71 qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté, nous avons trois amendements qui font l'objet d'une discussion commune, on commence par le 175 madame Assassi, vous avez la parole madame la présidente. Merci madame la présidente, nous considérons qu'il y a une contradiction un chatbot bottes et un un logiciel qui dialogue avec un un utilisateur n'a jamais été un outil franchement rassurant : il y a ici donc une des déshumanisation de l'interaction entre police et justice avec une mise à distance de de de la victime, c'est un fait, l'instauration d'un chapeau

par l'introduction d'un suivi de la plainte de Saint-par un agent de police judiciaire, le plaignant ne sera donc plus livré à lui-même, dans l'attente d'une réponse souvent tardives, voire inexistantes du ministère public, la plainte sera suivie et il sera avisée des suites qui lui sera donnée par lettre recommandée à l'issue d'un délai de 3 mois après son dépôt. Chers collègues, nous passons à la présentation de l'amendement 70 par Monsieur qui ne souhaitent pas effectué de démarches en ligne, vous allez me dire que peut-être c'est quelque chose qui est satisfait, en fait, les 15 dernières années montre que ce n'a les ça ne l'est pas, en fait, monsieur le rapporteur, et donc nous voulons poser les choses d'une manière claire puisque ce texte le permet, 22 pour 100 des personnes ne dispose pas leur domicile ni d'un ordinateur dis d'une tablette aujourd'hui 8 % 100 des Français n'ont pas d'adresse Mail ni personnel ni professionnel 15 pour 100 des Français n'ont pas de connexion internet à domicile avec les problèmes de pouvoir d'achat et les problèmes d'énergie aujourd'hui, je pense pas qu'on va résoudre ce problème très facilement et très rapidement ces chiffres, ils proviennent d'un rapport du 18 février 2022 du 16 février les ils sont parents s'a du défenseur des droits, la dématérialisation totale de la procuration de vote, j'en ai parlé et la généralisation de la plainte en ligne doivent nous alerter sur l'accès aux services publics des citoyens les plus fragiles, ce dont j'ai parlé, qui éprouve des difficultés avec les outils numériques, une politique d'inclusion numérique d'ampleur doit être menée, or elle n'est pas aujourd'hui à la hauteur des enjeux et des modifications des changements que vous voulez apportées par ce texte, il est donc nécessaire de bâtir pour chaque procédure dématérialisée guichets dans les commissariats et gendarmeries pour accueillir physiquement les personnes souhaitant effectuer de procuration de vote par exemple ce besoin de présence dans nos territoires est une demande répétée des acteurs locaux, qui voient les services publics déserter nos campagnes, mais aussi de nos hein désavantagé, à l'heure où nous faisons-nous Sénat des propositions pour permettre l'implantation de médecins dans les zones sous-denses il apparaît étrange de ne pas voir notre majorité sénatoriale aspirer aussi à un maillage territorial réel des services publics et donc il nous apparaît étrange de voir que cet amendement ne soit pas autre chose qu'un avis défavorable pour l'instant. Merci vous présenter, le 72 monsieur Ménard. Oui, madame la présidente, c'est pareil, c'est le recours croissant aux télé-procédures ne suppose pas la suppression des démarches en présentiel à aguicher. En supprimant ce qui est la politique du gouvernement et en renforçant la suppression des guichets de service public en général, comme c'est par exemple le cas dans les préfectures pour les prises de rendez-vous pour les titres de séjour sans tenir compte du handicap réel et d'éloignement de certaines personnes nous IT numérique, c'est la politique de ce gouvernement et le développement des points d'accueil France : dans les préfectures. Suffira-t-il à garantir à nos concitoyens un égal accès aux démarches administratives ces dernières offrent un accompagnement les maisons France service pour la réalisation des démarches en ligne mais non pas pour obliger d'effectuer à la place de l'usager, ces procédures, le défenseur des droits, toujours dans ce rapport de débat sur la dématérialisation dénonce l'usager devient coproducteur malgré lui, c'est à lui qu'il revient de s'équiper de s'informer, le cas échéant de se former et, partant, d'être en capacité d'effectuer ses démarches en ligne tout en répondant aux canons fixés par l'administration, comprendre les enjeux de la démarche, le langage administratif ne pas connaître d'erreurs au risque de se retrouver en situation de non-accès à ces droits et on voit le nombre de non-recours au droit qui qui qui augmente sur les épaules de l'usager ou de ces aidants repose désormais la charge et la responsabilité du bon fonctionnement de la procédure, face à ces dématérialisation demande en réalité aux usagers de faire plus pour que l'administration fasse moins et donc pour qu'on économise des ressources, là encore, je m'étonne que la majorité sénatoriale de soutiennent pas un amendement qui cherche à éviter, en plus de grever sur les finances locales, les dépenses de l'ambition gouvernementale, je rappelle donc que sur le plan budgétaire, les collectivités territoriales financent une grande partie des espaces froid service et perçoivent une aide de l'État qui n'est pas suffisante, détaillent les opérateurs partenaires contribue au coût de fonctionnement de plus de 1100 France : service à hauteur de 30000 euros par an, soit le coût d'un agent local de chacune d'entre elles, fait donc supporter le coût de la fermeture des guichets des services publics aux finances des collectivités territoriales, ce qui n'est pas souhaitable. Merci monsieur. Que le rapporteur, avis de la commission sur les trois amendements. Non, l'avis est défavorable sur les trois amendements pour des raisons différentes en ce qui concerne Madame Assassi Madame Assassi

j'ai lu comme c'est mon rôle dans le détail, le rapport d'orientation présenté par le ministre, il est écrit noir sur blanc d'améliorer l'accompagnement des usagers lors de leurs démarches en ligne et de réduire la fracture numérique chaque télé-procédures devraient être doté d'un moyen d'accompagnement effectif est adapté à tous les usagers : si on adopte l'amendement de Madame Assassi on supprime cette phrase qui justement garantie que, il y aura moyen adapté à tous les usagers et Monsieur Bénard je reprend ces procès d'intention des amendements précédents je lui pour la même chose, ces amendements sont satisfaits et cette phrase est claire et elle dit les choses avec clarté défavorable. Si Monsieur le Ministre.

prendre des rendez-vous pour que les gens puissent porter plainte dans certaines brigades de, de, de, de, de, de la campagne de la ruralité, parce que ça ne sert à rien, parfois d'avoir un gendarme qui fait le pied de grue comme ça à attendre le chaland ben non, on prend un rendez-vous et on a un service comme il faut plutôt que d'attendre et que les forces de sécurité soient vraiment sur le terrain, par exemple, autre exemple de la gendarmerie que j'aime beaucoup, c'est d'aller prendre des plaintes à domicile de manière électronique, ils ont à des ordinateurs portables, ils vont le faire aussi pour les gens qui n'ont pas cette faculté parfois, comme vous l'avez dit de l'électrolyse, on l'entend bien, et je ne suis pas pour le tout électronique, mais c'est un sujet supplémentaire, non, je crois que les forces de de l'ordre, le ministère de l'Intérieur, essaye de faire des efforts pour gagner du temps, homme de terrain et c'est de cela dont nos compatriotes ont besoin, et je trouve que c'est quand même plutôt bien de l'encadré par la loi, je voterai donc, comme l'a dit monsieur le rapporteur, contre ces amendements, merci monsieur, ma chère, je vais mettre aux voix l'amendement 175 qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour.

Le 139 présenté par Monsieur dessus. augmenter ça été rappelé par ma collègue assassiné, mais pour celles et ceux à qui cette partie au aurait échappé, je vous livre un un petit résumé dans la première partie du chapitre le ministre semble avoir pris conscience des limites de son enthousiasme un peu forcenés pour la nouvelle technologie, il dit à raison que que que l'ajout de plus en plus d'équipements dans la panoplie des agents multiplie le poids et les interactions homme-machine, ce qui n'est pas satisfaisant, ça j'ai cité le le le rapport et donc il faut y remédier mais alors la solution au problème est-ce que ça serait réduire les, les, les équipements ou questionner le le leur, leur légitimité mais bien sûr que non, puisque la solution c'est donc de déployer des exosquelettes pour pouvoir aider le policier à supporter le poids grandissant de ces équipements, donc on continue dans la dans dans la fuite en avant et donc dans le ridicule, cette logique s'ajoute le côté le plus, un peu plus qu'effrayant du résultat puisque le policier demain visiblement c'est Paul Verhoeven, qui l'avait imagine Robocop, il sera bardé de de de capteurs et d'Intelligence artificielle, voilà qui, à coup sûr. Permettra de rapprocher la police et la population comme cela et bien démontré dans le film, à noter également que dans le monde militaire qui a inspiré, c'est Didier cette cette idée d'augmentation des personnels, les projets d'exosquelette sont abandonnés, les uns après les autres, comme le projet à os américain en 2020 en raison d'une ergonomie incertaine d'un coût financier et énergétique important et d'une inadéquation entre les dispositifs et les objectifs tactiques du terrain, mais pour cela il faut fixer des objectifs, monsieur le Ministre afin que le ministère dont vous avez la charge se ridiculise pas avec des fantasmes coûteux, inefficace et dangereux, nous vous proposons de donc de supprimer ses alinéas. Madame la présidente, je crois que le le fantasme dans la tête de l'auteur des des rapporteurs, parce que je suis toujours sidéré de voir à quel point les membres de votre groupe Monsieur dessus, remettent en cause la possibilité pour la séance d'évoluer, on est dans une loi d'orientation et de programmation à 5 ans la réalité des exosquelettes et de la capacité. D'avoir pour notamment pour les pompiers, on a vu les grandes difficultés de la sécurité civile cet été et la nécessité de franchement de tout faire pour aider nos sapeurs-pompiers, il y a aujourd'hui techniquement toute une série de techniques qui pourrait évidemment avec des précautions avec de l'expérimentation avec de l'évaluation des expérimentations, nous nous permettre d'avoir une efficacité accrue tout en maintenant, évidemment, les forces en place et donc, vous êtes tout le temps dans le scepticisme du vieille de la séance en en nous faisant croire que c'est Orwell que c'est vers Owen ou que c'est Robocop non pas du tout, excusez-moi de vous dire, j'ai conduit avec mon collègue du hein et mon collègue de Belley, il y a pas si longtemps, une mission sur les questions d'Intelligence artificielle et d'utilisation des algorithmes sur les questions de reconnaissance faciale ou bien sûr, il faut mieux protéger les libertés, mais il y a toute une série de technologies et nous avons le privilège en France d'avoir les meilleures entreprises du monde, qui maîtrisent cette technologie qui nous permettrait d'avoir des résultats beaucoup plus efficient donc se priver de Maistre ce mot de réalité augmentée dans un un projet d'orientation à 5 ans c'est à mon avis une grosse erreur défavorable. Merci madame la présidente, il faut dire que le l'objet de votre amendement, enfin j'ai en tout cas son explication évoquait déjà le le ton de votre prise de parole puisque je cite la première phrase pour ceux qui ne l'auraient pas lu la présente partie du projet de loi des vols, le coeur de la pensée technos autoritaires de ses auteurs, bon alors vous complice étiez d'ailleurs pour ça, c'est encore une fois une attaques à nominem mais par des propositions extrêmement coûteuse parfaitement irréaliste et totalement déconnectée de vision apaisée, la sécurité,

justement pompiers comme a très bien dit monsieur le rapporteur, de pouvoir porter des charges lourdes, alors que même connaissent des difficultés, extrêmement fortes, éviter des maladies professionnelles extrêmement difficile, mais aussi permettre à des pompiers, notamment de pouvoir continuer à vivre du fruit de la passion et de nous aider en allégeant leur souffrance au travail, en fait, ce que vous aimez, c'est que les gens souffrent quoi c'est votre truc n'est pas possible autrement, c'est c'est pas possible indépendamment de la la détestation du progrès, et vous avez pas envie, par ailleurs, il faut vraiment que ce soit très difficile il faut vraiment subir le tripalium pour reprendre un mot sur le travail. Pour pouvoir arriver assez, assez, assez l'extrémité, je pense que votre intervention mérite et ce, sans cesse, sans doute, qu'on mette la caserne de sapeurs-pompiers au milieu du village.

pour cet amendement, je vais plutôt demander à un enrichissement de la technologie que vous proposez, puisque dans la veine des autres solutions présentées par le rapport pour améliorer l'efficacité des forces de l'ordre. Trouve donc les caméras piétons les caméras embarquées ces caméras installées sur les policiers en patrouille ou sur leurs véhicules, qui sont destinés à filmer les interventions sur le terrain. Et donc l'utilisation de ces dispositifs dans le cadre des relations police-population en France lorsque l'on regarde les discours du ministère de l'Intérieur semble suivre un objectif principal, rendent les citoyens plus Poli et respectueux, face aux forces de l'ordre puisqu'ils sauront qu'ils sont filmés, c'est effectivement une nécessité de se montrer respectueux envers nos forces de l'ordre, dont je salue le travail mais ce respect doit être et si réciproque et lorsqu'on regarde d'où viennent ces caméras piétons, à savoir les États-Unis et au Canada, ces dispositifs ont été installés sur les policiers dans une logique inverse à la nôtre puisque eux ne font pas l'autruche sur certains comportements déviant, c'est-à-dire rassurer la population, pour dissuader les voleurs, les violences éventuelles et les abus d'autorité, sachant que chaque intervention serait filmé comme ce ce rapport souhaite améliorer le lien entre vos services et la recherche académique, regardons les études puisque plusieurs ont été menées pour l'efficacité de ces caméras, donc les études canadiennes ne montre pas forcément une efficacité importante mais les études américaines entre montre que les caméras ont permis une nette amélioration de la relation police-population et aucune n'a eu des résultats négatifs, je prends une étude qui a eu lieu en 2013 à Rialto qui a déterminé que l'emploi de la force par les policiers étaient 2 fois moins fréquents et qu'il y avait eu une baisse de 87 % des plaintes contre la police pendant la période d'essai, mais il y a un point important dans tout Clusaz sont nord-américaine de ces caméras, il y a une condition centrale qu'on ne retrouve pas actuellement en France, les caméras doivent être allumé en permanence, pourquoi serions-nous le seul pays qui laisse le choix aux policiers d'allumer les caméras pour filmer le moment où ils sont à leur Avantage, occulter les autres pourquoi permettre à ces dispositifs, de devenir un autre vecteur de défiance avec la population, voilà pourquoi nous vous proposons dans un but de justice et d'apaisement que si les caméras piétons, il y a alors celles-ci doivent être allumé en permanence et l'agent qui étend sa caméra pour une raison ou pour une autre doit fournir un compte rendu,

monsieur le rapporteur. Comment peut-on défendre à quelques semaines d'intervalle, le tout et son contraire, nous avons fait la loi sécurité globale, on l'a examiné avec le ministre Darmanin dans cet hémicycle, il se trouve que vous aviez les deux même rapporteur mon collègue Loïc Hervé qui est membre par ailleurs de la CNIL a a pris un soin tout particulier à ce que l'on garantisse la protection des libertés publiques et à ce qu'on soit dans un usage proportionné des caméras dont je rappelle c'est l'ingénieur qui vous parle. Qu'elles ont une batterie et que vous pouvez pas non plus enregistré en permanence, faute de quoi, vous avez des gros problèmes techniques pour utiliser caméra ça c'est autre chose, mais tout ça pour vous dire que les caméras aujourd'hui ont un usage proportionné, qui a été défini réglementé, avec l'accord de la CNIL et et qui a été validé par le Conseil constitutionnel et à respecte les droits et les libertés, on doit rester dans le cadre de ce respect, on ne doit pas vouloir aller au-delà parce qu'on se trouverait confronté à un problème juridique cette fois-ci défavorable. Merci, monsieur le Ministre, même avis même avis. Et Monsieur Beuchere pour explication de vote. Juste pour dire, madame la présidente, que je suis un peu surpris que le de la part du groupe écologiste on demande toujours plus de caméras

Merci madame la présidente, cet amendement a pour objet aussi de définir l'utilité de la caméra piéton et de préciser son but. J'ai, j'ai entendu que certains alinéas particulièrement sur la captation en continu semblé vous convenir mais j'ai plus de difficultés à connaître vos réticences sur les autres points ce rapport n'est qu'une feuille de route à Khadr pour les futures prises de décisions budgétaires réglementaire, législative, il nous paraît important avec mon groupe du voir apparaître ses objectifs et ses limites dans le développement des caméras piétons, j'ai bien du mal à comprendre la réticence de notre assemblée à inscrire dans la ligne directrice du ministère de l'Intérieur, l'encadrement du développement des caméras piétons, c'est tout ce que nous demandons l'utilisation de ces caméras individuelles doit avoir pour objectif 1er, la diminution des cas de recours illégal à la force et la prévention des violences comme l'a expliqué mon camarade Thomas Dossus en ce sens leur utilité dans le contrôle, a posteriori de l'agent de l'action des agents notamment par la transmission des images captées aux autorités judiciaires, administratives ou disciplinaires dans le cas d'une mise en cause éventuelle d'un agent pour une infraction commise pendant l'exercice de ses fonctions dans le cas d'une procédure judiciaire à la Côte d'un agent ces images devraient être transmis sous scellés pour en assurer l'authenticité réaffirmé ce principe dans la loi, nous apparaît essentiel, il s'agit aussi d'exclure explicitement le traitement des images issues des caméras embarquées par des logiciels de reconnaissance faciale, ces derniers faisant craindre des risques de surveillance de masse de la population, les débats suscités par cette technologie ne font que grandir en janvier 2020 la pré-publication du Livre blanc sur la tige os artificiel de la Commission européenne, envisager la mise en place d'une interdiction temporaire des technologies de reconnaissance faciale dans divers secteurs, la reconnaissance faciale ne doit pas être considéré comme une technologie d'identification biométriques comme les autres, le RGPD garantit aux citoyens le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage selon la définition du profilage inscrit dans l'article IV l'usage de la reconnaissance faciale notamment de façon automatisée autre contradiction avec l'article 5 du RGPD enfin parce que la reconnaissance faciale à part. C'est la catégorie plus large et biométriques à l'autre, également en contradiction avec l'article, j'ai terminé interdissent le traitement des données biométriques. Là vous pouvez pas Monsieur Bénard chaque argumentaire dépasser le temps de parole, sinon on va pas en sortir Le respecter, à chaque fois une fois oui 2 fois oui mais c'est, sinon on va vraiment déraper dans le temps sur l'examen du texte, merci monsieur le rapport. Sur les 2 premières parties de ce que demande Monsieur Bénard je le renvoie au rapport il y a une phrase que j'ai mis que je lui ai cité ce matin et qui répond parfaitement ce ces 2 premières parties sont satisfaites sur la reconnaissance faciale nous avions interpellé le ministre là-dessus, il s'est exprimé, il nous a dit qu'il faudrait une loi spécifique jeux olympiques entre guillemets ou une PPL venant de l'Assemblée ou du Sénat, et nous avons à l'initiative du président buffet fait une mission sur la reconnaissance faciale qui prend en compte tout ce qui vient de dire sur le RGPD, etc, avec mes collègues du de Belenet et qui fait des préconisations je le renvoie, ce rapport qui a été votée par la commission : avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Je ne reviendrai pas sur les caméras individuelles, la président parce que je crois que le rapporteur a évoqué, puis on a eu des longues discussions pendant le la loi sécurité globale sur la question des nouvelles technologies appliquées aux images qui est finalement votre intervention, monsieur le sénateur, je voudrais vous dire que d'abord le choix qui a été fait par le gouvernement et voilà une différence parce ce secteur heures durant avec le 1er texte déposé, c'est d'avoir retiré les dispositions qui pourraient des ordonnances pour régler le problème du statut unique des images peu conseiller d'État nous avait dit mais la CNIL avec le Conseil d'État votre multiplication des vecteurs technologique, la caméra piéton la caméra tout court, le drone le le la caméra héliporté c'est une multiplicité de statut alors qu'il faut le font dans un statut, un seul et unique statut et il nous inviter à faire ce statut unique de l'image très important mais très complexe également et par ailleurs, on doit mettre notre législation à l'aune du RGPD nouvelle formule, je parle des caméras de vidéoprotection classique. Donc on a des partis sur une ordonnance, est nous écoutons le Parlement et ministre des Relations avec le Parlement, premier qui dit non malheureux, pas d'ordonnance, même s'il était prévu par le général, il faut quand même considérer que c'est pas respectueux du Parlement, et donc nous avons dit aux sénateurs Hervé sénateur de Bresse retire les dispositions et coordonnant c'est est pas une ordonnance dans ce texte, puisque la seule ordonnance de transformant en dur dans quelques instants,

et j'ai dit au rapporteur, que si elle venait du Sénat, nous serions très heureux sur le statut des images soit elle viendra d'une loi spécifique Jeux olympiques mais je pense que c'est encore mieux, c'est une proposition de loi pour que nous réglions le sujet, je me suis déjà exprimé pour dire que j'étais opposé à la reconnaissance faciale,

dans les dispositifs de d'images, c'est autre chose que de la reconnaissance faciale voilà mais je sais bien que vous économique je je parle pour lui, donc je suis pas favorable à la reconnaissance faciale dans les images, quels que soient ses supports et le Sénat dans son a fini sagesse et monté sans doute proposera un texte sinon le gouvernement prendra si. Merci, Monsieur le Ministre Monsieur Bénard Roche : demande d'explications de vote. pourquoi ne pas inscrire dans la feuille de route de votre ministère, c'est une feuille de route pour 5 ans, ce que vous venez de vous dire monsieur le midi, c'est tout ce que c'est tout ce que je dis, j'ai bien compris, il y aura une loi mais pour des tas de sujets qui sort dans cette feuille de route, il y aura des il y aura aussi des décisions qu'elle soit réglementaire ou législative, pourquoi celle-ci il a pas droit. Alors je je vais mettre aux voix l'amendement 103 qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté le 116 Madame de Marco. Merci mais ne le présidente, monsieur le Ministre, les terribles incendies qui ont connu la Gironde et les Landes cette année et le développement d'incendies en Bretagne ont témoigné d'une force nouvelle de la nécessité de déployer une seconde base de sécurité civile, dans l'ouest de la France, c'est une demande de plus en plus forte des élus locaux, elle a été formalisée dernièrement par une demande conjointe des présidents des départements des Landes et de la Gironde, tous les acteurs sont unanimes : plus le feu repérer traiter rapidement, plus les chances de l'État ne se renforcer au regard de l'Exposition colossal des forêts de l'ouest de la France et notamment des forêts de pins au risque incendie, il est indispensable de rapprocher les moyens de la sécurité civile des foyers à risque une création d'une telle base est en outre parfaitement compatible avec les promesses présidentielles d'étoffer la flotte de Canadair via un effort européen, il serait alors possible d'équiper, c'est une nouvelle base Sasa moins dire les capacités de la baisse de Nîmes, j'attire malheureusement attention car nos Canadairs sont vieillissants sur 12 avions Canadair seuls huit serait opérationnel en même temps qu'en est-il du renouvellement de la flotte, la France va-t-elle se contenter des 2 Canadair bombardiers d'eau, commandé par l'Europe est-ce que les comptes Bombardier promis son type commandés, je vous remercie. nous ne pouvons pas prendre cet amendement ça s'il sera à faire une injonction au gouvernement et ce serait pas constitutionnelle, pour autant, le ministre, il a un choix compliqué au soit on décentralise dans les régions, avec évidemment une dispersion, soit on centralise avec une économie de moyens sur maintenant c'est entretien, c'est à lui qu'il appartient de prendre cette décision, donc il va vous répondre, mais nous, nous ne pouvons pas prendre ce cet amendement telle qu'il est écrit : ce serait une injonction, donc je suis défavorable. Merci monsieur le ministre. Alors, Madame la sénatrice, je vous propose, si madame la présidente, on est d'accord peut être de sous-amender votre amendement pour qu'il ne soit pas impératif, mais qui permettent la conditionnalité puisqu'il s'agit de la tentation de d'étudier. Je voudrais répondre en même temps, ah Monsieur le le sénateur du Gard. Quelle est notre difficulté. Si vous créez plusieurs bases qui peut apparaître intelligent a priori vous allez diluer les moyens, et quand bien même nous rachète aurions le même nombre d'avions et pour des raisons que je pourrais vous expliciter ce n'est pas possible non pas budgétairement mais matériellement les fameux Canadair ne sont plus produits, donc il faut d'abord produire l'usine qui produit des canadairs, c'est un de nos problèmes, bien évidemment, indépendamment du fait que nous ne pouvons pas acheter ce matériel parce qu'il manque, et il manque au niveau européen et c'est pas une question budgétaire si nous dispersent on les lieux, nous allons rendre difficile par la spécificité des mécaniciens qui réparent la nuit quand les avions volent le jour parce que les Canadair par exemple ne volent que le jour ce matériel qui permet à flux tendu dans l'intervention des avions. Et ce mécanicien et ses pilotes extrêmement spécialisés que nous avons du mal d'ailleurs à payer vis à vis de la concurrence du privé, nous en avons peu les chérissons, si j'ose dire et la base de Nîmes-permet de réparer la nuit, les avions qui volent le jour. Si on a de base dans 2 territoires différents, nous ne serions pas capables aujourd'hui de maintenir en fait le même niveau d'intervention aérien pour les feux de forêt, et vous l'avez très bien dit Madame la sénatrice, ça aurait pour en en repérant tous des feux qu'on arrive à les éteindre dès qu'il dépasse 5 10 hectares, si j'ose dire c'est déjà perdu et c'est pour ça que les avions partent dans feu pour aller vers un autre, non pas pour abandonner un territoire qui est en feu, mais pour aller éteindre les autres feux qui laisse et c'est pour ça qu'ils reviennent, je voudrais aussi vous dire que l'aérien n'est pas la façon la plus certaine d'éteindre un feu, on sait tout ce que c'est l'entretien des forêts et que c'est par ailleurs le travail des soldats au feu au sol aériens fait permet de, de, de tenir mais ne permet pas d'état mais je reviendrai si vous souhaitez donc moi je n'ai rien contre l'idée de créer une 2ème, base des faudrait savoir où on le long là mais ce que vous évoquez la Gironde mais si je vous dis que la moitié des feux, c'est dans le nord de la Loire, l'autre moitié au sud de la Loire, c'est une 2ème, base, elle sera peut-être plutôt au nord de la Loire qu'au sud de la Loire,

D'abord parce qu'on y réfléchit, madame sénatrice ça peut me dire au sénateur du Gard, qu'il a parfaitement raison et nous nous battons pour que la base de Nîmes-soit non seulement la la base de l'excellence française ce qu'elle est, mais la base européenne et si nous sommes très ambitieux, la base Europe méditerranéenne, puisqu'elle est idéalement placé. Avec des gens de pointe, un département qui accueille depuis très longtemps, la sécurité civile, avec des moyens technologiques très important et que nous devons renforcer, vous le savez bien, monsieur, donc le commissaire européen les les laïcs viendra très certainement et très bientôt, conformément à ce qu'on a fait pour la présidence française de l'Union européenne Nîmes je me rendrai avec lui sur la base aérienne de Nîmes pour consacrer, je l'espère le statut européen de la base de la base de Nîmes je pense que votre travail depuis très longtemps, sera ainsi récompensé. Alors ce que je vous propose parce qu'il y a 3 demandes de parole, donc moi je vous propose d'abord on va écouter les trois demandes de pas de d'explication de vote et après, si vous le voulez bien mais on en reparlera ensuite est-ce qu'on fait pas un amendement rectifié, c'est comme vous le souhaitez, un amendement rectifier c'est plus rapide, un sous-amendement faut l'écrire hein rectifier si l'auteur de l'amendement, on est d'accord, ça peut aller plus vite, si on est d'accord sur la rédaction Monsieur le ministre, on en reparle après on les écoute On écoute, et après, si vous le voulez bien, on se met d'accord sur la rédaction on le rectifie. Allez madame Ribet. Oui, j'ai, j'aimerais rappeler dans le sens que de de ce qu'a dit le rapporteur, Monsieur le Ministre, je, je, vous avez posé la question en tant que sénatrice de la Gironde habitant sur le secteur de Landiras, je vous avez posé cette question lors de votre audition, moi j'ai bien compris et je suis soucieuse de l'équité territoriale de tous les territoires parce que c'est vrai qu'on peut avoir des incendies partout et nous, nous avons proposé un amendement en commission, qui a été intégrée au texte où nous parlons de maillage territorial nécessaire, alors on peut, on peut éventuellement ajouter plusieurs qui mais nous, on l'avait fait exprès dans cette intention, c'est-à-dire de ne pas jouer la concurrence des territoires, mais de mettre en avant parce que c'est ça qui est important, le maillage territorial et pas une région plutôt que plutôt qu'une autre, donc dans ce sens-là, je pense que la l'amendement le sous-amendement serait satisfait dans la mesure où on parle de maillage territorial dans la version de la commission, mais on peut éventuellement ajouter plusieurs bases plusieurs bases territoriales. Merci, cher collègue Monsieur Grenier. Oui merci madame la présidente, monsieur ministre monsieur le rapporteur, je rejoins le propos de notre rapporteur. Et je suis heureux de la réponse de notre ministre. Le sujet, et il est quand même réelle. Je suis de l'Est de la France qui aurait imaginé que massif vosgien et autant de départs de feu. Comme le massif jurassien, donc il y a un vrai sujet aujourd'hui par rapport à l'Exposition des massifs forestiers, la richesse forestière de notre pays, qu'existe et aujourd'hui effectivement dont j'entends le débat, il faut l'élargir et effectivement il y a une notion de de de territoire et d'Exposition de ces territoires, à ses risques d'incendie qui, pour certaines, certains de ses massifs forestiers, c'est pas de connaissent qu'une connotation négative, c'est pas des broussailles, c'est souvent une forêt qui a un siècle, voire 2 siècles, c'est un Patrimoine économique terrible, et en plus, souvent avec une présence humaine très habitée massifs forestiers des Vosges et un des massifs les plus habitées des massifs forestiers de France, donc il y a un vrai sujet mais je j'irais plus loin Monsieur Luigi monsieur ce Ministre, monsieur le rapporteur. J'ai cru lire qu'effectivement au niveau communautaire à Monsieur le Ministre, vous n'faire allusion qui avait effectivement une situation identique d'Exposition dans d'autres États membres et je pense qu'effectivement par rapport à l'Est de la France, proximité des massifs allemand on on a peut être une opportunité d'avoir une dimension européenne sur ces sujets, mais c'est un sujet vraiment important et il y a urgence de se positionner sur cette notion territoriale de protection de notre richesse forestière. Merci monsieur Grenier et il nous reste la demande d'explication de vote de madame De Lattre. Oui merci madame la présidente, comme mes collègues en Gironde et et et plus particulièrement avec Laurence est arrivée, nous avons été touchés puisque évacué toutes les deux dans nos zones respectives, c'est une question qui s'est posée : qui se pose je salue votre sagesse, monsieur le Ministre, de proposer un un sous-amendement, alors c'est vrai que dans cet amendement et noté la création qui pourrait coûter de 7 secondes base entre 16 8 et 18 millions mais ça c'est l'investissement, après il y a le fonctionnement, donc je pense qu'il faut effectivement avoir une réflexion très large, je vous remercie, monsieur le le ministre-d'associer le Sénat dans toute sa composante parce que comme nous représentons les territoires, je pense que, de notre réflexion peut venir aussi une aide pour le positionnement de de cette base, il n'en reste pas moins que tout le monde ne pourra pas avoir une seconde base je pense que en alerte canicule, il serait intéressant de pouvoir prépositionner c'est-à-dire que Bordeaux, Nîmes, Bordeaux c'est 45 minutes d'avion quand ils sont pleins, peut être un peu plus mais cela permettrait déjà d'être rassuré, c'est vrai que dans ces périodes d'alerte, de savoir que nous pouvons compter sur la rapidité d'envoi de de ces avions que nous pouvons abriter sur les bases soit militaire puisque nous en comptons quelques-unes notamment Cazaux et et Mérignac, soit sur des bases civiles qui permettent de, de, de, les, de type d'avion, en tout cas merci monsieur le Ministre de de votre écoute en Gironde, nous saluons votre proposition. Merci, cher collègue, peut-être, si vous le voulez bien comme monsieur le rapporteur demande à parler avec Monsieur le Ministre, veut s'exprimer suite aux propos de nos intervenants, monsieur Dobres commencer Monsieur le Ministre va nous. Faire un résumé et une proposition finale. Compte tenu, compte tenu de, de l'ouverture qu'a fait le ministre moi ce que je propose, ce qui serait le plus simple pour le pour la séance et qu'on fasse un amant de Marco face un amendement rectifié qui dirait le gouvernement étudie l'opportunité de la création d'une seconde base pour les canadairs et autres aéronefs de la sécurité civile, afin de pouvoir intervenir au plus vite lors des départs de feu et ensuite il y a une méthodologie qui sera employé mais je pense que si on veut répondre à la préoccupation des uns et des autres, c'est mieux de l'écrire comme ça et et ça nous permettrait de pouvoir le voter avec un il, la commission n'a pas étudié a-t-il personnel, j'y serais favorable. Madame de Marco, on est d'accord pour que Monsieur le Ministre, dise, hein. Oui. écoutez bien évidemment en espérant que le gouvernement va l'étudier très prochainement cette opportunité n'est-ce pas Monsieur le ministre. Merci madame de co-donc monsieur le ministre, je vous donne la parole. non mais oh, de plus, une si je peux me permettre, puisque c'est votre amendement que je suis amende sur le maillage territorial, j'ai peur que ça ne satisfasse pas tout à fait la demande même la sénatrice puisque il s'agit pas simplement du maillage, il s'agit d'une base vous avez déjà achète rien parce que vous avez des pélicans Drôme dans votre département, donc je pourrais jouer aux naïf et ainsi répondre assez facilement que vous, mais je vous mentirais en me disant que ça suffirait dans la réflexion de la sécurité civile pour une 2ème base j'ai bien compris votre demande, un peu comme le Gard voilà, bon c'est c'est c'est un peu la la demande. Deuxièmement, il y a déjà du prépositionnement d'avion, on le fait, notamment en Corse, on le fait parfois dans notre territoire, moi je voudrais quand même attirer votre attention sur la stratégie de la sécurité civile. Ces concentré. De façon extrêmement forte, l'intégralité de la flotte aérienne pour pouvoir éteindre le feu, ce qui n'est pas la même chose que de repérer le feu s'il s'agit de repérer le feu, les pays qui ont Drôme des hélicoptères on on renouvelle dans la que je vous propose les drônes permettent de repérer le feu, mais une fois que vous repérez le feu, il faut l'éteindre et ça ne marche que lorsque vous avez toute la flotte ou quasiment toute la flotte, qui intervient sur le feu, donc si vous divisez. Sur le territoire national le la flotte aérienne vous repérer les feux mais la belle affaire, on paiera plus vite les feux ben très bien et en même temps on les verra tous plus voilà donc la deuxième base ne va que si on résolve de problèmes et quelque part, les 18 millions sur les 15 milliards ne sont pas le problème, c'est un est ce qu'on est capable d'avoir une autre flotte aérienne à peu près équivalente à celle du Gard ailleurs

même si on avait l'argent, on ne peut pas les acheter aujourd'hui et tous les pays sont dans la même difficulté que nous et la 2ème des choses c'est qu'il faut trouver les spécialistes de la spécialité, comme dirait Godard pour pouvoir les conduire parce que c'est très spécifique comme métier et pour voir les réparer, donc ensuite il y a l'implantation et je pense que cette heure que on discute ensemble de cette implantation, donc vraiment je vous dire que c'est pas parce que vous, des avions partout, sinon on l'aurait déjà fait qu'on qu'on arrive à être plus efficace : voilà, il faut vraiment bien comprendre ça, c'est sûr que pour nos concitoyens, c'est pas toujours facile à comprendre, mais c'est le gage de notre efficacité. Merci, monsieur le Ministre, alors si vous le voulez bien je vais vous proposer qu'on relise le la proposition d'amendement rectifié pour être bien d'accord sur l'amendement que nous allons voter, l'heure, Alina 60 compléter cette Linea à par une phrase hein. Rédigé le gouvernement étudie l'opportunité de la création d'une seconde base pour les canadairs et autres arrêts aéronefs de la sécurité civile en Nouvelle Aquitaine. C'est pas ça.

que je viens de vous faire parce que, oui, mais après, moi c'est moi, je, je, j'interviens comme rapporteur et compte tenu du débat, telle que nous l'avons instauré et pour essayer de répondre à la question, il me semble, et j'ai écouté ce que dit monsieur grenier, on entend ce que dit le ministre, on entend ce que disent nos, nos collègues du du moi je pense que il faut que cette étude se fasse, qu'elle prenne en compte tous les paramètres et ils sont nombreux, et le ministre, il en d'indiquer plein de paramètres techniques le mieux, si on veut trouver un consensus et de rectifier l'amendement en disant le gouvernement étudie l'opportunité de là. Création d'une nouvelle base

le gouvernement étudie l'opportunité de la création d'une seconde baisse pour les canadairs et autres aéronefs de la sécurité civile, point terminé on va voter donc sur cet amendement rectifier là, si tout le monde en est d'accord.

ça va de soi, ça va sans dire. ça va de soi Madame Goulet, vous avez la parole. Oui, madame la présidente, monsieur le Ministre, je note avec avec intérêt cette rédaction et je me demande si dans le PLF qui arrive, nous venons d'instaurer une nouvelle jurisprudence pour éviter d'avoir des rapports rejeté si on pourra, dans le cas du PLF qui arrive à voir un certain nombre d'amendements, sur lequel le gouvernement réfléchit à telle et telle chose pour pour pouvoir avoir des dispositifs qui finalement me semble une rédaction bien astucieuse et que je voterai tout à fait, je vous remercie, Monsieur le Ministre. On est d'accord, on s'arrête à sécurité civile je mets aux voix l'amendement 116 rectifier ainsi rédigé : qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il. Bien. Monsieur Richard s'abstient, il est adopté. Amendement 176 présenté par Madame Cuq Hermann Maier, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous me permettrez, même s'ils ne sont pas en discussion commune de fait de de présenter les 2 amendements puisque ils ont, en tout cas la la même philosophie, loin de nous, mais la présidente ça si le rappelait dans son intervention générale de remettre en cause tout recours bien évidemment aux possibilités offertes par le numérique reste j'oserais dire des hiérarchies est-ce que c'est demain le numérique placé en priorité stratégique définira la politique de sécurité intérieure ou est-ce que c'est la politique de sécurité intérieure qui, une fois définis et développés s'appuiera sur la capacité du numérique il nous semble donc l'année Linia 70 et 73 pour l'amendement 176 à La Linea 74 et 78 pour l'amendement 177 la volonté d'ériger le numérique en fonction stratégique pour nous, en tout cas, interpelle-t-elle et le sens de ces deux amendements. Merci. Collègue monsieur le rapporteur, avis sur le 176. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment, et ce sera le même avis pour le suivant. Bien, Monsieur le Ministre. Oui, très rapidement, madame la sénatrice, je comprends votre votre la rédaction faisait penser que c'était le numérique et la priorité du ministère de l'Intérieur comme objet d'intervention de c'est un service public, je serai prêt même à voter votre moment si j'étais sénateur mais c'est pas l'objet de la la situation, c'est une loi aussi de moyens, et vous savez qu'on vous êtes dans un service de police et que vous êtes obligé de faire des photocopies et d'imprimer sans cesse des exemplaires alors que vous pourrez très bien le faire de manière numérique et les les policiers le demande d'ailleurs pour une très grande partie à condition du numérique soit simple, efficace et qui fonctionne vous gagner énormément de temps et c'est une facilité. Le numérique, il vous êtes dans votre travail de sénateurs le le le fait d'avoir mis des ordinateurs et d'avoir émis des tablettes permet d'améliorer votre travail et de vous concentrer sur la choses. Une importante donc, faut bien que vous compreniez ça changera sans doute pas votre opinion sur la maman sur le sur le texte, mais qu'il s'agit pas d'utiliser le numérique comme finalité mais comme moyen voilà et que nous avons mis à intérieur une dette numérique comme on dit très joliment aujourd'hui extrêmement importante et que c'est ça contribue aussi à la souffrance au travail, aux difficultés que connaissent les agents de police que vous connaissez aussi.

Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 177 qui a reçu le même avis même vote il n'est pas adopté le 141 monsieur dessus. Merci madame la présidente, donc on l'a bien compris la technologie va être amené à prendre de plus en plus de place dans le quotidien des forces de l'ordre et pour que cet objectif soit mené à terme, il faut naturellement des marchés publics d'équipement, il convient de donc de lui adjoindre d'agents à la technologie, un certain nombre de garde-fous et aux marchés publics aussi indispensable compte tenu d'un certain nombre de dérives qu'on a pu connaître récemment dans les technologies de surveillance concernant les marchés publics du ministère de l'Intérieur, l'éthique des marchés publics nous semble primordial, nous souhaitons poser un principe clair : pas de marcher avec des entreprises qui ne respectent respectent pas les droits de l'homme, cette inquiétude est légitimée car nous avons appris par la presse que l'État envisageait un à un moment de signer un contrat avec l'entreprise israélienne NSO Group, connu pour son logiciel espion Pegasus, qui je le rappelle, fait l'objet d'une commission d'enquête européenne et qui a été utilisé par de nombreuses dictatures à travers le monde pour ficher et contrôlé, alors à la fois l'opposition et la population, la signature a été évité de justesse par ordre du gouvernement mais il n'est pas normal que ce soit le fait du prince, qui a empêché ce contrat scandaleux, nous souhaitons donc ici que le ministère de l'Intérieur mette en place une politique proactive d'enquête envers ses contractants, particulièrement dans le domaine sensible des nouvelles technologies. Si mais. Le rapporteur. Le le problème s'amendement j'ai dit en commission, c'est qui qui n'est pas opérationnel, comment le ministère peut s'assurer de l'ensemble de l'activité des entreprises et des co-contractants des entreprises donc telle qu'il est rédigé, on est obligé d'être défavorable. Merci, monsieur le Ministre, même avis. Et ce qu'il a, c'est une question un peu naïve, mais ce que vous connaissez un Label qui nous permettrait peut-être parce que, effectivement, je crois que ce sera monsieur le rapporteur a raison de dire que vous voyez c'est c'est complexe quand même de faire de démarche éthique moi j'entends ce que vous dites est-ce qu'un Label, comme sur d'autres sujets, notamment environnementaux on ne demande pas à chaque entreprise de vérifier qu'ils sont en effet conforme à nos émissions carbone mais ils ont des labels est ce qu'un Label qui permet de le faire. écoutez monsieur Villet, je vous invite à vous retourner vers 2 à ce nombre d'ONG par exemple Amnesty International qui fréquemment liste un peu les entreprises qui qui se compromettent avec un temps de dictature et puis qui font aussi quelques rapport sur l'état de la police en France et les techniques matière Lord par exemple récemment, donc vous pouvez peut-être vous aurez vous tournez vers cette organisation. donc. Je mise aux voix, l'amendement 141 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté le 140 monsieur dessus. Merci madame la présidente, donc dans la rédaction initiale de la partie relative aux aux relations entre le ministère de l'Intérieur et le monde universitaire se trouvait une injonction assez étonnante envers les universitaires, il était ainsi écrit que le monde académique devra nouer des partenariats privilégiés avec le ministère de l'Intérieur et donc je remercie les collègues du groupe socialiste qui en commission sont venus rectifier cette injonction en inversant la logique et en affirmant qu'au contraire c'est au ministère de nouer des partenariats privilégiés avec le monde académique dans la logique de cette correction, je vous propose d'aller un peu plus loin en rappelant tout d'abord l'existence des libertés académiques dans notre pays qui sont, je le rappelle, érigé au rang de principe des principes fondamentaux des lois de la République, à ce titre, nous voulons rappeler que le déroulé des travaux universitaires ne saurait tolérer la moindre ingérence ou tentative d'influence sur les résultats de la part du ministère, nous voulons également précisé que le ministère devra soutenir avant tout les recherches ayant lieu dans le Champ des sciences sociales, particulièrement celles relatives au renforcement du lien entre police et population, nous estimons que la véritable priorité se trouve ici plutôt que dans les domaines des nouvelles technologies de sécurité c'est ce Champ-là qui, qui doit être investi de toute urgence pour apaiser nos politiques de sécurité à ce titre, les universitaires peut-être. Peuvent être d'une grande aide si on les laisse travailler correctement et c'est précisément le but de cet amendement. Merci messieurs de ce monsieur le rapporteur. J'ai accepté en commission l'amendement du groupe socialiste qui était fondée, qui disait, il appartient au ministère de d'essayer d'avoir des relations avec le monde universitaire, mais là on est à nouveau dans un procès d'intention sur ce que pourraient être des moyens de pression, je ne sais quoi franchement avis défavorable. Monsieur le Ministre. Même avis je mets aux voix cent quarante avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté, nous avons cet amendement qui font l'objet d'une discussion commune dont 2 identique, le dix-huit pour commencer, c'est monsieur Sueur qui le présente. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, vous le savez, cet amendement porte sur un sujet très sensible, puisqu'il s'agit de la police judiciaire et de la réforme du projet de réforme visant à unifier l'ensemble de l'organisation de la police, d'abord au niveau départemental, ce qui est contesté et sous l'égide d'un directeur départemental qui aurait autorité sur l'ensemble des services de police, y compris la police judiciaire, beaucoup de représentants de la police judiciaire, on dit que le risque existait de déconnecter la compétence territoriale de la police du Champ d'activité du haut du spectre de la délinquance, notamment la délinquance organisée, le grand banditisme, la délinquance financière, qui intéresse aujourd'hui les directions régionales et inter-régionale de la police judiciaire et ne se limite pas au périmètre départemental, vous avez entendu Monsieur le Ministre, les propos de monsieur le procureur général près la Cour de cassation et aussi ce qui est dit par de nombreux professionnels aussi par les magistrats, par les avocats d'ailleurs, je me permets, madame la présidente, une petite suggestion amicale, je pense qu'il serait utile que monsieur le garde des Sceaux, fut au banc sur un tel sujet et je pense qu'il ne manquerait pas d'éclairer le débat. Mais il n'est pas venu nous avons vu, Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, il est reparti mais je lui envoie le message que ce serait bien qu'il demande à ce que sur ce sujet, le garde des Sceaux, soient également présent, c'est normal que vous soyez présent Monsieur le Ministre, mais votre collègue, pourrait l'être aussi, donc, vous remarquerez qu'il s'agit d'un sujet qui est tout sauf anodin, mes chers collègues, et c'est pourquoi nous demanderons un scrutin public sur cet amendement, ainsi que sur le suivant.

Madame la présidente, dans la mesure Monsieur le Ministre, où vous avez pu déclarer que sur ce sujet qui est très sensible qui suscite beaucoup d'émoi des motions de protestation par rapport auquel vous avez expliqué tout à l'heure votre philosophie, vous avez annoncé que la mise en oeuvre éventuelle de ce dispositif n'aurait pas lieu avant le second semestre de l'année 2023, dans ces conditions, mes chers collègues, et je me permets d'attirer votre ration votre attention là-dessus, est-il opportun pour calmer les esprits, de proclamer des aujourd'hui dans un rapport annexé que cette réforme est nécessaire, inéluctable et ce sera fait, moi je pense qu'en déposant ces deux amendements et notamment celui-ci : Monsieur le Ministre, et si vous vouliez bien donné un avis favorable, ce qui n'enlève rien ce que vous avez dit il n'est absolument pas nécessaire que ce sujet soit abordé dans le rapport annexe puisque d'ailleurs. Aucun des articles de loi de la loi du poids du projet de loi, aucun des alinéas aucun mot ne traite de ce sujet donc en bonne logique, législatives, pourquoi vous savez on nous parle tout le temps de l'article 45 n'est-ce pas, mais alors pourquoi introduire cela. Alors qu'il n'en est pas question dans ce cas des articles du texte, c'est une question donc Monsieur le Ministre, vous voyez bien que si vous souteniez cet amendement remarqué, vous pouvez aussi mieux soutenir le dix-neuf que le 18 mai dans les 2 cas, le message serait le même d'une certaine façon, vous accepteriez de retirer quelque chose si aujourd'hui crée une très grande de très grande préoccupation et je pense que ça irait dans le bon sens pour le dialogue que nous souhaitons qu'il nous paraît nécessaire sur ce sujet. Monsieur le questeur alors Monsieur Bénard je vous avez la parole pour le 75. Quoi. Oui, madame la présidente, l'autre amendement va exactement dans le même sens que les 2 amendements présentés par monsieur sueur en fait rarement, un projet de réforme, a reçu en plus une opposition aussi unanime par une si grande variété d'acteurs, associations, syndicats de magistrats, syndicat d'agents de police judiciaire, enfin, de nombreuses interrogations et inquiétudes et, la dernière étant en fait le limogeage du directeur de la PJ, Éric Arella, à Marseille, qui fait un peu les frais de de cette opposition générale d'ailleurs laissé ses ont manifesté d'une manière très calme d'ailleurs leur opposition justifiée, comme toujours, cette réforme est présentée comme émanant du bon sens, du pragmatisme, la commission des lois, s'en est inquiété d'ailleurs au point de créer une mission sur le sujet et quand, dans le groupe quoi mais. Le groupe socialiste d'ailleurs propose de supprimer toute mention de cette réforme dans le texte qui nous est présentée, je suis surpris que la commission des lois ne soient pas d'accord en fait avec nos propositions, cette réforme fait l'objet de critiques, toutes circonstanciée comme la crête de traitement dégradé de la délinquance, la DDPS, attachée à la culture du chiffre et du résultat risque, on le sait, de renforcer le traitement des dossiers des petits litiges et contentieux de masse ou des traitements du trait au détriment, il est à craindre aussi une disparition progressive de spécialisation de la PJ par rapport aux missions de la police au quotidien en plus les les membres de la PJ pourrait être placé en priorité sur des missions de sécurité au quotidien surchargés de dossiers leurs compétences. Pourrait se diluer et se renforcée par les résultats des départements ayant déjà expérimenté la réforme ou dans lesquelles elle s'appliquent déjà cette réforme au nom de la. Politique du chiffre et du tout sécuritaire entraînera de façon insidieuse en plus une confusion entre les pouvoirs judiciaires et administratifs en établissement Délia fort entre les services de police judiciaire et les préfets conduisant à terme à une soumission des services d'enquête Parquet Police au pouvoir exécutif le secteur souffre d'une crise des vocations, il ne parvient plus à fidéliser ses agents, la réforme va accentuer le phénomène de départ et la perte d'attractivité de cette vocation. Monsieur Ménard Roche madame De Lattre, madame la présidente, vous avez la parole. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement fait donc écho aux inquiétudes des acteurs de la PJ quant à l'exercice de leur métier, mouvement soutenu par les magistrats instructeurs tout aussi préoccupé par l'avenir de la filière judiciaire, le choix de bâtir un dispositif sur le département, donne le sentiment d'un abandon de l'investigation zonal interdépartementales et interrégionales, voire international, au bénéfice de la seule gestion des affaires courantes, monsieur le Ministre, j'ai lu avec grand intérêt votre interview dans le JDD, où vous dites que les affaires liées à la criminalité conserveront la même organisation qu'aujourd'hui que la cartographie restera la même, que les magistrats pourront continuer à saisir le service enquêteur de leur choix, alors pourquoi ne pas proposer d'amender votre rapport ou en attendant de réécrire les alinéas concernés de les supprimer, puisque ces derniers sont devenus caduques par vos propos rassurants pour que le dialogue soit réinstaurée plus facilement merci. Merci, chers collègues, nous passons à la présentation de l'amendement 179 il est présenté par Madame Assassi. Qui n'était pas du tout. Bon je je crois que j'ai défendu à plusieurs reprises cet amendement en fait en évoquant notre proposition de loi sur la police de proximité, donc on peut considérer qu'il est déjà défendu. Merci madame la présidente et nous passons 133 Monsieur Bénard. Oui, cet amendement est présentée par mon collègue monsieur Breuiller il est défendu par tout le groupe, il a pour objet de maths fait à à une incohérence, je parle à sa place à à mon collègue monsieur brouillés à laquelle j'ai souvent été confronté comme maire Daniel Breuiller a été longtemps maire d'Arcueil lorsqu'on interroge les forces de l'ordre sur leurs modalités d'intervention, elles mettent parfois en avant la suffisance d'effectifs, or les élus locaux. Non, pas ou peu d'informations sur les moyens humains attribué au commissariat ou à la gendarmerie dont ils dépendent et cela peut créer l'impression que certains territoires sont plus douter que d'autres l'objet donc de cet amendement est de fournir aux maires 2 informations : d'une part, pourrait précis et régulier sur les effectifs affectés au commissariat ou à la gendarmerie dont il dépend, d'autre part, les critères objectiver prévaloir la répartition des forces de l'ordre sur le territoire national, ces critères existent sans aucun doute, on imagine mal une répartition aléatoire des forces de l'ordre leur publication aux élus, permettra de mieux appréhender les modalités de répartition et d'en débattre, le cas échéant. Madame la présidente, monsieur le Ministre, nous sommes sur la même difficulté et je crois qu'il y a unanimité sur le trouble qui atteint un certain nombre de professions, notamment les professions judiciaires dans un rapport qui est annexée à une loi, certes importante, mais ça reste un rapport annexé, on aurait pensé que pour un sujet de cette importance bien, nous aurions eu une loi. Voilà. Complète parce que le sujet est d'importance, on risque de porter atteinte à la séparation des pouvoirs tels qu'il est prévu dans nos dans nos démocraties représentatives et je pense que je partage la la vie de mon collègue, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul sur ce texte et cet avenant, il a pour but non pas de s'opposer définitivement à la loi qui a par ailleurs de grande qualité mais de faire en sorte que le doute qui subsiste sur l'organisation du rapport de la police judiciaire avec le pouvoir exécutif. exécutif. Me semble-t-il, de demander au moins un report et une étude d'ailleurs, j'ai cru noter que lors de le l'étude des amendements. Ces amendements avaient été préservés, c'est le n'aime le terme qui et que donc on n'avait pas pris du côté de la commission un avis définitif sur la question. Oui monsieur Favreau, monsieur le rapporteur, avis sur l'ensemble de ces amendements. sur l'ensemble de ces amendements. Tout le temps, mais je suis dans un état provisoire de mobilité restreinte, merci de votre compréhension mais je vais me lever sur ce sujet très important pour rappeler la position de la commission. D'une part la départementalisation de la police qui est envisagée par le ministre dans une réforme importante. Il se trouve que mon père était fonctionnaire de police, je l'ai entendu parler de cette réforme en mille dans les années 1990 c'était monsieur Joxe, qui était ministre de l'Intérieur. Un grand ministre. Et. à l'est de nature réglementaire, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain le ministre exprime. Le fait que ils pensent que l'organisation par filière ou en Momcilo comme vous voulez, de la police nationale, pose des problèmes en terme d'efficacité qu'il est souhaitable de dettes départementaliser de toute une série de Cécile silos pour une meilleure efficacité et une meilleure gouvernance. Nous nous disons, et la commission a dit clairement que, il y a une spécificité de la police judiciaire. Qui. Qu'il faut tenir compte de cette spécificité, j'ai été encore plus clair dans la discussion générale puisque, j'ai dit cela suppose que nous exprime clairement que, premièrement, la police judiciaire doit rester sous l'autorité du procureur. ça va sans dire, mais c'est bien de l'écrire, deuxièmement, que la police judiciaire doit garder toutes les affaires sensibles. Parce qu'on voit bien que si ah mutualisation des moyens, ça peut être.

des créations peut être zonal, qui permettrait d'avoir une vision plus générale sur toute une série de filière, on pense en particulier aux filières de délinquance relatives à la drogue. J'ai dit à mon collègue Jérôme Durain et à ma collègue bé lurons qui sont en charge de par la volonté du président François Noël Buffet d'une mission d'information que c'était à ce stade, sans préjuger des une idée des de de ce que va dire la mission les orientations que nous ne pouvions apporter mais que si j'allais plus loin comme votre rapporteur je préjuger des de de ce qu'allait dire cette mission qui fait des auditions. évidemment que nous en avons fait nous-mêmes des auditions, on a entendu je, je le dis parce que les collègues, je viens de citer monsieur Durin qui assisté à toutes les auditions et et des autres groupes, donc, vous avez entendu ce qu'on dit, la conférence des procureurs, vous avez entendu ce que dit le le barreau, vous avez entendu ce que disent certains responsables de la police judiciaire, on en a aussi auditionné le directeur de de la police judiciaire d'Île-de-France qui dit que lui, ça pose pas de gros problèmes, enfin on a toutes les opinions là-dessus. Mais il y a une mission d'information, j'ai dit à mon collègue du hein, si vous voulez, mais c'est, c'est eux qui sont rapporteur de cette mission : aller plus loin, à écrire les quatre choses que je viens de vous dire ou d'autres, c'est eux qui sont au stade où ils en sont, on pourrait prendre à l'amendement. Mais là, vous nous dites : il faut. Enlevé le terme du rapport, alors c'est un rapport d'orientation et que l'un des axes majeurs de la gouvernance future qu'envisage le ministre, c'est cette réforme de la départementalisation, vous nous dites, faut aller plus loin, supprimer la départementalisation j'ai, moi de vous dire, ce n'est pas la position de la commission, la commission a dit que on laissé sert plus, c'est du domaine réglementaire mais que il fallait tenir compte des spécificités de la police judiciaire. Et moi je dis ça suppose des choses très claires sur l'autorité très clair du du du procureur lors lors lors des enquêtes ou du juge d'instruction lors des enquêtes préliminaires, en particulier, ça suppose des choses très clair sur le fait que les affaires sensibles resteront exclusivement du du ressort de la police judiciaire, ça suppose des choses très claires sur la manière dont on dont on enjambe la limite départementale pour faire face à la délinquance organisée, en particulier des différents trafics, prostitution Rafic de voitures et trafic de drogue, voilà moi j'en suis là et donc sur la position de la commission, je, je, je dois refuser les amendements madame Assassi et elle a fait un complément d'amendement revenant la police de proximité, mais je dirais le raisonnement est le même, même si elle a, elle, fait un ajout et le dernier amendement, et il serait bon que les maires Fust informé de tout cela quand on mettre en place des des modifications de structure de gouvernance au ministre qu'il appartient de dire les modalités selon lesquelles il va informer les maires, mais dans ce qu'il a dit : j'ai entendu que de toute manière il tiendra informer les maires, mais à ce stade, j'entends que vous demander un scrutin public. Je dois donner un avis défavorable sur tous ces amendements pour autant pour autant la position de la commission et de dire que nous prenons acte de la volonté du ministre de faire sept départements lundi à 0 virgule, sous réserve des spécificités de la police judiciaire et dans l'attente des conclusions de la mission d'information qui a été demandé par le président de la commission des lois.

enfin franchement, on va avoir ça va partir à l'Assemblée nationale, ça va revenir dans une navette, il va y avoir une CMP d'ici là, je pense que la mission Durin va nous dire un certain nombre de choses et moi compte tenu, ce que je vous ai dit et compte tenu, ce que je vous ai dit publiquement, nous pourrons adopter un certain nombre d'amendements complémentaires mais au stade où nous en sommes, je dois vous redonner cette position là, parce que ce ne serait pas ni cohérent ni en phase avec ce que la commission a voté de vous dire autre chose, je suis obligé d'être défavorable à ces amendements. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci madame la présidente, bon c'est une question très importante, elle mérite effectivement qu'on qu'on s'y arrête. Quel est le constat parce que là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que personne ne parle du constat, bon, le constat c'est que nous avons. Une augmentation de la délinquance, que tout le monde vient à dénoncer. Et les taux d'élucidation qui sont. Nullement en baisse sur une délinquance la plus haut du spectre comme on dit, je pense notamment aux homicides. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce constat. Peut-être que nous sommes mal organisée, ça tombe bien : 7 rapports sénatoriaux depuis le ministre-Geox. Qu'il y a pas de ma famille politique qui a eu le 1er, l'idée de cette réforme. Ont conclu les sept. Et je ne parle que des rapports sénatoriaux, je ne parle pas des très nombreux rapports de la Cour des comptes, je ne peux pas des rapports de l'Assemblée nationale, je ne peux pas les témoignages de très nombreux spécialistes de la spécialité. Que l'organisation en silo de la police nationale était une mauvaise chose. Alors c'est très drôle parce qu'en plus, je me suis entre guillemets pour les biens de notre débat public intéressé à qui était l'auteur de ce rapport, le 1er rapport qui faisait suite à la proposition de Monsieur Joxe, c'était un sénateur RPR Monsieur Lucien Lanier. Rapport de 30 mai 1991. Puis on a eu un rapport de monsieur Evry Montesquieu, donc là c'est un sénateur radical qui dit que c'était la même chose, un rapport de monsieur Van der donc. der donc. Socialistes qui dit exactement la même chose, un rapport de monsieur. Qui dit quand même chose qui maintenant est tellement éminent juristes qui siège, me semble-t-il, au Conseil constitutionnel et je pourrais multiplier puisque j'ai évoqué, monsieur Bouton il y a pas si longtemps que ça faisait partie du groupe socialiste. Et de monsieur Grosdidier qu'a pas si longtemps que ça faisait partie du groupe UMP LR. Les 7 rapports disent cette fois la même chose. Et là, monsieur le sénateur, je pense qu'il faut arrêter de relayer des faits que nous si vous le permettez. C'est vraiment très insultant de dire que c'est attentatoire à la séparation des pouvoirs, ça veut dire que la gendarmerie depuis 2 siècles, vit en totale concertations avec ce que nous faisons un tendon d'une d'un état démocratique. Que la préfecture de police ne serait pas démocratique. C'est le contraire, la direction générale de la police nationale et la seule des 3 force à être organisé comme ça, donc arrêtons de dire des choses inexactes, d'autant, monsieur le sénateur que rien n'est législatif est-ce que vous pensez un seul instant que si la réforme de la police nationale venait à toucher le fonctionnement démocratique du pays, nous pourrions le faire qu'avec des règlements et des arrêtés. Pas une mesure législative, l'article 12 du code de procédure pénale est entièrement respecté, le magistrat a libre choix du service en scooter, il sera entièrement respecté la police judiciaire. Pardon de vous décevoir, je ne vous suffit pas, Monsieur le Président, sur, j'en suis fort désolé. Mais la police judiciaire est un service du ministère de l'Intérieur, il y a c'est vrai des discussions. des six discussions Monsieur le sénateur sueur pour dire qu'il faudrait que la PJ, soit auprès du ministère de la justice connaissez ces débats comme l'administration pénitentiaire doit être auprès du ministère de l'Intérieur, on peut s'amuser effectivement à des changements d'organigramme mais c'est pas l'objet de la réforme puisque ça a toujours été un service du ministère de l'Intérieur et j'espère que ça ne sera, mais, mais, monsieur, mais monsieur Sueur, vous êtes trop fin juriste, cette reconnaissance ces questions pour pas être vous-même pas convaincu par argument 90 pour 100 des enquêtes judiciaires, c'est la sécurité publique. C'est vous, commissariat, choisi par les procureurs de la République 90 pour 100 des enquêtes judiciaires, c'est les commissariats de France, la police judiciaire, c'est 10 pour 100 des enquêtes judiciaires, donc il faudrait qu'à tout moment, monsieur le garde des Sceaux puisse répondre à vos questions. Alors, on la vit très bien volontiers : il est le bienvenu, bien évidemment, mais je pense qu'il ne faut pas non plus voir dans la réforme de la police nationale, ce qu'elle n'est pas elle n'est pas un changement de statut. De la police judiciaire, elle n'est pas la modification des Liens entre magistrats et un service mis ça d'ailleurs que la police judiciaire, elle n'est qu'une modification réglementaire et elle n'est qu'une petite partie de la réforme de la police nationale, mesdames et messieurs les sénateurs, vous avez déjà accueilli. Le président de la République ou la première ministre parfois mise intérieur sur un tarmac d'aéroport par exemple qu'est-ce qu'on y voit. Pressé. Un patron de gendarmerie et 4 policiers. Mais jamais fait cette réflexion. Il y a un préfet. Il y a un gendarme et il y a 4 policiers, ils vous disent bonjour, je suis le directeur départemental de la sécurité publique après oui bonjour, je suis directeur départemental de la police aux frontières après il me dit bonjour monsieur, directeur départemental de territoriale, bon, je vois bien que physiquement qu'il y a un problème. Non, mais parce qu'aujourd'hui, la délinquance, mais tout le monde le sait, c'est pour ça que monsieur Joxe avait cette idée de bon sens et qu'elle est évidemment très difficile à mettre en place la délinquance aujourd'hui encore plus qu'aux années 90 elle est multiforme. Et que c'est pas qu'une question de sécurité publique et que c'est pas qu'une question de police aux frontières et c'est pas qu'une question de renseignements tout ce monde doivent travailler ensemble, ce que font les gendarmes unicité de commandement ce que fait la préfecture de police unicité de commandement et si on perd du temps dans les zones de police, c'est parce qu'on fait parfois des protocoles entre services de police je suis atteinte d'une administration qui fait des protocoles entre directeurs dans les mêmes services, d'un même ministère pour savoir s'ils peuvent se passer des informations. très franchement je. C'est c'est pas renverser la pyramide de Kelsey dans ce que je raconte c'est extrêmement pragmatique, pragmatique et tout le monde s'en est absolument rendu compte d'ailleurs, l'immense majorité des syndicats de police sont favorables à cette réforme depuis très longtemps, alors qu'il y ait des interrogations, moi je suis prêt, monsieur le rapporteur. à amender l'amendement proposition ne soit pas un amendement de suppression, sinon ça n'a pas de sens, est ce que vous voulez qu'on mettrait dans le texte de loi, même si ce n'est pas logique. Natif que nous allons laisser aux magistrats Libre instruction et le libre choix des services, moi je suis d'accord, si c'est pas obligé de la réforme est ce que vous voulez qu'on écrive, monsieur le rapporteur, que, il y a pas un policier de police judiciaire 5000 policiers et judiciaires sur 150000 policiers. Dont 2500 à la RPP ah la la, direction, pardon, de la préfecture de police, donc 2500 qui ne sont pas concernés par la réforme donc sur les 150000 policiers, nous parlons de 5000 agents tout à fait respectable, évidemment, sur 5000 M hein Jean il y en a 2500 qui ne sont pas concernés puisqu'ils sont déjà dans la réforme puisque vous à la préfecture de police, donc on parle de 2500 sur 150000. Est-ce que pour les rassurer, vous le souhaitez, tout ce que nous mettons ce que j'ai écrit il y a pas un policier de PJ qui fera autre chose que la la PJ pour des enquêtes au du spectre, je suis d'accord pour qu'on arrête, est ce que vous souhaitez, monsieur le rapporteur, et je dis à à chacune et à chacun, ici, qu'on dit ce que tout ce qui concerne la délinquance financière et la probité des élus, ce ne soit pas avec nous à l'échelon départemental mais régional ou zonal, je suis d'accord est-ce que vous souhaitez qu'on dise qu'on ne changera pas la cartographie, il y aura toujours des offices, les mêmes toujours des antennes régionales, les mêmes, je suis d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on voit que, il y a une délinquance qui augmente. Un taux d'élucidation qui baissent à la direction générale de la police. Finale parce que les services fonctionnent comme effectivement du temps de Clémenceau, j'aime beaucoup Georges Clémenceau.

le délibératif du rapport annexé, monsieur le sénateur, c'est pour respecter le Parlement, de dire ce qu'on va faire, mais ça n'a rien législatif, effectivement, on aurait pu pas le mettre mais j'ai préféré être honnête vis-à-vis du Parlement. est drôle de ministres que de présenter une grande réforme. Sans la mettre dans son rapport d'orientation donc avouer que, au moins nous avons grâce à ça, ce débat. Et ce qui me permet de vous dire monsieur le Direct,

J'ai été ministre des Comptes publics lorsque votre gouvernement monsieur Sueur courageusement à fusionner la comptabilité publique avec administration fiscale et on avait les mêmes grèves, on avait les mêmes manifestations et on a dit : oh la la, le préfet, il va connaître les contrôles fiscaux ou la là tout le monde va arrêter de faire des contrôles fiscaux, parce que, parce qu'évidemment on n'a pas envie de sanctionner et on fera que l'aide aux collectivités locales, hou là là, ce sera pas le même métier, qui se plaint aujourd'hui la direction générale des finances publiques. Qui aujourd'hui ne voient pas que c'est une admiration moderne qui prend en compte les difficultés des autres tant que le contrôle fiscal il était multiforme et le préfet, j'ai été trois ans ministre des Comptes publics, il y en a eu d'autres ici ne commente pas les contrôles fiscaux sur les élus sur telle ou telle chef d'entreprise et le secret fiscal plus que secret d'instruction, tout le monde aujourd'hui est très heureux de dire oh là le secret de l'instruction, tout le monde s'intéresse au secret d'instruction, c'est une très bonne chose parce que ça me pas sauté aux yeux, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, mais en tout cas, je peux dire que le secret fiscal est absolument garder. Et le préfet n'est pas au courant des contrôle fiscal que fait le le le l'agent fiscal, même le directeur des finances publiques départemental n'est pas au courant de ça, vous savez très bien, donc je ne vois pas objectivement ce qui empêche en effet. En fait, moi je suis tout à fait d'accord avec le rapporteur, de compléter l'orientation de la réforme, mais de grâce, ça fait 35 ans quasiment, que tout le monde essaie de faire cette réforme, qu'il fallait rassurer je pense que j'ai multiplié les signes positifs ni nous n'y voyons pas. pas. Mesdames et messieurs les sénateurs, une atteinte à la démocratie, là où il y a une efficacité des services parce que la vraie atteinte de la démocratie, c'est pas d'expliquer aux personnes. Comment, enfin, pardon, c'est de ne pas savoir, explique personne qu'on arrive pas à retrouver l'auteur d'un homicide, ça c'est une atteinte à la confiance démocratique notre régime de de d'expliquer qu'il faut faire des protocoles entre services de police et de perte du temps quand on fait des écoutes téléphoniques ou quand on fait des filatures, ça c'est une atteinte à mon avis à notre amour de la démocratie et du respect de l'État de droit, donc encore une fois aucune disposition législative, ce qui est la démonstration par l'absurde la preuve du pudding, c'est ce qui se mange qu'a pas de changement dans nos rapports avec la justice, aucun. Je pense vous dire, redire devant la Haute Assemblée, je suis même prêt à amender les amendements qui évoque, qui n'évoque pas la suppression du service, il y a jamais eu autant, monsieur le Président, sueur, de gens qui s'intéressent à cette réforme, que dans ce que je propose, démocratiquement, il y a un rapport de l'IGA de l'IGPN et j'ai proposé que Lee Gigi l'inspection des services judiciaires face le rapport sur l'évaluation. Service de la police nationale avoué que on pourrait tout de suite m'ont dit que ce serait bien aussi qui ou IGGN face parfois des rapports avec l'inspection de la justice, ce sera une qualité très. Bon pour qu'il puisse être rendu ce rapport monsieur Sueur sera rendu public et je discuterai avec une réunion syndicale, et madame la sénatrice faut également, rapport à l'assemblée pareil. Alors, à moins qu'on n'ait pas envie de faire la réforme et dans ces cas-là, il faut le dire, il faut dire que on veut que la PJ soit rattaché directement au ministère de la justice, il faut dire que ben oui, il y a des taux d'élucidation en baisse et on propose autre chose, mais que proposez-vous, d'autres où il faut dire que peut-être Monsieur Joxe, comme les 7 rapports parlementaires se sont trompés depuis 35 ans c'est toute c'est tout à fait possible mais dans ces cas-là, il faut vite qu'on sentait que s'intéresse à savoir comment fonctionne la gendarmerie nationale et comment fonctionne la préfecture de police, donc bien sûr c'est une habitude à changer, j'ai le plus profond respect pour les policiers de la police judiciaire, monsieur le sénateur, je ne partage pas votre opinion parce que je pense que quand on manifeste, on manifeste pas cagoulés ou masqués dans des services locaux de police, mais ça c'est une autre façon d'imaginer les choses, donc il y a bien sûr des contestations, des tracts, des grèves et c'est tout à fait normal, mais il y a des limites quand on est la police de la République, moi je pense que c'est mon rôle de chef que de le dire, et indépendamment de ça, je suis prêt à faire la réforme non pas au forceps mais on écoute simplement au bout de 35 ans, discussion, je pense qu'on peut conclure. Monsieur le ministre, monsieur Sueur, vous avez demandé la parole pour explication de vote. C'est difficile, hein, parce que Monsieur le Ministre, expliqué non pas son vote mais sa position pendant 12 minutes. Donc on va voir un 6ème du temps pour dire très de manière lapidaire : premièrement, que monsieur le rapporteur, nage dans la contradiction, tout le monde comprend que il nous dit que la commission des lois, est en train de faire un rapport pour savoir s'il faut ou s'il ne faut pas aller dans une réforme, une de la police judiciaire dont on ne sait pas, il y a pas de position de la Commission, sinon de travailler sur le sujet, et vous dites, mais il faut néanmoins marqué dans le rapport qu'il y aura le rattachement de la police judiciaire au directeur départemental alors vraiment c'est incompréhensible si on fait un rapport pour étudier, on ne doit pas affirmer une position qu'on ne peut pas affirmer, puisque le rapport n'a pas été remis 1er point deuxièmement Pierre Joxe, alors je connais bien perd Joxe, il a beaucoup parlé de la police et de réforme de la police, mais voyez-vous, je ne pense pas qu'on puisse. Aller rechercher dans les actes, tous les propos de Pierre Joxe, quelque chose qui portait qui porterait atteinte, si peu que ce fut à l'indépendance de la justice à l'indépendance, mais vous dites cela, c'est votre position, je ne pense pas que vous puissiez enrôlé Pierre Joxe dans cette opération et enfin Monsieur le Ministre, naturellement, vous avez beaucoup de talent, je le reconnais mais alors que nous vous disons et sincèrement. Nous, nous pensons que vous auriez intérêt à accepter notre amendement pour retirer ses quatres lignes ce qui serait le signe par rapport aux policiers de la PJ que finalement il y a un dialogue que ce n'est pas terminée, et alors vous nous dites : mais non, on ne va pas faire ça, oh, on peut amender pour ajouter : dopage,

qu'est-ce que vous voulez, on ne va pas aller dans ce sens mais enfin ce serait perçu comme une véritable provocation que d'ajouter de pages alors que Monsieur le Ministre, nous avons parlé parlé dans l'intérêt du gouvernement et je pense que vous serez, vous y serez sensible, madame la présidente. Merci monsieur le questeur, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Je voudrais redire les choses clairement, sur le calendrier, après les explications que vient donner Monsieur le Ministre. Au stade où nous en sommes, on aurait pu en amont, je le redis, rajouter non pas de pages monsieur Sueur quatre lignes très claires. Oh à l'amendement du Rhin qui quelque part a pris rendez vous a pris date en disant : laissez-nous faire notre mission d'information. D'ici, la commission mixte paritaire les conclusions principales de cette mission d'information seront connus, moi je m'engage ici après à vide mon président parce que c'est la logique de la commission, à ce que, à la commission mixte paritaire, nous défendions une rédaction qui n'est pas la rédaction actuelle mais qui tiendra compte parce que le ministre dit des choses et c'est normal, il est dans son rôle mais le le la mission d'information fera des préconisations, le président là faut le fera sans doute voté en commission et moi je peux rajouter un certain nombre de choses qui prendra acte des principales conclusions de la mission et nous défendrons cette position en commission mixte paritaire, mais si nous prenons vos amendements tels que vous les faites ça veut dire qu'on supprime du texte, la départementalisation est-ce que c'est moi de vous dire, ce n'est pas la position de la commission position de la commission et de dire : nous voulons qui est lié de manière plus claire dans la rédaction, la prise en compte de la spécificité de la police judiciaire. J'ai été encore plus clair puisque j'ai dit les 3 ou 4 choses qui me semblait fondamental et qui est d'ailleurs, pour être clair, recoupe ce que je nous avons entendu dans nos auditions venant en particulier du monde judiciaire, mais pas que et donc moi je je prends cette position et je jeudi devant mes collègues, nous défendrons ah mais, sinon, à quoi sert qu'on fasse des missions d'information. et pourquoi les parlementaires vont travailler pendant des jours et des jours et auditionné parce que le ministre a sa position et il fera les les avancées qui qu'il croit devoir faire, il est dans son rôle, mais nous, notre rôle c'est de faire des propositions qui garantissent des choses. Et je dis : nous devons garantir que la police judiciaire, mais il vient de le dire, si vous voulez un amendement qui dit qu'on garantit que ces reste sous l'autorité judiciaire, je suis d'accord si vous voulez un amendement qui garantissent que les affaires sensibles restent du domaine de la police judiciaire, je suis d'accord si vous voulez un amendement qui disent que, pour la criminalité ou la délinquance organisée, il faut qu'on dépasse les les frontières et que vous trouvez des structures appropriées, je suis d'accord, j'ai entendu dire ça, je suis comme vous, comme moi, donc moi je vous dis, il y aura 3 ou 4 phrases n'ont pas de pages monsieur sueur que que nous demanderons en amendement au moment de la mixte paritaire parce qu'autrement je préempte. Les résultats de la mission d'information et je suis désolé, ce ne suis pas dans mon rôle de rapporteur de la commission des lois. Merci. Monsieur Debré, la parole est à madame De Lattre, madame la présidente. Oui merci madame la présidente, chers collègues, je vais retirer mon amendement parce que je pense que compte tenu des manifestations et des amendements qui sont des amendements d'appel, nous avons été entendus et que les propos rassurants du du ministre- mais aussi des engagements de notre rapporteur dans la suite du du du processus sont de nature aujourd'hui à à nous permettre d'avancer sur cette question et d'avoir pu faire écho des inquiétudes et de faire largement avancer le débat, donc je je retire mon amendement merci. Merci, cher collègue alors ah Monsieur Monsieur Roche, explications de vote. la contradiction effectivement, me semble-t-il, du rapporteur je partage 100 % de ce qu'a dit Jean-Pierre Sueur en fait dans dans la réalité, on dit à la fois aux crée une mission d'information parce qu'on se pose des questions. Sur le rapprochement, mais en mais en même temps on préempte j'utilise les mêmes mots que vous en prie préempte les résultats de la mission d'information en laissant quand même ce rapprochement dans le texte, sans vouloir lamenter et sans vouloir le supprimer, pour l'instant donc la option est plutôt là, moi je la vois plutôt là, et en hommes et en même temps, monsieur le rapporteur, vous dites par ailleurs c'est une orientation générale du ministère et donc on n'a pas à discuter de ces augmentations ben alors je me demande pourquoi on fait des amendements depuis tout à l'heure sur le débat et sur le rapport de 4 à 6 pages alors du fait que ça depuis tout à l'heure, on a effectivement une orientation et en discute des éléments de cette orientation et on a même voté des amendements qui remettent pas fondamentalement les orientations principales parce que ça ce serait compliqué, même si on les met quand même nous en en en en, on ne va pas dire à défaut mais on les met en question et donc là c'est pareil, là il y a un élément principal de l'orientation que nous ne partageons pas voilà et

telle qu'elle est prévue par ailleurs, je rappelle que énormément d'acteurs y sont opposés et que nous avons aussi à signale alors à donner que ce signal, il va pas être donné en rajoutant 4 conditions et pour terminer, je dirais simplement à monsieur le Ministre. Attendez Darmanin que ils n'étaient pas cagoulés, les policiers, ils étaient. Qui et je on a les vidéos et cetera, il était pas particulièrement menaçant, je comprends qu'il puisse être sanctionné, c'est pas de ma responsabilité et c'est de la vente et je l'accepte volontiers mais il était pas cagoulés voilà. Merci, cher collègue, monsieur le ministre. Peut-être pour revenir sur ce qu'a dit Monsieur sur parce que je peux pas lui, c'est dire que ça porte atteinte quoi que ce fût à l'indépendance de la justice encore une fois, monsieur le président de la commission des lois, vous ne pouvez pas dire ça sans sans faire que de la politique et je vous connais trop, je sais que vous n'en faites pas. ce serait sans doute tromper et tromper les gens qui nous écoutent et il ne faut pas tromper les gens qui nous écoutent, encore une fois, il n'y a aucune modification législative. Dans la mise en place de la réforme de la police nationale. Et vous savez mieux que personne que si nous devions toucher les rapports entre les magistrats, l'autorité judiciaire. Et les forces de l'ordre, ce serait forcément du législatif, donc je crois que la démonstration, une nouvelle fois qu'il n'y a pas de modifications dans les rapports. Entre l'autorité judiciaire et les services qui sont coup courant du ministère de l'Intérieur, c'est que je n'ai besoin d'aucune disposition législative pour créer la police nationale, nouvelle formule, comme la gendarmerie comme l'ATP, et là, jetons départemental donc franchement, soulignons-le et rossignol. Deuxièmement, on ne peut pas dire et j'ai entendu de votre part, aucune proposition, personne ne fait une autre proposition que celle que je propose, mais c'est normal parce que c'est pas la mienne, ça fait 35 ans que monde propose la même. Nous avons des homicides. De moins en moins résolu une délinquance de plus en plus multiforme de plus en plus complexes, de plus en plus internationale. Notamment des stupéfiants ou la délinquance financière qui s'était certes c'est terminé, les gangs à la papa, qui sont désormais. Extrêmement complexe, extrêmement technologisée et nous avons une filière. Investigations dont tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont en souffrance et qu'elle est pas assez efficace. Par manque d'énergie, de la part des pouvoirs publics pour la remotiver. Donc, une fois qu'on a fait tous ces constats, je viens avec la proposition que font une grande partie de mes prédécesseurs et la haute assemblée et j'ai montré à quel point c'était éclectique dans ses propositions que j'ai entendu, en général, on me répond : vous avez raison, monsieur le ministre, il faut rien changer, ben, je suis désolé, c'est pas ça la politique, donc si on est d'accord pour dire que les homicides, ce sont en augmentation que trafic de stupéfiants sont de plus en plus complexes qu'ils pourrissent la vie de nos concitoyens que les sudation n'est pas au rendez-vous et que l'investigation est en souffrance, il faut en tirer des conclusions. Alors moi je vous donner parfois la situation absurde dans laquelle on peut se trouver, mais ça c'est la réalité du quotidien dans 2 affaires d'il y a quelques jours, je ne donnerai pas les noms évidemment pour le secret d'instruction, une enquête, faire la fête, la PJ et une enquête fait par une sûreté départementale,

dans un territoire du sud de la France, la Sûreté départementale, c'est-à-dire ce qui relève des 90 % la direction de la sécurité publique, elle fait vingt-et-un kilos de saisie de drogue et 3 écrous sur 2 affaires de drogue différentes dans 2 départements différents, comment peut-on dire aujourd'hui. Qu'il y a d'un côté, la PJ qui ferait que l'eau du spectre et là, des CSP la sécurité publique, qui ne ferait que ce que j'ai entendu le petit judiciaire, ce serait d'abord c'est insultant envers les 90 % d'enquête saisis par les policiers de sécurité publique et on voit bien que ce qui était vrai sans doute il y a 40 ans n'est plus vrai aujourd'hui, c'est tous les jours que dans des commissariats de France désormais ont fait des dizaines de kilos de cannabis des tentatives d'homicide des homicides. Et que les officiers de police judiciaire ne sont pas formés ou accompagné de telle sorte que il soit dans une chaîne judiciaire qui leur permettent effectivement de bénéficier de la technologie des échanges internationaux, des informations de la formation de leurs camarades de la police judiciaire qui sont effectivement des policiers très qualifiés. enquêteur de police judiciaire en France, il y en a 5000 de la PJ en là 15000 dans les commissariats aujourd'hui la PJ c'est 5000 personnes demain avec la réforme, ce sera 20000 personnes parce que la réforme que nous proposons et qui est proposé depuis très longtemps, ce n'est pas d'appauvrir la police judiciaire, en lui retirant ses 5000 enquêteurs s'est donné 15000 enquêteurs qui dépendent de la sécurité publique à la filière judiciaire. Parce qu'en plus l'OPJ qui rentre dans un commissariat. Bien sûr qu'il fait du petit judiciaire comme on dit, et personne, mais ça viendrait à l'idée de personne de mandat des grands enquêteurs des brigades très spécialisés. Tu allais faire des violences intrafamiliales dans les commissariats, mais ça n'a rien d'infamant on enfin on je pense que tout le monde raconte. Prix que c'était pas discours que je portais depuis très longtemps, en revanche, qui est très intéressant c'est quand l'OPJ particulièrement dynamique et capable de repérer que le point de deal et le CHUV qui à côté de chez lui, il est en lien peut-être avec un réseau plus important et on peut s'évertuer mesdames et messieurs les sénateurs à mettre autant d'effectifs de police que vous souhaitez, si c'est pour arrêter que les détaillants jamais les grossistes on peut mettre beaucoup d'effectifs de police pendant très longtemps,

et malheureusement nous constatons aujourd'hui que. Ce que vous avez peut-être connu dans des services de police ce différend a beaucoup changé parce que la délinquance elle s'est beaucoup transformée, alors après il y a 2 solutions, monsieur le sénateur sueur. Mais je vois que vous ne me suivez déjà plus, bon, il y a 2 solutions, parce que c'est une question très importante. Soit vous considérez que vous êtes contre la réforme, pour des raisons politiques, est ce que je peux très bien comprendre puisque nous on de la politique dans ces cas là, effectivement, les possibilités de modification d'amendements et d'explications de mission sont un peu vaine, soit on considère que c'est une réforme qui, depuis 30 ans, a essayé d'être tuer par tout le monde, dans des conditions sans doute difficile et j'aurais sans doute plus attends les élections professionnelles pour la faire parce qu'il y a des élections dans un mois, évidemment dans la police nationale, comme partout dans la fonction publique, mais comme j'aime bien faire des choses qui me paraissent conformes à l'intérêt général, je propose cette réforme que nous discutions depuis un certain temps et on accepte d'évaluer concrètement, comme le dit monsieur le rapporteur. Les des TPN qui existe déjà en territoire ultramarin, d'ailleurs il n'y a pas un procureur général qui explique le contraire lorsqu'il a vu ce que c'était le direction unique de la police nationale ou les 10 départements qui ont été expérimentées en métropole, vous avez ici des sénateurs qui connaissent cette expérimentation dans leur département. Et nous avons de mission parlementaire et moi je fais une proposition : président de la commission des lois, quand on aura le rapport. De l'Gigi de l'IGPN et de l'IGA je viendrai s'ils m'invitent, comme je l'ai fait. ça demande vous le présenter le rende public et il sera encore temps évidemment de à certain nombre de choses puisqu'encore une fois, ce n'est que réglementaire et dans ces cas-là, si c'est une question d'amélioration, je je suis devant vous et je vous dis, modifiant la maman pour mettre toutes les conditions que vous évoquez. Et vous ne leur prenait pas au bon, j'ai dû, je pense qu'au bout d'un certain nombre de discussions votre envie et plus d'embêter le gouvernement que de réformer la police nationale. Merci, monsieur le Ministre, alors je pense que nous allons pouvoir maintenant procéder au vote en commençant ah pardon, monsieur Kader. madame la présidente, monsieur le Ministre de l'intérim a mis le doute dans l'esprit et donc j'ai été regardé quelques archives sur la fameuse réforme Joxe porté par monsieur Marchant porter ensuite par monsieur qui laisse est annulé en 93 par monsieur Pasqua. Je tiens à le préciser et cette réforme portée effectivement sur une territorialisation non pas des 4, police et deux 3 police la police aux frontières, la sécurité publique et les Renseignements territoriaux, la police judiciaire n'a jamais été intégré dans les rapports que vous évoquez, depuis tout à l'heure monsieur le Ministre, je voulais quand même le préciser, la police judiciaire n'a jamais été évoquée dans les réformes portées par les gouvernements socialistes de l'époque, voilà pour l'histoire commune de chacun. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Alors Monsieur Monsieur Kader, pardon, mais vous avez vous-même dit qu'il y a eu plusieurs ministères qui se sont succédés et que celle qu'imaginait par monsieur Joxe, je vous renvoie à son discours de 1000 900 89 n'a effectivement pas été celle de monsieur Marchand et il se peut que parfois certains ministres ne porte pas les autres, même dans la même couleur politique, c'est tout à fait possible voilà et je vous je trouve. Bien bien énergique pour désormais l'héritage, je ne me suis pas ce quoi puisque aujourd'hui vous êtes finalement dans la même position que monsieur Pasqua, par un retournement, l'histoire, voilà qui sans doute fait que avec expérience sans doute on se droitise

Bouton de 2018, c'est quand même, il y a pas si longtemps que ça, hein, qui évoquait lui-même l'unification départemental. Le plafond. Je veux je veux je veux non mais je, je sais que j'ai très bien connu Monsieur Joxe Monsieur Marchand, c'est sûr, mais ce que je veux dire c'est que, oui, très bien bon monsieur, monsieur, monsieur le président, sur notre difficulté, encore une fois c'est est-ce qu'on discute sur des arguments qui fonde la discussion d'intérêt général Keller me connaissait bien pour savoir que je peux très bien aussi faire de la politique de mauvaise foi, je crois que nous connaissons ce sujet. Donc ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi une insulte, hein, je je voudrais le préciser, ce n'est pas une attaques à nominem soit nous considérons que nous discutons d'un sujet très important pour la nation. Et la sécurité de nos concitoyens et je veux bien souligner que cette démarche n'est pas du tout médiocre de la part de tous ceux qui interviennent et j'entends les interrogations légitimes d'une très grande partie de jeu, de gens qui aujourd'hui se pose des questions et nous avançons pour encadrer la discussion. ça fait trois fois mesdames et messieurs les sénateurs, que je vous propose d'amender moi même la réforme que je vous propose ne peut pas dire mieux en mettant les critères, parce que vous m'accusez de choses graves qui méritent au moins une défense, si ce n'est pas ça du garde des Sceaux, c'est celle de l'indépendance de la justice et du fait qu'il n'y a pas de remise en cause de l'État, droit de la démocratie, ben, je sais, je suis en tant que ministre en charge des libertés publiques, c'est moi le ministre en charge, libertés publiques, c'est le garde des Sceaux et en charge, libertés individuelles mais moi je suis en charge des libertés publiques, j'ai même une direction des libertés publiques, qui représentait ici sur ce banc Je suis très attentif comme tout démocrate et tout républicain et je vous dis chiche pour vous montrer qu'il n'y a aucun problème et que c'est une grande partie de ces choses-là sont défectueuses. Comme on dit en bon patois. Et mettons le dans l'amendement. Article 12 du code de procédure pénale absolument inchangée libre choix du service par les magistrats, le fait qu'il n'y a évidemment aucune remise en cause de l'indépendance des magistrats, le fait qu'évidemment il y a pas un policier de PJ qui fera autre chose de fait qu'il y a pas un service qui fait autre chose, vous ne le prenez pas au bon j'en déduis quand même. Monsieur sur soit que la gendarmerie nationale, préfecture de police, vivent dans une. Un état de droit parallèle qui est une forme de dictature qu'on avait pas reconnu depuis 200 ans, et dans ces cas-là, il est urgent de, de, de, de réformer la gendarmerie nationale, la préfecture de police, mais c'est pas ce que propose la haute assemblée, soit que, effectivement, c'était un combat politique parce que les manifestations et je le comprends très bien, mais dans ces cas là, effectivement, je peux plus rapporteur Daubresse a raison comme vous ne prenez pas la balle au bond de la proposition de travail en commun, je suis bien obligé de constater que, moi aussi, je donne un avis défavorable à ces amendements de suppression alors que ma vie à mon avis personnel c'est quand même de travailler ensemble, je ne sais pas, la police judiciaire du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, monsieur le président, et je que je crois profondément, on n'a pas créé la police nationale pour les ministre de l'Intérieur pour les directeurs, quel qu'il soit et pour les policiers, on a créé la police nationale pour protéger les gens et pour lutter con la délinquance quand nous avons un constat que ça ne marche pas, il faut savoir en tirer des conséquences, et même si ça bouge les habitudes,

ne mettons pas de faux arguments sur une réforme. Qui mérite un débat et je crois que je vous montre que nous sommes très convaincus de la réussite de cette réforme donc je constate que vous ne comprenez pas la balle au bond, également défavorable, ça ne retire rien, monsieur le rapporteur, ce que j'ai dit, devant la Haute Assemblée et Monsieur le Président de rende public le rapport commandé par l'administration y compris que les migrations de la justice et de pouvoir en discuter avant, j'en prends mon engagement vont vous avant le moindre changement réglementaire de textes du ministère de l'Intérieur. Merci, monsieur le Ministre, je pense qu'on a épuisé les demandes de prise de parole, donc je vous propose maintenant de passer au hein non voilà monsieur Favreau. Favreau. On sait les choses, je retirerai mon rapport sur l'affirmation que effectivement sur l'obstacle que j'évoquais dans mon amendement, c'est-à-dire sur

pour lequel j'ai été saisi d'une demande de scrutin public, donc par le groupe socialiste, écologiste et républicain concernant l'amendement dix-huit je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est défavorable. Il va être procès de scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos.

de votre accordé par les sénateurs aux groupes politiques et à la présidence, nombre de votants 343 Nombre de suffrages exprimés 335 pour l'adoption 93 contre 242 le Sénat n'a pas adopté. Nous passons à l'amendement 19 pour lequel je suis saisi d'une demande de scrutin public, il retourne il retire non monsieur, vous le retirer. Très bien, donc je le mets aux voix sans scrutin public donc, avec qui un amendement 19 qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour.

Merci madame la présidente, cet amendement porte sur l'alinéa 5 du rapport annexé qui nous dit que la transparence et l'exemplarité de l'action des policiers gendarmes seront mieux garantis, le travail des inspections sera conforté est rendue plus lisible pour les citoyens, et ça fait écho au débat que nous avons eu tout à l'heure sur les nouvelles technologies leur usage dans le cadre de l'action des des forces de sécurité intérieure, nous ne sommes pas par principe hostile à cette technologie, que ce soit la vidéosurveillance, que ce soit un certain nombre d'outils d'Intelligence artificielle et nous pensons même qu'ils peuvent concourir à différents éléments attendus des forces de l'ordre par la société, à savoir la pacification des actions de police administrative, la conduite des enquêtes, la qualité des investigations et le contrôle par les inspections quand le cas échéant, il y a des cas litigieux des sanctions à prendre des allégations de mauvais comportements pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il peut être utile d'ajouter une mention qui permettrait de faire appel à l'Intelligence artificielle, dans ce cas-là, utile, parfois pour la résolution des enquêtes, mais aussi dans toutes les contributions qu'elle peut apporter à la défense des usagers, des forces de police des citoyens dans des cas qui peuvent être problématique, donc voilà le sens de cet amendement que nous proposons d'ajouter au rapport annexé. hein, monsieur le rapporteur. Alors madame la présidente, ben j'ai dit en commission que que l'amendement pour moi était déjà satisfait que comme le ministre avait annoncé, il vient de leur dire qu'il aura une loi sur l'image et notamment dans la perspective des JO, ce serait plutôt là qu'il faudrait trouver sa place maintenant si le ministre nous dit dans son avis qu'il lui est favorable, honnêtement, je ne pense pas trahir l'état d'esprit de la commission, en disant que je laisse la sagesse se faire parce que l'argumentation se Thiam, pour moi c'était satisfait et on pouvait le mettent dans une autre loi, mais il y a pas de difficulté à ce qu'on la mette dans celle-ci. Monsieur le Ministre. à contrôler les actions d'ailleurs, donc moi j'ai j'ai aucun problème, l'Intelligence artificielle, encadrée alors c'est c'est évidemment du déclaratif, donc il faudra regarder endure quand arrivera le texte de loi image mais moi je suis favorable à à la phrase rajoutée par le sénateur du si la commission n'est pas trop vexé de cette position ministérielle. Merci monsieur le ministre, donc on on considère que c'est favorable pour vous monsieur le. Ses sagesse à titre personnel, j'y suis favorable. hé bien, je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 20 qui a reçu une sagesse de la commission, pas vraiment d'avis défavorable du gouvernement plutôt un avis favorable, si j'ai bien compris donc un avis favorable du gouvernement, je le mets aux voix qui est pour.

quoique vous en disiez, ici les citoyens et les citoyennes ne ne sont pas forcément égaux dans leurs rapports avec la police, selon l'endroit où vous vivez ou quel âge vous avez le nombre de contrôles d'identité par exemple est très variable, je vous invite, quand vous rencontrez les scolaire dans un lycée ou dans un collège en fonction des territoires de leur demander qui a déjà été contrôlé, vous verrez, c'est assez variable en fonction de, de là où vous allez, par exemple pour les, les, les jeunes des quartiers populaires, les contrôles ont lieu plusieurs fois par mois pour certains sans aucun motif apparent parfois et quand vous vous faites contrôler de manière répétée pour ne pas dire abusive l'image que vous pouvez avoir de la police et l'État est nécessairement dégradé et donc, nous vous proposons ici que les statistiques de contrôles d'identité soit rendue publique par tranche d'âge et par zone géographique, l'idée est d'objectiver les faits pour arrêter de faire l'autruche et de se renvoyer à des caricatures peut-être que lorsque l'on se rendra compte qu'un jeune vivant à La Courneuve a infiniment plus de chances de se faire contrôler qu'un jeune vivant ici par exemple dans le 6ème arrondissement de Paris, les politiques commenceront à changer les pratiques sur le terrain, elles-mêmes, mais peut-être que ça démontre, à l'inverse et donc seule une transparence les indicateurs objectifs pourra nous éclairer. et qui cite de manière limitative les cas dans lesquels les contrôles peuvent être réalisés il y a pas lieu de rajouter des statistiques et des analyses qui vont une fois de plus encombrait la lourdeur administrative, alors que nous attendons que nos policiers soit maximum sur le terrain défavorable.

que tout le prouve et que tous les témoignages le montre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas lieu d'avoir plus de contrôles d'identité à des endroits en fonction de situations délictueuses ça veut juste dire qu'aujourd'hui il y a aucun critère qui nous permettent d'évaluer si ces contrôles d'identité sont fait effectivement de manière homogène et de manière concrètement concrètement circonstancié, c'est tout, et on demande ça et et et vous le savez très bien, c'est une des raisons aussi de, de, de la perte de confiance de Grenoble de citoyens, c'est pas ce qu'on pense que les contrôles d'identité sont pas fait d'une manière on va dire cohérente entre les différentes couches sociales, raciales et cetera, donc disons-le donc à part non mais, disons-le, c'est la vérité, tout le monde le sait, donc, du moment qu'on le dit. peut-être mais enfin, on utilise les mots qui sont ceux qui viennent et qui sur ceux qui sont utilisés par les gens aussi, donc je vous le dis, les contrôles d'identité sont pas fait de la manière dont il devrait faire et en tout cas, s'il le sent, on aimerait bien effectivement avoir des éléments statistiques, je suis désolé, monsieur le rapporteur, qui nous permettent de le juger, qui nous permettent, qui nous permettent d'en faire une étude, une étude sociologique qui nous permettent d'en tirer des conclusions qui seront valables et qui sera utile à tout le monde, y compris au ministre de l'intérieur et à la police. Monsieur le sénateur, je pense que vos propos ont dépassé votre pensée. Parce que ce que vous dites clairement, c'est que la prise de la République, une partie d'entrer des racistes, puisque si on pas et si on base des contrôles que vous dénoncez sur une forme raciale, c'est donc, effectivement, que l'on distingue selon une race et donc elle serait raciste. Ces propos sont profondément blessant et insultant pour les policiers de la République, vous pas en avoir beaucoup pour imaginer qu'il y a par ailleurs qu'une type de politique, un type de policiers dans la police nationale, c'est une insulte à tous ceux qui, issus eux-mêmes de l'immigration contribuent par leur courage à avoir qu'une couleur de peau, c'est le drapeau bleu, le rouge qui épouse lorsqu'ils acceptent d'être gardien de la paix, vous être gendarme, d'ailleurs, monsieur le sénateur, vous imaginez bien facile votre discours en évoquant jamais le fait que même son et, ça, c'est tout à fait vérifié l'objet d'insultes racistes. aux des policiers mais vous c'est pas drôle du tout, en fin d'accuser les gens de racisme, je pense que vous devriez pas vous amuser de ce point et me fait pas le discours de de des quartiers populaires, j'en viens, j'ai dirigé une commune et cher ami, je pense que vous n'avez aucune leçon d'embourgeoisement de au 6ème arrondissement et vous avez je me semble-t-il, pas d'expérience ni humaine ni politique que j'ai pu avoir dans ma commune, je suis d'ailleurs toujours élu

une liberté de parole dans cet hémicycle, permettez-moi d'défend les policiers, les gendarmes de la République et c'est tout à fait conforme à ce que dit monsieur Mélenchon, de manière générale, il y a bien une filiation politique manifestement et vous êtes bien isolée dans cet hémicycle, puisque je crois qu'un certain nombre de vos collègues de votre formation électorales ont bien pris soin de se démarquer de cette situation, parce que vous savez, monsieur le sénateur, et aujourd'hui ce qui se passe surtout c'est, quand des policiers. Des gendarmes qui ont des couleurs de peau différente de ceux qui le contrôlent, ils sont traités de de harkis qui pourrait d'ailleurs est une insulte, et qui pour moi ne l'est pas, ils se font traiter de traître alors que ils ne font qu'appliquer les lois de la République, en essayant de protéger leurs concitoyens, parce que vous oubliez une chose et c'est pour ça d'ailleurs qu'une grande partie des Français aiment leur police nationale parce que il n'y a pas de désaveu des Français, la police nationale. C'est l'administration la plus aimée de toutes les administrations, mesdames et messieurs les sénateurs, ce qui est sûr, c'est que votre gauche à vous et la quitter, les forces de l'ordre à force de ne pas voir que il protéger les plus populaires d'entre nous et que c'est les populations qui sont les plus pauvres, souvent issus d'immigration qui vivent les difficultés de délinquance au premier parce que les plus riches d'entre nous. Ils ont les moyens d'avoir leurs propres caméras de vidéoprotection leurs propres quartiers parfois leurs propres police et c'est parce que vous avez abandonné les policiers, les gendarmes de la République par c'est beaucoup pour ce discours vous kyste et racialistes. Que vous faites que vous faites un procès, un procès qui est inacceptable, Monsieur le Sénateur, inacceptable et c'est ignorer le droit monsieur le sénateur, c'est ignorer le droit vous qui prônez l'action de la justice que de savoir que vous le dit, monsieur le rapporteur, qu'il n'y a pas un policier de la république il y a pas un gendarme qui fait pas un contrôle entité sans l'autorisation d'un procureur de la République, donc en plus de dire des choses qui sont profondément blessante, vous dites des choses qui reprend proférant fausse. Merci, la parole est à Monsieur Gontard. Monsieur le Ministre, c'est ce que vous avez dit est profondément blessant aussi dans dans votre manière de de l'exprimer et surtout dans cette outrance, vous n'avez pas d'autres éléments, qu'est ce qu'on demande dans cette dans dévaluer d'avoir des statistiques à disposition pour pouvoir discuter et justement pour être dans l'apaisement alors je je comprends bien dans vos propos que l'apaisement, c'est pas quelque chose que qui vous caractérise, c'est bien dommage parce que je pense qu'on a besoin d'apaisement, on a besoin d'apaisement, on a besoin de de rassembler les Français et de leur avec leur police et le fait d'avoir des statistiques, des chiffres, une évaluation précise ça permet ça et c'est certainement pas à travers vos propos, qu'on arrivera justement à apaiser cette cette situation, je le regrette, regrette vivement et je ne comprends pas, en tout cas j'ai pas eu un argument qui ferait que cet amendement ne soit pas votée juste pour avoir des des éléments réels. Merci, cher collègue, alors je vais mettre aux voix l'amendement. 144 qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté alors ben écoutez, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21 heures 30 pour la suite de l'examen de ce texte, la séance est suspendue.